L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finance adoptée par l'Assemblée nationale pour 2020 nous poursuivons l'examen au sein de la seconde partie du projet de loi de finances des différentes missions. Le Sénat va examiner les crédits de la mission cohésion des territoires, l'article 73 à 75 la parole est à monsieur Philippe Dallier, rapporteur spécial de la commission des finances pour les programmes hébergement parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables, aide à l'accès au logement Urbanisme territoires et amélioration de l'habitat et politique de la ville, et tout cela en 7 minutes, monsieur le Président d'Alliés. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le Ministre, mes chers collègues, cette année, la mission cohésion des territoires et doté de 15,2 milliards d'euros en crédits de paiement à nouveau en baisse de 1,2 milliard ou à périmètre constant de 1,5 milliards les dépenses fiscales atteignent un montant équivalent, je vais vous présenter les crédits du programme 177 109 135 et 147 couvrant les champs du logement d'hébergement l'hébergement d'urgence et de la politique de la ville et Bernard Delcros vous présentera les autres programmes. S'agissant du programme 177 les crédits du logement adapté comme de l'hébergement d'urgence sont en hausse de 100 millions mais rappelons que nous venons d'ouvrir 180 millions en elle et faire au titre de 2019 les crédits proposés pour 2020, ce sont donc une nouvelle fois inférieurs à ceux effectivement ouvert pour l'année en cours d'agents dès maintenant, Monsieur le Ministre, qu'il nous faudra y revenir en cours d'année puisque la demande d'asile explose, que les Cada sont toujours saturés et que l'hébergement d'urgence sert malheureusement de palliatif à cette situation. Or dans le même temps, on constate que le logement adapté, malgré la volonté affichée du gouvernement peine à prendre le relais de l'hébergement d'urgence pour sortir les personnes sans abri de la précarité, quant à ceux qui accèdent à un logement autonome, leur nombre ne progresse pas non plus le manque de solutions pérennes conduit donc à une augmentation, apparemment inéluctable de l'hébergement en hôtel, nouveau record en 2019 solutions dont le coût est très élevé, lool Salvan et solutions qui manquent d'accompagnement pour les personnes ainsi héberger un mot également sur le projet pluriannuel de convergence tarifaire des CHRS, donc j'ai soutenu le principe ici depuis plusieurs années, cette convergence tarifaire telle qu'elle est appliquée sur le terrain, monsieur le ministre est mal ressentie car elle ne prend pas en compte la totalité des facteurs objectifs de coûts, notamment celui du foncier qui varient énormément d'une région à l'autre, cette réforme manque donc de lisibilité et apparaît à beaucoup d'acteurs comme une simple recherche d'économie budgétaire, ce qu'elle ne devait pas être à l'origine, les crédits du programme 109 consacré aux aides personnelles au logement, explique quasiment à eux seuls la diminution des moyens de la mission, alors que les crédits était de 15,5 milliards en 2017, ils ne seront plus que de 12 milliards en 2020, soit 3,5 milliards d'économies, la mission cohésion des territoires et le logement en particulier sont donc toujours vos principales sources d'économies budgétaires, cette année la diminution des crédits du programme 109 et de 1,4 milliard cette baisse affectera d'abord pour 1,2 milliard les bénéficiaires des aides personnelles au logement puisque l'article 67 prévoit une revalorisation limitée à 0,3 pourcent bien inférieure à l'inflation bénéficiaire également impactés par la contemporain Lisa Sion des revenus pris en compte dans le calcul des aides si cette réforme est justifiée dans son principe, pour ceux qui seront très au-dessus des plafonds de ressources, sa mise en oeuvre, au risque de susciter de très nombreuses incompréhensions chez ceux dont les revenus varient dans l'année et se situe à la marge du seuil de sortie du dispositif d'un trimestre à l'autre, il pourrait alors perdre le bénéfice de l'APL et peut-être en retrouver le bénéfice le trimestre suivant, je crains, monsieur le Ministre, que nous soyons en train de créer une nouvelle trappes à inactivité, cette mesure de rendement budgétaire va à coup sûr fragilisé les plus précaires, alors pour une entrée en vigueur au 1er janvier prochain il n'est certainement plus possible, eu égard à la complexité technique de la réforme de modifier les règles que vous avez choisi, mais je suis certain que vous serez obligés d'y revenir pour en corriger les effets pour ces populations les plus précaires, la réduction du loyer de solidarité passe quant à elle de 900 millions à 1,3 milliards d'euros et s'accompagne donc d'une diminution des aides versées au locataire toutefois en conséquence de l'accord intervenu le 25 avril 2019 avec le gouvernement, la fameuse clause de revoyure, les bailleurs sociaux bénéficient en 2020 de mesures de compensation, l'article 73 prévoit en effet qu'Action Logement prendra en charge l'an prochain le financement des ailes à la Pierre, pour un montant de 300 millions un mot justement sur Action Logement, qui est très mal récompensé les efforts fournis pour compenser la RLS puisqu'un prélèvement de 500 millions tomber sans aucune concertation, dont la seule finalité est de réduire à due concurrence la subvention d'équilibre versées par l'État au FNAL est prévue à l'article 75 ces dispositions que le gouvernement justifie par la bonne santé de l'organisme pourrait en effet remettre en cause si elle était pérenniser les équilibres issus de la convention quinquennale signée en 2018 et semble ignorer les engagements pris par Action logement pour financer des investissements que l'on peut qualifier de massif à hauteur de 9 milliards d'euros dans le logement social et intermédiaire, mais aussi pour l'ANRU la commission vous proposera donc de supprimer ce prélèvement c'est également sur ce programme 109 que je vous proposerai au nom de la commission de rétablir l'APL accession par un virement de 50 millions monsieur le Ministre, les chiffres du logement pour 2019 ne seront pas bon tout juste médiocre au mieux entre 100 et 100 10 1000 logements sociaux financés et pour la construction privée, nous sommes sur une pente toujours descendante très loin du choc d'offre que vous aviez promis cette mesure comme d'autres, adopté en première partie, et certaines, je l'espère, en seconde partie, pourrait contribuer à redresser ses chiffres, les crédits de paiement du programme 135 sont en augmentation de 65,3 millions mais le programme bénéficie d'un transfert de 60 millions en provenance du programme 174 un bonifié le dispositif Habiter mieux sérénité de l'Lana dans le cas de la réforme du CICE à périmètre constant, les crédits sont donc stable concernant la main 170 1000000 800 ici destinée, on peut penser que cela sera suffisant, mais je sais que certains collègues émettront des doutes à ce sujet, s'agissant enfin du programme 147 relatif à la politique de la ville, je peux surtout faire observer que le NPNRU commence enfin à prendre forme, dans la mesure où près des 2 tiers des projets ont maintenant été validé l'État a promis en 2017 on s'en souvient, une enveloppe de 1 milliard d'euros sur les 10 milliards de crédits budgétaires. Qui est surtout financée par Action Logement et les bailleurs sociaux, cette enveloppe budgétaire sera donc principalement à la charge du prochain quinquennat c'est en effet vers 2000 23 août 2024 que les dépenses atteindront probablement le niveau le plus élevé, notons d'ailleurs que le rapport de gestion de l'ANRU évoque une nécessaire redéfinition des conditions de financement à cet horizon, c'est le risque du fameux retour de la bosse de l'ANRU qu'il conviendra donc d'éviter, en conclusion, si on peut difficilement se satisfaire de crédit qui diminue pour une politique essentiel, aussi bien pour l'économie de notre pays que pour les Français, les crédits relatifs au programme que je viens de présenter correspond en grande partie, pas sur tous les sujets bien sûr à la clause de revoyure signée par le gouvernement et les acteurs du logement social, je vous proposerai donc l'adoption de ces crédits, telle que modifiée par le moment sur l'APL accession, ce qui ne vaut cependant pas Monsieur le Ministre satisfecit sur la politique que vous conduisez qui manifestement ne donne pas les résultats que vous aviez promis.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis particulièrement heureuse de saluer en votre nom, la présence dans notre tribune d'honneur, une délégation de l'Assemblée populaire nationale de Chine, conduite par monsieur John John, membre du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine et vice-président de la commission des Affaires étrangères, cette délégation est reçue par le groupe d'amitié France-Chine présidée par notre collègue Claude rénal, elle est accompagnée en tribunes par notre collègue Catherine Dumas, vice-présidente du groupe d'amitié, le groupe d'amitié organise cet après-midi, la 9ème session de la grande commission parlementaire qui se tient chaque année entre l'Assemblée populaire nationale de Chine et le sénat français cette année, les sessions de travail porteront sur l'ouverture commerciale et le multilatéralisme l'administration numérique et les relations entre l'Union européenne et la Chine en votre nom à tous, permettez-moi, mes chers collègues de souhaiter à nos homologues chinois la plus cordiale bienvenue au Sénat et de fructueux travaux.

La parole est maintenant à Bernard Delcros, rapporteur spécial de la commission des finances pour les programmes impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire et intervention territoriale de l'État pour 7 minutes chers collègues. madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, chers collègues, je vais évoquer donc de programmes, le programme 112 impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire qui progresse en autorisations d'engagement pour 2020 de près de 5 pourcent 4,9 pourcent et qui comporte pour la prochaine année 2 nouveautés. D'abord. La création de l'agence nationale de cohésion des territoires au 1er janvier prochain qui sera doté de près de 50 millions d'euros dans 10 millions fléchés sur l'ingénierie territoriale, ce qui est une inscription que nous soutenons, même si elle nous paraît insuffisante, j'y reviendrai. Il s'agit, à travers cette agence qui va rassembler plusieurs structures existantes de mieux coordonner l'action de l'État auprès des collectivités, avec comme délégués territoriaux, les préfets de chaque département, alors Monsieur le Ministre, cette agence, elle suscite à la fois une forte attente dans les territoires parce qu'il y a un réel besoin. En même temps elle suscite aussi beaucoup d'interrogations et beaucoup de doutes par rapport à sa réelle efficacité voilà quel est aujourd'hui l'état d'esprit des élus dans les territoires et je voudrais, pour ma part insister particulièrement sur le besoin d'ingénierie dans les territoires ruraux parce que les écarts en matière de capacité d'ingénierie sans source d'inégalités territoriales, c'est pourquoi je je proposerai au nom de la commission des finances de rehausser les crédits dédiée à l'ingénierie territoriale à la manière dont ils seront fléchés concrètement dans les territoires au plus près des territoires parce que c'est là que se trouve le besoin d'ingénierie, l'enjeu est, nous semble-t-il important, nous serons donc attentifs à la mise en place de cette agence et il faudra évidemment un petit peu plus tard, évaluer et mesurer le niveau d'efficacité sur le terrain, en tous les cas, nous sommes disposés à donner toutes les chances de réussite à cette agence 2ème nouveauté pour 2020 du programme 112 c'est la mise en place des maisons France service pour beaucoup de MSAP qui seront labellisés en maison France Services 2 millions de crédits y sont consacrés, nous sommes évidemment favorables à l'amélioration de l'homme de service dans les territoires et les Maisons France services peuvent contribuer à apporter des réponses, mais nous veillerons également à la question du financement si de nouvelles missions, notamment pour le compte de l'État par exemple à travers la réforme des trésoreries devait être confiée à ces maisons France service évidemment le soutien financier de l'État devra être au rendez-vous, nous suivrons donc concrètement cette mise en place et là aussi il faudra évaluer pour voir comment ces Maisons France services permettent d'améliorer l'offre de service dans les territoires, quelle valeur ajoutée et surtout les évolutions en matière de besoins de financement, notamment dans le cas où il y aurait des charges transférées je voudrais évoquer 3 autres sujets du programme 112 premièrement la quasi-disparition de la prime à l'aménagement du territoire, cette aide directe versée aux entreprises pour soutenir l'emploi dans les territoires ruraux, vous proposez une nouvelle baisse de 4 millions d'euros que je trouve parfaitement inopportune, d'abord parce qu'il n'y a pas d'enjeu financier. Nous parlons de 4 millions d'euros à l'échelle nationale. Et deuxièmement parce que l'effet levier. De cette prime à l'aménagement du territoire a été démontrée, elle a fait l'objet d'une évaluation en 2017 et je vous livre la conclusion de cette évaluation, la prime à l'aménagement du territoire constitue un outil solide et pertinent pour soutenir le développement économique des territoires fragiles dans ce contexte, je vous le dis la baisse proposée est incompréhensible et nous proposerons des amendements pour revenir au niveau de 2019 2ème sujet et l'avenir des zones de révélations rural puisque les dispositifs fiscaux qui les accompagne, relève du programme 112 les ZRR ont fait leurs preuves dans les territoires ruraux avec mes collègues Frédérique Espagnac et Rémy Pointereau, nous avons présenté un rapport et fait de nouvelles propositions pour des dispositions plus ciblées, prenant mieux en compte les niveaux de fragilité des territoires, mais dans l'attente de la mise en place des dispositifs, nous proposerons un amendement de prorogation du dispositif jusqu'en 2021 enfin l'avenir des outils de contractualisation entre l'État et les collectivités locales qui devrait faire l'objet d'une remise à plat au cours de l'année 2020 avec les CPER qui sont dotés de 123 millions d'euros et qui vont être renégociés, nous considérons que la nouvelle génération de contrat de plan État-Région devrait systématiquement intégré 3 volets : l'offre de soins. Parce que c'est un enjeu majeur des territoires dans quasiment tous les territoires, la question de l'agriculture et de la forêt et leur nécessaire adaptation au nouveau contexte climatique et troisièmement rechercher une meilleure, une meilleure coordination entre l'État et les régions pour renforcer la solidarité infra-régionale, les contrats de ruralité. Je me réjouis que la principale proposition que j'avais faite dans le rapport que j'ai présenté en juillet dernier, était retenue et qu'une 2ème génération de contrats de ruralité soit envisagée en effet la dilution de ces contrats dans son contrat unique de cohésion territoriale comme prévu initialement, peser, peser un risque de dilution et de non prise en compte réelle des enjeux ruraux dans la politique contractuelle de l'État, enfin, l'épave de développement territorial qui ont été mis en place en 2019 dans en ce territoire et doté de 11 millions d'euros pour 2020 devront trouver je pense une déclinaison et une cohérence sur l'ensemble du territoire national. Concernant le programme 162 Interventions territoriales de l'État, 4 actions déjà inscrite en 2019 sont reconduites l'action en faveur de la Corse, le plan littoral 21 pour sa 2ème année, le plan gouvernemental en faveur du Marais Poitevin avec seulement des crédits de paiement puisqu'il est destiné à se à se terminer et enfin le plan chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, où là, nous proposerons une légère augmentation des crédits, de manière à répondre aux enjeux sanitaires de ce de ces territoires qui sont extrêmement importants, enfin, de nouvelles actions sont ouvertes, l'action 10 avec le fonds interministériel de temps forts, transformation de la Guyane et la reconquête de la qualité des cours d'eau en Pays de Loire. En conclusion, je voudrais rappeler une fois de plus, qu'il me semble que la politique d'aménagement de territoire de l'État et trop peu lisible et qu'elle est dispersée sur 12 missions et 29 programmes ce qui évidemment fait perdre toute sa visibilité, je pense que tout le monde aurait à gagner d'une clarification, les élus et les acteurs locaux et au bout du compte, les territoires gagnerait à une politique nationale de développement territorial plus cohérente, plus stable et plus durable, plus lisible, mieux articuler peut-être Monsieur le Ministre, pourrions-nous confier cette mission à l'agence nationale de cohésion des territoires en tous les cas je vous soumets cette proposition, mes chers collègues, je vous propose, avec la commission de finances de voter les crédits correspondants à cette mission pour ce qui concerne les programmes 112 et 162 je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Madame Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques pour les programmes hébergement parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables, aide à l'accès au logement et Urbanisme territoires et amélioration de l'habitat pour 3 minutes. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, pour la 3ème année consécutive, les crédits du logement diminue encore à hauteur de 1,4 milliards d'économies, la commission des affaires économiques a décidé décidé tout néanmoins de donner un avis favorable à l'adoption de ces crédits pour 3 raisons : le respect de la clause de revoyure avec le mouvement HLM, la mise en oeuvre en 2020 des APL en temps réel et la poursuite des créations de places d'hébergement en faveur des personnes vulnérables, le projet de loi de finances pour 2020 mettent en oeuvre la clause de revoyure l'impact de la RLS hé bien ramené de 1,5 à 1,3 milliards d'euros dans un esprit de responsabilité, la commission a souhaité en donner acte au gouvernement, mais vous le savez nous estimant qu'elle ne va pas assez loin, par exemple en termes de TVA réduite sur le logement social, nous regrettons aussi que l'État est repris ce qu'il avait donné, en ponctionnant Action logement de 500 millions d'euros au delà de ce budget la santé financière des bailleurs reste un sujet d'inquiétude majeure, le RU à et l'avenir de la RLS sont des épées de Damoclès alors que l'on voit ces derniers jours, fleurir les rapports sur le milliard d'économie que l'on pourrait encore faire chez les bailleurs sociaux ou l'entrée d'acteurs privés, comme vous le savez, par rapport aux dépenses tendancielle, ce sont 7 milliards d'économies qui seront faites entre 2016 et 2020, il serait temps, Monsieur le Ministre, de dire Stop à Bercy, le logement social n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue pour des milliers de nos concitoyens, quand vous dites que vous voulez préserver le modèle français, je veux bien vous croire, mais encore faut-il vraiment passer de la parole aux actes, la commission a aussi souhaité donner son accord de principe sur la réforme du calcul et du versement des APL en temps réel, cependant, même si les paramètres sont inchangés, les simulations manque et toutes les craintes ne sont pas levées, vous aurez peut-être là-dessus monsieur le ministre, des éléments nouveaux à nous apporter la Commission a voulu également apporté son soutien à l'effort de création des places pour l'hébergement des personnes vulnérables, nous avons là aussi des motifs d'insatisfaction, les nuitées hôtelières ne cesse d'augmenter et sont à un niveau historiquement élevé, selon les associations, le nombre des sans-abri aurait augmenté de plus de 50 pourcent depuis 2012 dans notre pays, enfin, nous souhaitons véritablement que l'accent soit mis sur l'accompagnement social indispensable à la réinsertion, je voudrais enfin dire un mot du budget de l'ANA qui se trouve sous tension en raison plus particulièrement du succès du plan chaudière, un besoin de financement de 90 millions d'euros sur 3 ans seraient identifiés aurait voulu déplafonner les quotas carbone mais un tels amendements aurait été irrecevable, nous vous demandons donc Monsieur le Ministre d'aborder son budget, sinon il y en aura pas assez de financements pour tous les programmes existants et encore moins pour ceux à venir, comme par exemple la rénovation des centres bourgs ruraux, je vous remercie, merci. La parole est maintenant à Madame Annie Guillemot rapporteur. Pour avis de la commission des affaires économiques pour le programme politique de la ville. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, Jean-Louis Borloo avait intitulé son rapport vivre ensemble pour une rue. Conciliation nationale il il voyait le danger de la montée, parfois violentes des revendications sociales et des expressions identitaires, il écrivait : si on ajoute les territoires ruraux délaissé et certaines villes ou bassins en grave des prix, ce seront plus de 10 millions de compatriotes qui sont éloignés du moteur de la réussite, et plus loin, à défaut, ferme trop loin des yeux le recroquevillée identitaire et le repli communautaire si trop de nos concitoyens ont le sentiment de ne pas participer au rêve républicain, cela m'a fait penser à la phrase Monsieur le Ministre, au 17ème siècle, Miron, conseiller du roi, mettez Henri IV en garde en ces termes : il est dangereux dans une cité d'avoir les maigres et les pauvres, d'un côté, les riches et les dodus, de l'autre, cela se pourrait cirque des balles Vince ricocher à votre couronne aujourd'hui c'est vrai que on craint l'explosion, même si ce ne sont pas des balles, mais ce sont les émeutes et je crois qu'il faut vraiment que vous soyez attentifs à la situation de nombreux de nos quartiers, selon moi, le budget que nous examinons n'est pas à la hauteur de cet enjeu, naturellement, il y a dans cette enveloppe budgétaire largement reconduite des motifs de satisfaction, comme le bon déploiement des postes sont JEP ou la poursuite du développement des écoles de la 2ème chance mais j'ai 2 sujets d'inquiétude au regard de ce que nous vivons dans les quartiers, le sort de l'Epareca et celui de l'ANRU je souhaite tout d'abord vous sensibiliser aux conséquences de l'absorption des cas au sein de l'ANC était à partir du 1er janvier vous nous dites, Monsieur le Ministre, que c'est l'Epareca qui insufflera à la nouvelle agence sa culture du terrain du projet et du monde économique, je voudrais y croire, le problème c'est qu'on a amputé les barricades, une de ses 2 jambes, les professionnels du commerce, ils ne seront pas représentés au conseil d'administration de l'ANC était et à ma connaissance, aucune procédure n'est prévu pour les inclure dans le processus de décision, or je peux témoigner en tant qu'ancienne présidente de l'Epareca, mais aussi avec toute mon expérience des quartiers que les professionnels ont toujours été précieux et participez étroitement aux décisions pour sélectionner les projets les plus pertinents si on n'y porte pas remède on aura cassé un outil qui fonctionnait et qui fonctionnait bien et ce sont les maires qui se retrouveront en première ligne sans aucun appui je souhaite ensuite aborder la situation de l'ANRU en juillet 2018, le président de la République a réaffirmé l'engagement de l'État d'apporter un milliard d'euros dans le cas du doublement du NPNRU, il a aussi promis 200 millions d'euros durant son quinquennat l'ANRU s'est remis à travailler sur les 450 quartiers concernés 329 ont vu leurs projets validés, je reconnais volontiers le travail qui a été accompli pour rattraper le temps perdu cependant très peu de choses auront été concrètement fait dans les quartiers pendant ce mandat municipal, alors que la situation est très préoccupante, je le disais dans ce contexte, je trouve grave que l'État ne respecte pas son engagement de financement de l'ANRU cette année l'État aurait dû inscrire 35 millions d'euros, seuls 25 sont au rendez-vous, à ce rythme, ce sont 2 quinquennats qu'il faudra pour tenir la promesse initiale, au contraire, l'État devrait être moteur et engager les programmes par avance pour rénover, écoles et collèges par exemple sous le bénéfice de ses observations, la majorité de la commission des affaires économiques, a décidé de donner un avis favorable au crédit politique de la ville. La parole est maintenant à monsieur Jean-Marie Morisset. Rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales pour les. Programme hébergement parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables pour 3 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des Affaires sociales Examen des crédits du programme 177 qui finance l'hébergement des personnes à la rue et et leur accompagnement vers le logement, la sous-budgétisation du programme se poursuit d'année en année et augmenterait même en 2019, l'écart entre les crédits ouverts pour cette année et la prévision d'exécuter d'exécution atteindrait 227 millions d'euros, dont 178 millions d'euros demandés dans le cas de la loi de finances rectificatif pour 2019 cette dynamique des dépenses a permis d'accroître le parc d'hébergement qui atteint 146000 places d'accueil, sans que la demande ne parviennent à être totalement satisfaite de nombreuses personnes demeurent à la rue dans les stations de métro, voire dans certains hôpitaux parisiens et dans ce contexte, le recours aux nuitées d'hôtel augmente inexorablement malgré la volonté de les limiter et dépasse aujourd'hui les 48000 places pour 2020 les crédits augmentent de 5,3 pourcent mais demeure inférieur à l'exécution 2018 et à la prévision d'exécution pour 2019, il pourrait donc s'avérer encore insuffisant ce budget 2020, met l'accent sur le logement adapté conformément aux objectifs du plan logement d'abord les crédits dédiés aux pensions de famille augmente de 11 pourcent et ce pour l'intermédiation locative de 23 pourcent, ce qui devrait permette d'accompagner la montée en charge de ce dispositif je mentionnerait 2 points d'alerte sur le logement adapté d'une part, le forfait de 16 euros par jour et par place pour financer les pensions de famille inchangé depuis 10 ans devrait être revalorisé pour faciliter leur développement, d'autre part, le budget dédié à l'aide à la gestion locative sociale est entamée chaque année par des redéploiements par des redéploiements de crédits au profit d'hébergement d'urgence, ce qui ne permet pas de soutenir correctement les résidences sociales concernant l'hébergement d'urgence et d'insertion des montants prévus augmentent plus modérément, il pourrait être insuffisant pour les places d'urgence compte tenu des 14000 places qui seraient ouvertes cet hiver concernant le CHRS les mesures de convergence tarifaire sont à poursuivre avec précaution afin que leur mission d'accompagnement ne soient pas mis en difficulté la contractualisation avec les CHRS doit être appliqué avec la même vigilance pour fixer des objectifs cohérents avec la spécificité des publics accueillis au total des efforts engagés sont à poursuivent pour consigne concilier l'inconditionnalité de l'accueil et la maîtrise des financements, la réussite du plan logement d'abord que nous soutenons sera conditionné au maintien d'une offre d'hébergement et d'insertion à la hauteur des besoins et au renforcement des moyens d'accéder au logement adapté ou en conséquence, la commission des affaires sociales a donné un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission, je vous en. Merci, La parole est maintenant à Louis-Jean de Nicolaï, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour 3 minutes. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, a émis un avis d'abstention à l'adoption des crédits des programmes 162 et 112 de la mission cohésion des territoires et des crédits du compte d'affectation spéciale consacrée au financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale du projet de loi de finances pour 2020, plusieurs raisons justifient ce soit d'abord, la Commission a salué l'inscription d'une ligne de 10 millions d'euros dédiée au soutien à la conception technique et financière des projets des collectivités territoriales dans la subvention qui sera versé à l'Agence nationale de la cohésion des territoires car c'est un point crucial pour soutenir les territoires les plus frappe les plus fragiles, naturellement j'apporterai mon soutien à la proposition de la commission des finances de relever de 10 millions d'euros, l'inscription budgétaire au bénéfice des crédits territoriaux. De la même manière, la commission est satisfaite de la première priorité accordée au développement de l'accessibilité, l'accessibilité des services publics, avec un budget en hausse de près de 3 millions d'euros pour accompagner le déploiement des Maisons France service ensuite les moyens dédiés au plan de lutte contre le chlordécone se renforcer en 2020 et c'est un événement positif, même si ce ne sont pas encore à la hauteur de la réalité de ce scandale environnemental et de ses conséquences sanitaires préoccupante toutefois 2 éléments principaux ont retenu l'attention de la Commission et ont conduit à modérer l'enthousiasme si je puis dire de pour ce budget 2020, il en va ainsi de la baisse continue dont sont victimes les crédits dédiés à la prime d'aménagement du territoire, le PLF ne contient que 6 millions d'euros en autorisations d'engagement pour la prime, ce qui est très insuffisant pour accompagner les territoires qui subissent encore les conséquences de la crise de 2008 et sont confrontés à la nécessité de renforcer leur attractivité à l'égard des investissements étrangers sur ce point je rejoins le rapporteur spécial Bernard Delcros, et nous avons chacun déposé un amendement pour augmenter les autorisations d'engagement dédié à la pâte à hauteur de 10 millions d'euros, comme en 2019 par ailleurs les autorisations d'engagement du programme 112 sont inférieurs de 20 pourcent au crédit de paiement de plusieurs actions et qui ont fait l'objet de transfert sortant de ces dernières années, ce qui témoigne d'une dynamique globale de décroissance et c'est une source d'inquiétude, alors que les politiques dédiées à l'aménagement des territoires sont plus que jamais nécessaire face face aux fractures territoriales, sociales numérique dans la et dans la mobilité, au-delà, je souhaite appuyer la démarche de mes collègues, Rémy Pointereau : Bernard Delcros et Frédérique Espagnac concernant les ZRR, dans le prolongement de leur récent rapport réalisé au nom de la commission de l'aménagement du territoire et de la commission des finances, la prorogation jusqu'en décembre 2021 du bénéfice de classement pour les 4000 communes sortantes à l'été 2020 et la progrès prorogation des et des exonérations fiscales active en ZRR sont une nécessité pour pouvoir conduire le travail souhaitée par le 1er ministre sur une nouvelle géographie prioritaire de la ruralité dans de bonnes conditions je conclurai mes chers collègues, mon intervention par 2 questions : d'abord, Monsieur le Ministre, qu'elle sort réservez-vous à la prime d'aménagement du territoire, à terme, ensuite, quels sont les prix en priorité d'action de l'ANC était pour 2020, je vous en remercie. Dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribués à chaque groupe. Pour chaque discussion qu'on prend le temps d'intervention général et celui de l'explication de texte, par ailleurs, le gouvernement dispose au total de 20 minutes pour intervenir, la parole est maintenant à monsieur Jean-Yves Roux pour le groupe RDSE. Ce pour 6 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le budget cohésion des territoires se caractérise par une forte hétérogénéité de ces programmes paradoxalement le principe même de fongibilité de ce budget ne participe pas tout à fait à cette cohésion tant attendu dès lors qu'il s'agit pour amender d'enlever à la politique de l'aide au logement pour donner au développement rural et vice versa, paradoxalement, ainsi le transfert cette année dans le budget, relations avec les collectivités locales des contrats de ruralité n'ajoute pas forcément à la cohérence et la lisibilité des dispositifs de soutien aux politiques territoriales telles que les élus l'appréhende au quotidien, sans doute, monsieur le ministre, il y a-t-il matière à gagner incohérences à périmètre constant, l'ensemble de la mission est en baisse de 1,5 milliard d'euros, la mission a fait l'objet de transfert de crédits, je pense au transfert vers le programme Habiter mieux ainsi que le transfert des pôles de compétitivité, ainsi que des compensations budgétaires comme la baisse des cotisations au final le fait saillant pour ce budget 2020, hé bien la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ce contexte général poser mes chers collègues, vous me permettrez tout d'abord plusieurs remarques et questions sur le 1er poste budgétaire des ménages, le logement et l'aide au logement, je salue l'augmentation des crédits dédiés à l'hébergement d'urgence, même s'il faut rappeler, car la matière, il y a un cap à tenir et un objectif exigeant et Hummer, la progression en nuitées hôtelières constater une fois de plus n'est satisfaisante pour personne aussi la diminution des nuitées dites sociales peu propice à la réinsertion, très coûteuses et sujet sa spéculation au profil d'un hébergement de plus longue durée doit être un objectif majeur à poursuivre, j'en viens à 2 questions plus conjoncturel, tout d'abord, alors que la construction de logements est en baisse depuis 3 ans que cette situation génère une tension sociale je vous interroge monsieur le ministre, sur les menaces de ralentissement de la construction de logements sociaux et intermédiaires due au remplacement de la taxe d'habitation départ la part départementale de la taxe sur les propriétés bâties les élus doivent pouvoir anticiper aussi Monsieur le Ministre : quelles sont les simulations du ministère à la matière 2ème dans le droit fil du rapport que nous avons rédigé avec mon collègue Ronan Dantec, notre pays pays subit les effets du réchauffement climatique, parfois de manière particulièrement dramatiques comme dans le Sud-Est, notamment il convient à la douter de favoriser dès maintenant des modes de construction qui permettront de tenir face à des périodes de canicule répétées, mais aussi dans les zones inondables, d'être adapté dans la mesure du possible, la décrue et précipitation destructif, là encore, le soutien aux politiques d'aide au logement devront aussi tenir compte de ces priorités, mes chers collègues, j'en viens, la nouveauté de ce budget, à ce titre, vous vous permettez de m'attarder sur le sort réservé au programme 112 impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire, les crédits de ce programme s'élève à 245 millions en crédits de paiement, ce qui correspond à une légère augmentation de 20 1 8 pourcent des crédits de paiement due pour l'essentiel à la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires en jeu au 1er janvier 2020, je dois vous dire combien nous sommes fiers que cette agence, fruit d'une pro position de lois et de la détermination du groupe RDSE voit le jour dans quelques semaines, vous comprendrez aisément que nous sommes particulièrement attentifs à ce que sa création sous sur les meilleurs auspices et puis être directement identifiées par les élus locaux, notamment ceux de la ruralité, cette année 2020 serait en effet une année d'installation des nouveaux exécutifs municipaux intercommunaux, mais aussi une année de lancement des programmes d'investissement local. Il nous paraît opportun que les nouvelles équipes qui vont diriger les exécutifs municipaux puissent bénéficier d'une agence de cohésion des territoires parfaitement opérationnel à leurs côtés, avec des moyens dédiés et surtout la capacité d'ingénierie suffisante nécessaire à l'impulsion de ce nouveau projet, il faut ainsi rappelé que la première année est traditionnellement une année où les investissements sont plus faibles et qu'il convient de leur donner toutes les chances de réussir, nous souhaitons, de ce fait veiller dès maintenant à ce que les élus de petites communes soit directement et immédiatement bénéficiaires cette nouvelle agence une campagne d'information aux nouveaux élus nous paraît adapté concernant les moyens consacrés à ces objectifs, le 1er budget de l'ANC, ONCT est ainsi abondé par une subvention de 49,7 millions d'euros dans 10 millions d'euros pour le soutien à l'ingénierie à destination des collectivités, elle disposera de 331 équivalents temps plein qu'en 2020, même si les recettes commerciales de l'Epareca qui intègre l'agence compléteront également le dispositif financier, nous ne pensons pas que la subvention initiale prévue sera suffisante, il faut en effet rappeler que 2020 correspond aussi à l'objectif du bon débit pour tous, pour lequel elle s'était via l'intégration de l'agence numérique sera bien utile 2020 verra également la naissance dans chaque canton de mes France ce service 20 coïncide également à la fin des programmes de subventions européen leader dont l'instruction va s'intensifier en fait, l'ANC était sera chargé de la mise en oeuvre des contrats de cohésion territoriale 11 Pacte de développement territorial dans une logique de différenciation selon les territoires ont été signés en 2019 associant l'État, les collectivités, l'ADEME, l'ANRU le CEREMA ainsi que les acteurs économiques et sociaux si la raison pour laquelle on en sous-groupes présentent des amendements permettant d'augmenter dès maintenant les crédits pour 2020 destiné au lancement de la TNT dans un contexte de gouvernement des équipes municipales et d'objectifs internes en matière d'aménagement du territoire, nous espérons, monsieur le ministre, que vous accorderez à ces amendements une attention bienveillante, comme tout ce que nous présenterons pour soutenir les projets de nouvelles équipes municipales, nos élus mérite mes chers collègues, d'être pleinement soutenus par l'Inde s'était et ce dès début le début de leur mandat, je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Françoise Cartron, pour le groupe LaREM pour 7 minutes. Madame la présidente, monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs, monsieur le Ministre, mes chers collègues, cela a été rappelé en introduction, en 2020, l'ensemble des crédits concourant à la politique d'aménagement du territoire représenteront 8,5 milliards d'euros, un budget répartis dans près de 30 programme politique transversale, si l'année je ne reviens pas dans cette discussion sur l'ensemble des points abordés précédemment mais sur 3 d'entre eux, plus spécifiquement sur le programme 112 tout d'abord, une hausse de près de 5 pourcent en autorisations d'engagement est à souligner, pour 2020 les crédits du programme 112 qui se nomme impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire s'élève en effet à 209 millions d'euros en autorisations d'engagement et 245 millions d'euros en crédits de paiement ce budget viendra porter tout d'abord, le déploiement de l'agence nationale de cohésion des territoires précédemment doté d'une subvention de 50 millions d'euros, cette nouvelle instance, que nous avons ici voté, instance créée à la demande des élus locaux sera composée de 331 personnel en équivalent temps plein, avec une tutelle assurée par la direction générale des collectivités locales si ces crédits correspondent en partie à ceux déjà affectés par le passé aux entités qui fusionnent dans cette agence, une ligne de crédit de 10 millions d'euros a été ouverte en plus pour financer l'ingénierie territoriale que cette structure apportera aux collectivités, et tout particulièrement communes rurales, une très bonne chose donc utile à tous les ministères et à toutes les collectivités, l'objectif, améliorer la coordination de l'action territoriale de l'État et de ses établissements publics nationaux afin d'accompagner l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements dans la définition de leurs plus de leur projet et dans la réalisation, ces projets aujourd'hui sont parfois en latence et il porte sur l'accès aux soins, l'accès au service public, l'offre de logements, le développement des mobilités et le développement économique durable, ces moyens se concentreront sur les territoires demandeurs qui en ont le plus besoin et notamment, je l'ai dit, en zone rurale, sur le programme 112 toujours la hausse des crédits correspond à un effort de près de 3 millions d'euros et de soutien au développement des maisons France service à compter du 1er janvier prochain notre rapporteur, a rappelé les chiffres, 1344 maisons de service public, M. P. dont la généralisation a été actée en 2013 sont d'ores et déjà implantés, mais un rapport 2019 de la Cour des comptes est venu dresser un double constat : d'abord une forte hétérogénéité selon les territoires dans la qualité des services et la nécessité de revoir le schéma de financement de ces structures, c'est pourquoi le 25 avril dernier le président de la République a a annoncé son intention de créer ce nouveau Label baptisé Maison France Services et de voir chaque canton couverts par une telle structure d'ici la fin du quinquennat. Soit l'équivalent de 2000, mais en France, ce service au total d'ici 2022 avec une règle simple : être accessibles pour chaque concitoyen à moins de 30 minutes du domicile. Le 1er ministre a précisé courant novembre, la localisation des 460 premières maisons qui bénéficient de ce nouveau Label et à l'issue du 4ème comité interministériel de la transformation publique pour mon département, ce sont les communes girondines de Sainte Foy la Grande Captieux que doc Rozan Pessac Lacanau Sainte-Eulalie qui ont obtenu cette reconnaissance, elles ont été les premières à se manifester, et aujourd'hui, elles ont donc ce Label, le mouvement, bien sûr, de labellisation va se poursuivre pour toutes les autres, d'autres qui seront bientôt reconnus, avec toujours ce même objectif : permettre de simplifier et d'améliorer la relation des usagers au service public et ce au plus près pour 2020 les crédits du programme 162 qui se dénomme Interventions territoriales de l'État sont également en forte augmentation, cela résulte en 1er lieu de la création d'une nouvelle action dédiée au fonds interministériel pour la transformation de la Guyane, notre groupe et en particulier les sénateurs du département concerné, Antoine Karam et Georges Patient l'fortement se sont mobilisés et aujourd'hui s'en félicitent, enfin, en tant que membre de la commission départementale de la répartition des crédits de la des de la dotation d'équipement appelé des de DETR et parce que certaines approximations circulent souvent, il est à noter que la DETR et la dotation de soutien à l'investissement local déciles ne baissent en aucun cas en 2020 et sont maintenus à leur niveau,

en particulier, elles accompagnent toutes ces communes et les communes les plus en difficulté pour répondre à cette promesse et à cette demande faite par le ministère de l'Éducation nationale, de la scolarisation des enfants dès 3 ans et du dédoublement de certaines du dédoublement de certaines classes de CP la DETR atteindra 1 milliard d'euros et la déciles 570 millions d'euros, cela s'inscrit en soutien à cette cohésion des territoires et ses lignes budgétaires d'ailleurs seront discutées ici même demain, alors que le texte, engagement et proximité est actuellement en navette parlementaire que le projet de loi 3D sera présenté au printemps au printemps prochain, c'est toute une réflexion globale qui s'est enclenché de financement en faveur de la cohésion et de l'égalité des territoires, tant attendu, mon groupe s'en félicite et votera donc pour ces crédits merci.

Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, pour la 3ème année le budget du logement va baisser et pas une petite baisse l'an dernier, il a baissé de 8,3 pourcent et cette année 7 9 en 3 ans, en tout cas depuis que le nouveau gouvernement est arrivé il y a une perte de 3,3 milliards qui ont été ponctionnés sur ce budget, or c'est un des Budgets les plus importants pour la nation et pour nos concitoyens, pour leurs conditions de vie pour le pouvoir d'achat car ça pèse lourd dans les dépenses des Français, et particulièrement des familles moyennes et modestes, deuxièmement parce que le droit au logement doit être garantie, on ne trouve pas assez de logements abordables, le logement est trop cher le logement social, trop rare. Il en va du pacte républicain, parce que si nous voyons augmenter le nom du mal-logement si nous voyons se maintenir ou s'accroître l'habitat indigne, l'on nous sommes incapables de faire vivre la mixité sociale et de lutter conte la ségrégation urbaine, c'est le pacte républicain qui est menacé. Troisièmement, le logement, crée de l'emploi et de manière importante sur l'ensemble du territoire et quatrièmement, il est un des piliers d'une politique du pour répondre au changement climatique et à l'urgence écologiste alors considéré que ce budget devienne l'un des plus gros contributeur aux économies qui sont exigées de l'État n'est pas acceptable car nous ratons des échéances majeures pour notre avenir et le quotidien de nos concitoyens, votre budget, monsieur le Ministre, n'est ni raisonnable ni juste ni écologiste nous voterons donc contre ce budget. D'abord je voudrais parler du pouvoir d'achat. Qui est largement ponctionné par le logement, vous savez que les Français dépensent 24,3 pourcent en moyenne de leurs revenus pour les dépenses de logement ça a augmenté en 2 ans de 1,1 pourcent alors on peut faire toutes les aides, les primes, etc, pour soutenir le pouvoir d'achat, c'est ce qui est donné, d'un côté et prix de l'autre, nos concitoyens le ressentent bien leur pouvoir d'achat ne s'améliore pas, deuxièmement, il y a de grandes disparités 48 pourcent des familles modestes de ce pays consacrent plus d'un tiers de leurs dépenses pour le logement et c'est justement ces catégories modestes que vous êtes que vous ponctionner en particulier avec l'alors on nous avait dit : le prix du logement va baisser Macron dans sa vision libérale nous vous annoncer le choc de l'offre et croyant spontanément, ça ferait baisser les prix, hé ben nous avons pas le choc de l'homme mais un conte choc bus, les mises en chantier, comme les permis de construire ont baissé en 2018, 4 5 pourcent pour les mises en chantier et 8,6 pour les les permis de construire, et ça continue la même tendance en 2019. Alors qu'en réalité vous n'avez pas voulu engager la régulation qui s'imposent des prix et nous regrettons toujours que l'encadrement des loyers dans les zones urbaines denses et dans les secteurs en tension ne soient pas mises en oeuvre, car ça ne fait qu'accroître les difficultés, deuxièmement, non, non seulement vous ne pas mais vous laisser filer les prix de l'immobilier puisque les prix de l'immobilier explose encore 3,2 pourcent de hausse cette année, contre 1,8 pourcent d'inflation et donc ça ne peut qu'accroître les difficultés à construire et à payer des prix raisonnables pour se loger, alors le comble est atteint, c'est que devant cette réalité, on pourrait penser que vous souteniez l'APL les aides personnalisées pour les personnes modestes en 3 ans, il y aura une baisse des APL de 7 7 milliards d'euros pris sur les plus démunis, les plus modestes et les les catégories moyennes, il y a eu la la PL : les 5 euros il y a eu le nom d'indexation, le gel de l'APL, puis une augmentation tellement modeste 0 3 qui est à des années-lumière de l'inflation, 3 fois moins que l'inflation et vous ajoutez à cela mette en oeuvre la ce qu'on appelle la contemporanéité, c'est-à-dire la le versement actualisé Direct en temps réel des appels vous allez ponctionner 1,3 milliards d'euros sur ces APL alors Madame la rapporteure Mesdames Estrosi Sassone a raison de dire, ça peut être une réforme de bon sens, sauf que là, c'est une vraie, une réforme de bon sens et de mauvaises intentions, parce que l'intention, c'est de prendre 1,3 milliard sur les APL, alors qu'il aurait fallu les actualiser et, en particulier mieux régler le problème des jeunes dont on sait que ça va être un de ceux qui vont avoir le plus de difficultés il y a une menace avec le alors vous savez quand on entend universel de la part du gouvernement, Monsieur le Ministre, moi ça me fait peur, ça me rappelle les retraites universel c'est c'est tellement universelle qu'on met la même somme pour tout ça a baissé pour tout le monde hé ben c'est la même chose un peu pour le RU puisque vous voulez à à à à prestations constante, avoir le même un plus de bénéficiaires pour le non recours et vous voulez mettent les allocations logement, or aujourd'hui, il y a 6,6 millions de Français qui touchent les allocations logement et parmi eux, près de 3 millions qui ne touchent rien d'autre que l'APL et pourquoi, parce que la paix, elle n'est pas un revenu de transfert ou à revenu de substitution a minima social, c'est une aide pour garantir le droit au logement, donc, notre groupe est opposé à la mise en oeuvre du terroir, mais les menaces ne sont pas seulement pour l'APL, elles le sont pour le logement social, alors certes nous approuvons le fait que le budget inclut la fameuse clause de revoyure mais le demeure, simplement il y a des compensations et du nouveau vous félicitons du vote du Sénat d'élargir la TVA à 5 5 à l'ensemble du logement plus logement social d'ailleurs Monsieur Dallier il y a pris une part importante de conclure, d'ailleurs, donc je veux dire que le logement social est aussi dans l'oeil du cyclone, il y a des menaces de privatisation à terme de cela, je veux dire aussi que les crédits de la nation, à des années lumières de ce qu'il a besoin pour la transition énergétique, je veux dire aussi que, par ailleurs, l'habitat indigne, voit ses crédits baisser après l'affaire de Marseille il y a expliqué : il faudrait pour l'hébergement d'urgence un plan de d'urgence, pas seulement d'urgence mais une programmation pluriannuelle pour prendre à bras-le-corps ces problèmes, il en va de notre avenir, républicain, il faut une volonté politique et un budget à la hauteur, il n'y a ni l'un ni l'autre, nous voterons contre ce budget. Merci. La parole est maintenant à monsieur Jean-Pierre de. Pour le groupe, les indépendants et vous avez 6 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la France est un pays riche de ces territoires, leur diversité et son atout sa particularité et sa spécificité, assurer la cohésion des territoires de notre pays est essentiel dans mon département : le Nord je crois indispensable dialogue et la cohésion entre la métropole lilloise et territoires ruraux qui la Borde entre les aires urbaines de Dunkerque, Valenciennes, Douai et les zones plus rurales de l'Avesnois des Flandres du Cambrésis cette cohésion a pour objectif de réduire les inégalités territoriales de réduire aussi les fractures sociales, mais elle a surtout pour objectif d'instaurer un équilibre dans le nécessaire vivre ensemble cher à notre pays la mission cohésion des territoires et ces programmes que nous examinons aujourd'hui, ce sont des outils indispensables à la mise en place d'une politique ambitieuse sur ce sujet, cette politique doit mettre en oeuvre et des évolutions d'aménagement équilibré de notre territoire, elle doit être accompagnée des juste moyen et d'instruments efficaces le budget présenté est en baisse de 1 milliard d'euros, 5 en crédits de paiement à périmètre constant pour l'année 2020, nous devons donc rester vigilant afin de conserver les moyens de nos ambitions, le programme 112 impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire voit ses crédits augmenter cela fait notamment écho à la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires doté de près de 50 millions d'euros pour sa première année d'exercice, la présence d'élus dans la gouvernance nous satisfait certainement la présence d'élus du littoral, comme réclamé par mon collègue Jean-François Rapin nous satisferait, bien sûr, la coordination mission principale de l'agence doit être un objectif saluer l'État et les collectivités sont partenaires pour tous les enjeux des territoires et leur relation est une des clés de la réussite de la cohésion des territoires, je note également le 10 millions d'euros en direction d'un soutien en ingénierie pour les collectivités territoriales, souvent nécessaire pour les collectivités qui n'en disposent pas parfois il faudra mieux accompagner les agences d'urbanisme comme à Dunkerque, Lille, Maubeuge, Saint-Omer, qui sont de l'ingénierie locale et durable pour les territoires qui en disposent, le partenariat s'incarne également de la contractualisation avec les territoires, notamment avec la nouvelle génération de contrat plan État Région nos exigences restent les mêmes que l'an dernier, le soutien au projet prioritaire des collectivités territoriales sur ce thème, le contrat de ruralité et son financement reste un sujet de préoccupation, autre sujet de préoccupation : la prime à l'aménagement du territoire l'an dernier, nous avions déjà lancé un cri d'alerte sur la baisse constante des moyens alloués à cette prime, nous demandions alors la stabilisation des autorisations d'engagement autour de 14,5 millions d'euros, elle est prévue cette année autour de 6 millions d'euros, c'est très insuffisant, ce mécanisme est indispensable pour le développement du tissu économique de nos territoires en ce sens nous soutiendrons l'amendement déposé afin de rehausser de 4 millions d'euros les autorisations d'engagement et toutes les réflexions pour repenser ce système, il en est de même pour les fameuses zones de revitalisation rurale, enjeu crucial pour nos territoires les plus fragilisés, nous attendons beaucoup de la mise en place des préconisations de l'agenda rural la labellisation de 460 maisons France service comme à Bourbourg Cateau-Cambrésis ou à 11 dans le Nord ainsi que l'augmentation du budget attribué à ces dernières sont des premiers pas, nous resterons attentifs, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, à leurs moyens dans les années à venir, sur ce point, nous devrons, d'ailleurs nous interroger sur le service bancaire d'accès aux espèces comme le souhaiterait, mon collègue Daniel Chassain, sénateur de la Corrèze, je voulais évoquer le programme 147 relatif à la politique de la ville qui diminuent notamment d'autorisations d'engagement et voit son périmètre se modifier avec un transfert vers le programme 112 impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire, le nouveau programme national de renouvellement urbain produit de premiers effets, nous serons évidemment attentifs aux évolutions budgétaires futures et à la poursuite de sa bonne mise en oeuvre sur tous les territoires des quartiers à la ruralité des banlieues au centre-ville, monsieur le ministre, à la cohésion des territoires est fondamental pour notre pays, nous devons continuer à investir dans nos territoires et les efforts visibles dans ce budget sont encore parfois insuffisant sur l'aménagement du territoire, pour cette raison le groupe, les indépendants, ça se tiendra sur cette mission en l'état. Merci. Parole est maintenant à monsieur Rémy Pointereau pour le groupe Les Républicains et vous avez 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le Ministre Mesdames, messieurs, chers collègues, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2020 nous arrivons à la discussion de l'ensemble de la mission cohésion des territoires pour ma part je souhaite consacrer concentrer mon intervention sur les crédits des programmes 112 et 162 relatifs à la question de l'aménagement du territoire, notre collègue Louis-Jean de Nicolaï pour le travail effectué au nom de la commission de l'aménagement du territoire, c'est vrai que la tâche n'est pas simple, je le sais pour avoir porté ce rapport pendant 10 ans et il est toujours désagréable qui plus est, pour un sénateur d'observer des diminutions de crédits consacrés à l'aménagement du territoire, vous, vous me direz, monsieur le Ministre, que cette fois-ci les crédits ont augmenté, c'est un effet le cas pour le FN FNADT il y a peut-être là une volonté de redynamiser le fond, je ne peux que partager mais pour l'avoir demandé depuis plusieurs années, c'est enfin arrivé, mais l'augmentation ne concerne pas tous les outils inscrits dans les programmes, par exemple, les crédits alloués à la prime d'aménagement du territoire patte font de nouveau connaître une érosion et celle-ci risque de lui être fatal, déjà divisé par 4 depuis 2013, des montants alloués dans ce PLF 2 vont atteintes que 6 millions d'euros, alors qu'ils étaient de 40 millions d'euros il y a encore quelques années, ce qui m'amène à l'interrogation suivante : monsieur le Ministre, souhaitez-vous la fin de la pâte, car tout ce rabotage s'apparente à une obsolescence programmée, je tiens à rappeler 2 choses concernant la prime, c'est l'un des derniers leviers d'aides directes aux entreprises qui s'installent dans nos territoires, sommes-nous en situation de plein emploi pour nous permettent autant de diminution, je ne le crois pas, ensuite l'étude qui a été commandée en 2017 par le CGET au cabinets d'audits Sahnoun avait confirmé l'intérêt de la pâte comme outil de cohésion territoriale, c'est un choix que je regrette fortement c'est pourquoi je soutiendrai des amendements visant à rétablir le montant de l'année dernière qui était beaucoup plus élevé concernant l'agence nationale de cohésion des territoires, je m'interroge, non pas sur ses prérogatives, mais sur les moyens qui lui sont consacrés, pour y répondre, il y a en effet un programme problème à cet égard, avec seulement 49 millions d'euros de budget, comment peut-on prétendent que l'agence deviendra un vrai pôle de proximité, de soutien et d'expertise et donc être compatible avec les besoins des territoires, nous aurions souhaité plus de moyens pour que cette structure soit une véritable agence de revitalisation rurale, ce qui risque de ne pas être le cas, j'en viens aux zones de revitalisation rurale avec mes collègues Frédérique Espagnac et Bernard Delcros nous avons récemment remis à la ministre, Jacqueline Gourault, notre rapport sur le sujet, c'est vrai que c'est un outil auquel nous croyons fortement, c'est l'un des derniers éléments d'attractivité pour les territoires ruraux, un des derniers moyens de résorption de leur fragilité structurelle puisque, en effet, la politique des pôles d'excellence rurale a été supprimé le Fisac a quasi disparu sans compter les contrats de ruralité qui ont été mises en place en 2017 et qui n'ont déjà plus de crédits alloués dans ce contexte, les ZRR apparaissent comme le dernier phare dans la nuit de l'aménagement du territoire à la croisée des chemins, il nous faut insuffler un nouvel élan au dispositif, c'est tout l'enjeu de notre rapport, et là, l'Assemblée nationale a voté un amendement pour Jean le dispositif jusqu'au 30 décembre 2020, soit une progression de 6 mois je ne pense pas que cela soit suffisant pour construire un zonage veut cibler plus efficaces pour la ruralité, c'est pourquoi nous proposons de proroger le classement actuel jusqu'au 31 décembre 2021, non pas pour le maintien d'un statu quo, mais bien pour prendre le temps de définir des critères plus adapté pour tenir compte des fragilités des territoires et d'améliorer le ciblage, ainsi que l'efficience des dispositifs associé au zonage, enfin je souhaite conclure sur un point que je dois l'avouer commence vraiment à nous, excédés, les uns et les autres et je sais que je ne suis pas le seul, même s'il sort du cadre des programmes en question, il s'agit du fonctionnement opaque de la DETR, nous discutons de la cohésion des territoires, je crois que cette notion, appelle à une cohésion des acteurs qui agissent dans et pour les territoires, or le fonctionnement actuel de la DETR ne s'inscrit pas dans cette logique, membre de la commission de terre dans mon département, celle-ci n'a ni connaissance des arbitrages de la préfecture ni connaissance des critères retenus ayant permis de donner un accord ou non à un dossier et un projet dont le montant de subventions est inférieure à 100000 euros d'ailleurs, nous avons la liste des dossiers retenus que seulement un an après, au fond, j'observe que la réserve parlementaire était bien plus transparente que la DETR. Ce sont les parlementaires qui chaque année. Ce sont les parlementaires, je le rappelle, qui, chaque année, votent le budget et le montant de la DETR, et non les préfets. Et je souhaite que tous les dossiers de DETR soit. Examiner avec les membres de la commission des élus, et ce à partir du premier Euro dépensé nous réclamons donc plus de transparence et des amendements en ce sens seront discutées, je vous remercie de votre attention. attention. La parole est maintenant à Madame Viviane Artigalas pour le groupe socialiste et républicain pour 4 minutes. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis 2017, le budget logement a perdu 3 milliards d'euros, il est devenu le 1er contributeur aux économies de l'État et les coupes ont été particulièrement violentes dans le secteur HLM qui en 2018 a perdu un milliard 3 et autant en 2019, ce qui remet en cause les politiques d'investissement et de production de logements sociaux, par opposition, le pacte social et écologique, présenté le 5 mars dernier par Laurent Berger, Nicolas Hulot, place à juste titre le logement au 1er rang des priorités nationales, car il ne faut jamais relâcher les efforts en matière de logement ou alors, et on le constate actuellement les résultats se dégradent très vite et les répercussions sur les ménages, l'activité et l'emploi sont immédiats perte de pouvoir d'achat recule de l'accession sociale à la propriété, baisse de la construction et des chantiers de rénovation et encore, nous prenons en compte les taux d'emprunt favorables, ce qui explique que les offices HLM ne sont pas encore en danger, la France doit produire du logement abordable et soutenir les familles modestes dans leurs projets d'acquisition, mais comment résorber l'habitat indigne, si nous ne nous pouvons pas reloger les familles : comment soutenir la production de logements sociaux si nous privant les organise HLM de leurs ressources, comment demander aux maires de mettre en oeuvre les politiques publiques, s'ils n'en ont plus les moyens, force est de constater que, dans la continuité des précédents Budgets, l'objectif du projet de loi de finances 2020 et encore de faire des économies sur le logement à compter de janvier 2020 la réforme des aides au au logement qui seront calculées sur la base des ressources du trimestre précédent, et non plus sur celle perçus 2 ans auparavant, va engendrer une économie de l'ordre de 1 milliard 4 prix aux familles les plus modestes au nom de la justice sociale qu'est le mesures ont été prises pour soutenir les ménages qui vont être privés brutalement de toute aide au logement de plus ce sont les jeunes de 18 24 ans, qui est en train d'activités qui vont porter une part significative des économies attendues car, oui, notre société avait la faiblesse de soutenir pendant quelque temps, ces jeunes confrontés à la tri dans la vie active et aux difficultés d'accès au logement, qui sont liées à la précarité de l'emploi, cette réforme associée à celle de l'assurance chômage, entrée en vigueur le 1er novembre va très durement impacté donc en citoyens et notamment les plus fragiles, dans ce contexte, le revenu revenu universel d'activité, mesure phare du plan anti-profs pauvreté annoncée par le président de la République, il y a un an, nous inquiète en raison de la conditionnalité du dispositif et de son financement à enveloppe constante, l'objectif affiché de la réforme, hé bien de conditionner le versement de cette aide unique à la recherche d'une activité dans ces conditions, l'intégration des aides personnelles au jeune au logement Vahirua pose problème car s'étonne ignoré les principes qui fondent depuis plus de 40 ans, les aides au logement, conçu pour aider les familles modestes à accéder à un logement correspondant à leurs besoins et donc plus de la moitié travaillent une telle, une telle réforme doit faire aucun perdant quelles assurances pouvons, pouvez-vous nous donner que la réforme ne sera pas l'occasion de baisser encore les APL ou d'en modifier l'organisation. Le président de la République a regretté tout récemment devant l'de jeunes étudiants, la baisse de 5 euros des APL, mais depuis le début du quinquennat les aides au logement sont la cible de votre gouvernement, avec en plus le gel des APL, puis leur sous-évaluation systématique, vous avez également supprimé les pas l'APL accession but 2017 l'impact de vos réformes sur les aides au logement, c'est l'aveu c'est l'avait déjà 7 milliards d'euros, ce sont autant d'atteintes portées au pouvoir d'achat des ménages les plus fragiles et plus jeunes dans ces conditions, monsieur le ministre vous croire quand vous parlez de justice sociale réelle relève véritablement de l'acte 2 fois. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à monsieur Jean-François Longeot pour le groupe Union centriste, si vous avez 3 minutes. Un petit peu de silence s'il vous plaît, écoutez l'orateur merci. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'acte II du quinquennat doit assurément être celui des territoires, nous pouvons effectivement observé la traduction de cet objectif par l'examen des crédits relatifs à la cohésion des territoires du projet de loi de finances pour 2020 crédits en hausse de 6 pourcent en autorisations d'engagement et 4,7 en crédits de paiement c'est hausse résulte ainsi de la mise en place d'un nouvel opérateur, l'Agence nationale de la cohésion territoriale des territoires, l'ANC été la création de nouvelles actions territorialisée, ainsi que la montée en puissance des moyens consacrés aux services publics de proximité avec la labellisation de 460 structures intitulé France : je me réjouis que l'agence nationale de cohésion des territoires, si elles ne constituent pas la réponse miracle aux inégalités et disparités territoriales mises sur le devant de la scène politique constitue bien un 1er pas pour y répondent sur le long terme car, à la veille d'un nouvel acte de décentralisation censée ouvrir la voie à la différenciation pour définir avec chaque territoire une réponse adaptée sur mesure cette agence doit être au service des collectivités de leur projet et de leur cohésion. Je salue également la stabilisation bienvenue des transferts financiers de l'État aux collectivités, de même que la mobilisation des moyens supplémentaires pour le développement des services publics dans les territoires, avec comme objectif qu'en 2021 chaque citoyen puisse accéder à un service public en moins de 30 minutes néanmoins plusieurs points de vigilance demeure quant à la pérennité de dispositifs essentiels aux dynamiques locales tout d'abord le faible montant accordé à la prime d'aménagement du territoire, la patte confirme une stratégie d'érosion progressive mises en Oeuvres depuis plusieurs années sur cet outil d'attractivité qui avait, qui a démontré son efficacité. Par la suite, la suppression du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, on l'a évoqué le Fisac retire des montants précieux en faveur des territoires ruraux les plus isolés qui sont pourtant ceux qui ont le plus besoin pour contrer leur dévitalisation, enfin je ne peux vous cacher mes inquiétudes face à l'avenir incertain des zones de revitalisation rurale les ZRR outil efficace pour un âge même aménagement équilibré du territoire ces inquiétudes résulte une fois encore des conséquences malheureuses de la loi neutre dans l'extension des périmètres intercommunaux approfondir non redessiner la carte du zonage Federer au 1er juillet 2020, ce sont plus de 4000 communes qui sortiront du zonage et cesseront de bénéficier des mesures associées au classement alors même que leur situation ne s'est pas ou très peu améliorée si l'Assemblée nationale a adopté un amendement permettant de décaler les effets de cette mesure au 31 décembre 2020, cette période est trop courte pour une réforme juste une réforme équilibrée, une réforme efficace et définir des critères plus adaptée à la réalité des périmètres intercommunaux, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant monsieur Mathieu Darnaud pour le groupe Les Républicains et vous avez 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, au coeur des conflits de notre société se pose plus que jamais la question de notre cohésion nationale et celle-ci repose pour beaucoup sur les opportunités et les obstacles créés par nos territoires, ce budget est d'abord Monsieur le Ministre, comme l'ont rappelé certains rapporteurs ainsi que notre collègue, Rémy Pointereau, l'a souligné à l'instant, marquée par une dangereuse érosion de la prime d'aménagement du territoire et l'avenir incertain des zones de revitalisation rurale, il se distingue aussi par la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires à l'ambition bien modeste puisque seuls 10 millions lui sont réellement attribués, le reste ne faisant que recycler sous des appellations novatrice des crédits ancien et constant et vous me permettrez d'insister sur ce point parce que c'était la crainte que nous formulions il y a peu, ici lorsque ce sujet venait en en débat et cette crainte s'accompagne aussi du fait que la gouvernance qui se profile, malheureusement, risque d'exclure, j'allais dire, toujours un peu plus les élus des territoires au profit de ce qu'imposera cette agence de l'État sur ce sujet, je rejoins d'ailleurs la : la position des rapporteurs et mise sur le programme 112 impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire qui manque cruellement de visibilité : comment, Monsieur le Ministre, dans ces conditions, le Parlement peut-il apprécier à leur juste valeur l'évolution de ces différentes actions nomades qui passe d'un programme à l'autre, c'est ce qu'il s'est passé pour les crédits de contrats de ruralité sorti de ce programme en 2018 et dont les 45 millions qu'il représentait à l'époque ont fondu de moitié après leur intégration au sein de la dotation de soutien à l'investissement local je regrette également le fait que dans le budget présenté par le gouvernement, les communes concernées par la sortie du dispositif des ZRR ne puisse faire l'objet d'une prorogation ainsi que celles qui était soutenu en raison de leurs charges dans le programme Petites Villes de demain, mais surtout avec la meilleure bonne foi budgétaire du monde, on aura du mal à percevoir des moyens nouveaux correspondant à l'agenda rural annoncée en septembre dernier par le 1er ministre comme réponse à la crise des gilets jaunes j'observe d'ailleurs que dans le texte, engagement et proximité, seule une mesure pardon cohésion des territoires du budget pour 2020 est aussi marquée par la labellisation des maisons de service au public en maison France service cette harmonisation par le haut, suis autant la volonté exprimée par le président de la République que par l'avis de la Cour des comptes que ces maisons puisse monter en gamme et faciliter l'accès des citoyens des communes rurales à davantage de services publics en permettant d'y affecter davantage de démarches administratives est une trajectoire que nous partageons, au moins sur l'affichage, mais une fois de plus entre l'ambition et la réalisation, il y a un effort financier conséquent que ce projet de loi de finances ne porte pas en faire ce lieu parfaitement identifiés, dont les habitants auront la certitude qu'en s'y rendant ils trouveront les réponses à leurs questions et pourront effectuer leurs démarches demande bien des moyens supplémentaires, enveloppe constante en maintenant la subvention de 30000 euros par maison, nous n'y feront pas entrer les services téléphoniques ou de visioconférence annoncée de plus sur les 1344 maisons de service au public, les préfets ont à ce jour décerner le Label France service à 460 maisons sur une liste de 700 initialement proposé, qu'en sera-t-il monsieur le Ministre, de celles qui n'auront pas à ce même pu se mettre à niveau avant la date du 31 décembre 2021 pour atteinte ce précieux Label, mettra-t-il un terme à son soutien, les laissant ainsi végéter dans une sorte de 2ème, division avec le risque de voir les collectivités se désengager de structures qui ne parviendront jamais à la dimension critique et j'en finirai par là à la crise des gilets jaunes, le gouvernement a répondu par des mesures attendues portant sur le pouvoir d'achat, mais ce qui crée l'attractivité dont les salaires et le pouvoir d'achat de demain, c'est l'investissement aujourd'hui pour qu'à l'avenir, vivre dans les territoires ruraux ne soit plus une somme de contrainte, mais un choix qui n'exonère pas la République de ses promesses, certes, je n'ai pu très pas à ce gouvernement l'entière responsabilité du désinvestissement dans la ruralité manifeste depuis l'abandon notamment des pôles d'excellence rurale mais il manque hélas la véritable stratégie nationale en faveur de notre cohésion nationale, il manque cette ambition qui permettrait de ne plus entrevoir le développement des territoires comme une série de dépenses, mais comme un Paris fondée sur des investissements je vous remercie. La parole est à Madame Annie Guillemot pour le groupe socialiste et républicain et vous avez 6 minutes. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues après Viviane Artigalas je vais revenir sur la situation du logement et des quartiers, monsieur le Ministre, sans arrogance mais avec une certaine sincérité, je crois pouvoir dire que vos décisions depuis 3 ans, sont révélatrices de votre vision du modèle français du logement social durement attaqué depuis le début de ce quinquennat avait même un tout récent rapport public sur l'ouverture au privé par l'IGF qui dépend de Bercy, réalisée à la demande du gouvernement, là vous ne pouvez pas dire c'est les autres, la financiarisation du logement social, même si vous minimisez-vous Monsieur le Ministre, ce rapport, d'autres pays ont essayé, comme l'Allemagne et, aujourd'hui, la ville de Berlin, qui vient de voter l'encadrement des loyers pour 5 ans, il semble en écoutant Action Logement, et pas seulement le secteur HLM qui ne censeur qu'après la ponction violente de plus d'un milliard en 2008, parce que les taux sont bas 6 milliards tout de même de ponction sur le quinquennat en écoutant donc Action Logement, il semble que c'est bien Bercy qui décide tout, même si vous en défendez pour qu'Action Logement évoque une forme de mépris, il faut dire que l'État continue de faire les poches non seulement de l'USH mais aussi pour 2020 les poches d'Action Logement pour financer à sa place le Fnac et le final 800 millions d'euros, il faut tout de même que Action Logement en est quoi AC. Cette offensive de l'État allant compte d'Action Logement n'est-elle pas le signe des prémices d'une remise en cause du caractère autonome d'Action Logement, comment ne pas s'interroger sur les impacts sur la trésorerie, sur le plan d'investissement volontaire de 9 milliards signé en 2 en avril dernier, l'aide à la rénovation énergétique cumulable avec les aides de l'Anah ou sur le milliard pour le financement de la mise aux normes des salles de Bains. Ce n'est pas comme si le logement rapporté plus à l'État qui ne lui coûte en 2018, les aides au logement, représenté 39 6 milliards d'euros, 4 moins 4,5 pourcent bien en-deçà des 77,5 milliards d'euros de recettes fiscales qu'il a généré plus 3 virgule 8 pourcent le logement, c'est tout à la fois un facteur de cohésion sociale de développement économique des territoires et de l'emploi, mais vos choix budgétaires assumez-les, le logement, hé bien malheureusement la variable d'ajustement du budget de l'État, nous voterons compte car nous considérons votre politique purement budgétaire ne répond pas aux nécessaires, enjeu de cohésion et accentue les inégalités, les chiffre ne manquent pas : la production de logements neufs étaient en repli en 2018 et cette tendance s'est confirmée en 2019, les conséquences sur la précarité ne sont pas fait attendre puisque, selon les chiffres récents de la Fondation Abbé Pierre, notre pays compte 4 millions de personnes mal logées, plus 12 millions de personnes qui connaissent une situation fragilisée par rapport au logement, le président de la République a reconnu la semaine dernière, traîner comme un boulet. La baisse de 5 euros des APL, passons, a-t-il dit, cela a été fait : ben non, nous nous ne passons pas Monsieur le Ministre, parce que le boulet ce n'est pas le président de la République qui le traîne ce sont tous ceux qui, le 20 du mois n'arrive pas à joindre les 2 bouts, ce sont ceux qui ont du mal à élever leurs enfants, surtout lorsque le président de la République reconnaît en même temps que l'assignation à famille ou l'assignation à origine s'est creusé ces décennies, assurant que la seule manière de combattre, c'est l'éducation, le savoir bien sur l'éducation, mais sans logement, sans emploi, c'est bien difficile, j'ai souvent dit et redit en 17 ans maire qu'il y avait bien sur l'éducation, la santé, le culture la culture, le sport, mais que quand il y a une famille à un logement pour s'abriter pour vivre son intimité un emploi pour vivre dignement la sécurité qui protège alors ensuite on peut, mais ensuite seulement, on peut faire faire face au reste, sans logement et sans emploi comment restons citoyen. Mais avec le logement et l'emploi, il faut aussi Monsieur le Ministre, le respect, l'espérance donner cette espérance, le respect, quelles que soient vos origines, votre religion, votre sexe et l'espérance d'un monde meilleur, d'un monde de progrès pour ses enfants, je rejoins Jean-Louis Borloo avec son titre vivre ensemble pour une réconciliation nationale, tant dans les villes, les banlieues que nos campagnes,

pour sur la paupérisation du logement social et des quartiers par l'ANRU 30 pourcent des locataires dit HLM aujourd'hui vivent sous le seuil de pauvreté, mais le pire cette année en 2018, plus de la moitié des attributaires des logements HLM sont sous le seuil de pauvreté, le logement social, si je peux dire ce spécialiste de plus en plus dans l'accueil des plus pauvres mais c'est dramatique, la moitié des attributaires, je le disais, l'absence de mixité sociale en géant, non pas des risques maintenant, mais des ghettoïsation un séparatisme social qui ne peut qu'engendrer affrontements et violences mixité diversité mais quand on parle tous. Quand on parle, vous, votre politique du logement d'abord renforce malheureusement les poches de pauvreté alors qu'il faudrait que le privé accueille aussi les populations les plus précarisées, les familles ne peuvent plus accéder à la propriété ne peuvent plus non plus supporter des loyers du privé qui ne cesse d'augmenter, vous partagez ce diagnostic, je le sais mais alors, qu'en faites-vous, on ne sent pas dans le le pour le logement, comme pour les quartiers de politique offensive alors que ces quartiers compte beaucoup de logements sociaux en plus la réforme de la taxe d'habitation va affecter par ricochet la DSU des communes les plus pauvres du fait de leur nouveau potentiel fiscal et quelle maire aura intérêt à construire du logement social, enfin, en matière de rénovation urbaine, vous ne respectez même pas l'engagement pris pour l'ANRU, certes, on arrive à la phase opérationnelle, mais durant ce mandat, les habitants n'auront vu que quelques démolitions, il y a pourtant des écoles à construire à rénover des Centres sociaux des équipements sportifs commerciaux rénover une école, c'est travailler avec les parents d'élèves, un sens social, c'est la construction d'un projet avec les habitants, vous me répondrez mais l'ANRU n'a pas besoin de crédits supplémentaires, les projets ne sont pas prêts mais l'État fait tout de même payer ses autres partenaires l'USH et Action logement, pourquoi l'État ne porterait-il pas comme en 2008, un choc, un choc d'avance de crédit avec dérogation aux marchés publics pour construire des des équipements publics avancer les projets de services publics qui font font l'unanimité, le gouvernement ne peut pas mettent sur la tape ce milliard qu'il a engrangé, alors qu'il a engrangé 2 milliards supplémentaires du fait de la réforme de la retenue à la source, la rénovation urbaine fait du sur place, défendez les territoires défendez les maires confrontés à des situations qui relèvent de la solidarité nationale, défendez les habitants de ces quartiers qui souffrent et pour la plupart, respecte la loi républicaine et souvenons-nous tous, comme le disait l'abbé Pierre que gouverner, c'est d'abord loger son peuple. La parole est maintenant, madame la présidente, Valérie Létard, pour le groupe de l'Union centriste.

2 ans après le vote de la RLS, un an après la promulgation de la loi élan la réforme du logement social que vous avez souhaité est en cours, dont acte, permettant une fois de plus 1,4 milliards d'euros d'économies sur les crédits du logement à l'État. Est-ce bien. Est-ce une interrogation. Sur laquelle il faut maintenant se pencher, il me semble que oui car, pour autant, le secteur du logement social présente un modèle économique régulier dont les évolutions structurelles ont modifié l'équilibre l'équation budgétaire imposée par la RLS complique l'atteinte des objectifs assignés au secteur qu'il s'agisse de l'engagement de poursuivre la construction neuve, à hauteur de 110000 logements sociaux sur la période 2020, 2022 ou de l'accroissement de 25 pourcent des rénovations, c'est la raison pour laquelle vous avez reconnu la nécessité d'une clause de revoyure aboutissant en avril dernier à un pacte productif avec les partenaires du logement social, mais aussi un plan d'investissement volontaires d'Action Logement sur le pacte productif pour répondre aux engagements de l'État, l'article 8 du PLF prévoyait une baisse de TVA sur certains logements sociaux en première partie de ce projet de loi de finances, le Sénat par des amendements déposés sur plusieurs bancs a rétabli et défendus par notre rapporteur Philippe Dallier particulièrement le taux de TVA à 5 5 pourcent s'agissant de la rénovation et de la construction du logement social sur l'ensemble du territoire, j'avais d'ailleurs appelé à plusieurs reprises, votre attention sur la situation D. et les besoins du bassin minier en la matière, devons-nous à ce titre, rappeler que le logement social est un bien commun de la nation par son objet et son mode de financement notamment et qu'il est porteur de dynamique positive en termes de réduction des inégalités d'emploi et de croissance, il faut donner de la lisibilité et les moyens d'atteindre ses objectifs au secteur qui s'interroge sur l'après 2022, la RLS sera-t-elle pérennisée, alors que la trajectoire d'endettement des bailleurs sociaux risque de progresser très rapidement dans les prochaines années, par ailleurs, si l'APL en temps réel est nécessaire, la méthode rapide et les études d'impact peut mesurer peu développer nécessite une grande vigilance sur ses effets de même de nombreuses inquiétudes se font jour concernant le futur Dominique Estrosi nous l'a rappelé il y a sur ce sur ces questions, l'intégration de l'APL qui pourrait porter atteinte significativement au monde du logement social, mais aussi aux aux publics éligibles permettez-moi ensuite monsieur le Ministre de m'interroger sur le plan d'investissement volontaires d'Action Logement, rendu public en avril dernier par lequel 9 milliards d'euros sont mobilisés par la structure, je n'en vois pour heure, pas de concrétisation, notamment sur un exemple le logement indigne alors que le drame de la rue d'Aubagne à Marseille, a eu lieu il y a plus d'un an action logement a plus que jamais besoin de déployer ses moyens financiers et humains, or la liste de décrets notamment en application d'élan et de l'habilitation à légiférer par ordonnance n'ont toujours pas fait l'objet de toutes les publications attendues, le comité des partenaires d'Action Logement, auquel je suis particulièrement attaché, n'est toujours pas installé, de même que dès que certaines mesures nécessaires au bon fonctionnement de la gouvernance pourquoi monsieur le Ministre, il me semble urgent de mettre en oeuvre ce pivot et à la convention quinquennale, mais les moyens financiers semble figée non dépensés aussi dans le cadre de sa mission de contrôle et d'évaluation de la loi, je pense que le Seigneur a serait fondé à évaluer précisément la mise en oeuvre de la réforme d'Action Logement, en plus de de l'état d'avancement des textes réglementaires je souhaiterais, Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous donner des éléments concernant le prélèvement de 500 millions d'euros prévue à l'article 75 du PLF est présenté comme une contribution temporaire d'Action Logement au final quelle pérennité pour cette mesure qu'il ne faudrait pas voir au-delà de 2020, comme une opportune substitution au financement de l'État, monsieur Dallier, nous pourrons vous soutenir un peu plus tard je partage entièrement les inquiétudes d'Annie Guillemot exprimée dans son rapport sur la politique de la ville et sur l'ANRU je n'irai pas plus loin, sur cet aspect complètement en phase concernant l'main en 2019, l'agence a performé sur tous ces secteurs d'intervention avec une hausse de 20 pourcent de son action et une vraie dynamique de rénovation sur l'habitat privé monsieur le ministre, le budget de l'ANA risquent d'être déstabilisés dès fin 2020 et a fortiori en 2021 alors que les nouvelles missions, notamment en faveur de la revue réalités lui seront confiés ont plus d'écho pro-dégradé des plans chaudière d'habiter mieux car il y a beaucoup de sujets comme ceux là qui vont monter en puissance, sauf évidemment, Monsieur le Ministre, si nous baissons les curseurs les critères d'éligibilité ou de financement pour contenir les choses, or aujourd'hui, vous l'avez dit, monsieur le ministre, et vous avez raison il faut massifier toutes ces questions, compensation de recettes de quotas carbone affectés à vous les avez plafonné l'année dernière à 420 il y a 840 millions de recettes de quotas carbone, c'est-à-dire qu'il y en a 420 qui part dans la réduction du déficit de l'État, Monsieur le Ministre, ne croyez-vous pas que ces 420 millions je sais que vous le partagez Bercy devrait vous laisser les investir au service d'une d'un développement et d'une massification de la rénovation thermique en tous points de nos territoires, vous l'avez entendu, vous l'avez compris les sujets ne manquent pas, urbains, ruraux, politique de la ville, rénovation thermique des logements sauver notre modèle du logement social, tant qu'il est encore possible de le faire, mes chers collègues, nous ne voterons pas contre cette cette mission budgétaire parce que Monsieur le Ministre, vous faites tout ce que vous pouvez pour y arriver, mais par contre, nous nous abstiendrons parce que si vous aider que nous abstenir parce qu'il faut que l'État que Bercy conclure le 1er ministre vous entendent. Merci madame la présidente. La parole est à notre collègue cher je babary pour le groupe Les Républicains. vous avez 3 minutes. pour l'ensemble de cette mission cohésion des territoires 15 milliards d'euros sont inscrits en autorisations d'engagement et 15,1 milliards en crédits de paiement ainsi comme les années précédentes, le budget de la mission est en baisse, pourcent pour les autorisations d'engagement et moins 7 53 pourcent pour les crédits de paiement, monsieur le rapporteur, l'a souligné, c'est la seule mission du budget général dans les crédits diminuent de manière importante, j'ajouterai même de manière constante, avec une diminution de près d'un milliard et demi d'euros c'est le budget le plus mis à contribution dans le cas de la réduction des dépenses publiques, le programme 109 relatifs à l'aide à l'accès au logement est fortement touchée il acte la réforme des aides personnelles au logement engagée par le gouvernement concernant le mode de calcul. Elles seront dorénavant calculés en fonction des ressources actuelles des bénéficiaires et non plus en fonction des ressources de l'année, elle moins de l'application de ces nouvelles règles, conduit à une réduction de 1,4 milliards d'euros des crédits budgétaires consacrés aux APL cette économie sera supporté aussi bien par les bailleurs sociaux que par les bénéficiaires de ces aides. En 2018, 6 6 millions de ménages ont bénéficié de la PLV des ménages locataires bénéficiaires avaient des revenus inférieurs au SMIC et 99 pourcent inférieur à 2 fois le SMIC, je m'inquiète de l'impact de cette mesure sur les plus jeunes, comme l'année dernière le programme 147 politique de la ville semble épargner 473 millions d'euros sont inscrits en autorisations d'engagement et 498 millions en crédits de paiement, la contribution de l'État au financement du nouveau programme national de renouvellement urbain NPNRU et de 25 millions d'euros pour l'année 2020, le budget 2018 avait acté le retour de l'État dans le financement du renouvellement urbain aux côtés d'Action Logement et des bailleurs sociaux, le gouvernement s'était alors engagé à porter le NPNRU à 10 milliards d'euros sur la durée du programme avec une part de financement de l'État d'un milliard d'euros, soit 200 millions par an au cours du quinquennat. Pourtant, dès 2018, le compte n'y était pas, seuls 15 millions d'euros sur les 200 étaient inscrits en autorisations d'engagement et en crédits de paiement en 2019, l'État avait augmenté sa participation à hauteur de 185 millions d'euros en autorisations d'engagement et 25 millions en crédits de paiement pour 2020, seuls 25 millions d'euros sont inscrits en crédits de paiement, on est bien loin des 200 millions promis, l'État ne respecte pas ses engagements en proportion de son engagement global, l'État finance toujours moins que les bailleurs sociaux et Action logement on observe cependant que le NPNRU commence enfin à prendre forme, plus des 2 tiers des projets de transformation ont été validés si on ne peut se satisfaire du fait que l'État ne respecte pas ses engagements, les mesures présente dans le projet de loi correspondent cependant aux accords signés entre les acteurs du secteur du logement social et le gouvernement aussi, et le gouvernement aussi, malgré de nombreuses réserves, le groupe Les Républicains votera les crédits de la mission, je vous remercie. Vous avez la parole merci beaucoup monsieur le président, Mesdames et messieurs Les les rapporteurs, monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs les les sénatrices et les sénateurs, je suis très heureux de m'exprimer devant vous sur ce budget, qui est d'une importance très forte, une importance très forte parce que le moment que traverse notre pays est un moment qui nous oblige, il nous oblige à lutter contre les fractures territoriales il nous oblige à lutter contre ce sentiment, cette perception cette réalité que beaucoup de nos concitoyens partagent celle d'être assigné à résidence, ou celle de tout simplement de ne pas avoir les mêmes chances que les autres en fonction du territoire d'où nous venons et donc le moment que nous traversons est un moment qui nous oblige d'autant plus dès lors qu'il s'agit de lutter contre ces inégalités territoriales des inégalités territoriales, il faut le dire, qui parfois sont la source même. D'une sorte de déterminisme social qui est l'un des mots les plus profonds que traverse notre pays, songez que dans notre pays si vous êtes ouvrier c'est votre arrière arrière arrière arrière petite fille ce qui peut-être aura une chance de devenir cadre ce déterminisme social plus accentuée dans notre pays que dans d'autres pays européens, il est en partie lié à ces fractures territoriales que connaît notre pays que nous dont nous discutons aujourd'hui est un budget qui est principalement orienté vers la lutte contre ces fractures territoriales, alors on aura, vous aurez l'occasion également de discuter d'une partie de ce budget demain avec Madame Jacqueline Gourault, mais le budget discuté cet après-midi et demain répondent dans les 2 cas au même objectif : comment faisons-nous en sorte pour que cette possibilité de réussite puisse s'exprimer à la fois que vous soyez dans un territoire dits périphériques à la fois que vous viviez dans nos ruralités ou à la fois que vous viviez dans les métropoles et je voudrais insister aujourd'hui sur 4 axes : qui sont les fondements de la mission le 1er axe c'est répondre aux citoyens d'un point de vue d'accès au service public et de rééquilibrage territorial ça passe notamment par la question des Maisons France service que beaucoup d'entre vous ont évoqué, qui sont au final un témoin du fait que les services publics, il faut le dire, ne sont pas aujourd'hui les mêmes partout sur le territoire et que pire encore, certains ont été accentuées en termes d'inégalités d'accès aux services publics, alors ces Maisons France service au 1er janvier 460 ouvriront et je voudrais par là même répondre à plusieurs questions qui ont été posées, celle d'abord de monsieur le sénateur d'Arnaud on a augmenté la dotation pour les maisons, France, service, elles étaient, vous le savez, Monsieur le Sénateur, à 25000 euros et nous les passons à 30000 euros, celle de monsieur le rapporteur Delcros, qui est essentiel, qui concerne la qualité de service de ces maisons France service l'objectif de ces maisons de francs de service et de ne jamais laisser de côté une MSAP jamais mais c'est de d'accompagner la MSA fait vers un niveau de qualité lui permettant d'avoir le Label France service et je crois, et Madame, la sénatrice Françoise Cartron, l'a très bien dit l'objectif. ne serait pas étonné, mesdames et messieurs les sénateurs, de mes propos, l'objectif c'est de faire, c'est de faire en sorte que ces maisons France service puisse être partout sur le territoire et notamment qu'il y ait au moins une par canton, le 2ème élément sur l'aménagement du territoire sur lequel je voudrais insister, c'est la question du numérique, vous m'avez plusieurs entre plusieurs fois entendu le dire aujourd'hui, le numérique est quelque chose qui a accentué les fractures territoriales, beaucoup l'ont présentée en disant : le numérique, ça va être la solution à tous nos maux, non le numérique au moment où je vous parle, ça accentué les fractures territoriales, songez que du fait des modifications que nous avons porté dans la loi élan et que vous avez adopté du fait de la réouverture du guichet France-mobile que nous avons annoncé récemment, en 2019, c'est plus de 4 millions de foyers qui vont être raccordés à la fibre, c'est 2 fois plus qu'il y a 2 ans, on a doublé le rythme d'accélération du numérique en 2 ans dans notre pays, je crois que nous pouvons en être fiers parce que nous sommes en train et il faut le dire, en train de bâtir le principal réseau de services numériques en Europe bien mieux que nos partenaires britanniques ou Queneau partenaire allemand, c'est enfin la question de l'appui en ingénierie et renvoie et Monsieur le le sénateur Jean-Yves Roux, vous l'avez très bien dit, à la question de la création de cette à une société qui sera effective à partir du du 1er janvier 2020, vous avez raison, Monsieur le Sénateur Delcros Line, c'était son métier, ça va être d'accompagner les territoires dans une logique de projet, c'est dire qu'au centre de tout, il y aura la question de l'ingénieur au centre de tout, ce sera le fondement même de la c'est aimer et renvoyé à cela, la question des Budgets, c'est 49 millions d'euros de budget qui seront attribués à la cité, dans le cadre de ce budget, qui est présenté, mais il ne faut pas. écarté le fait que l'Inde, c'était son objectif même sera de travailler avec l'ensemble des opérateurs et l'ensemble des missions programmes que l'État bâti, que ce soit l'Lana, que ce soit l'ANRU, que ce soit la mission France mobiles, que ce soit Action coeur de ville, que ce soit la mission bourg centre que nous sommes en train de de constituer et donc, il serait faux de concevoir la c'était comme ayant comme simple budget ses 49 millions d'euros parce que plus encore l'nécessité a justement vocation à fédérer l'ensemble des programmes des agences qui travaillent pour le compte de l'État ou avec l'État sur l'ensemble des territoires

de l'activité de l'Epareca par là, c'était et c'est ça qui était d'ailleurs conforme à la loi que vous avez adopté s'agissant de la création de l'ANC sur les territoires, notre action, elle va porter aussi dans la poursuite de cette nouvelle politique que nous avons lancée, qui s'appelle Action coeur de ville pour lutter contre contre la dévitalisation et pour la revitalisation d'un certain nombre de nos centre-ville je me retour ne sur vis-à-vis de ça va faire beaucoup de de sénateurs et notamment le sénateur Martial Bourquin avec qui nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet, c'est plus de 4000 projets projets qui sont en cours de financement dans les 222 villes Action coeur de ville alors sur la nos ruralité, l'aménagement du territoire, il y a la question des ZRR le sénateur Delcros, le sénateur Louis-Jean de Nicolaï, monsieur le sénateur, point trop ou encore Monsieur le Sénateur, bonjour, vous avez tous évoqué les ZRR, souvenez-vous, il y a 2 ans quand ici même dans cet hémicycle avec monsieur le ministre, Jacques Mézard nous défendions déjà la reconduite du dispositif ZRR là où plusieurs villes devaient sortir, on les avait réintroduite et aujourd'hui ce qu'on vous propose, c'est de se laisser jusqu'à fin 2020 pour déterminer quel doit être le schéma qui sera celui qui qui viendra en succession du dispositif ZRR, il faut prendre le temps de la discussion avec l'ensemble des élus concernés pour voir quel est le bon schéma, moi je suis très attaché attaché pardon et je pense qu'il nous faut prendre le temps de cette discussion, c'est pour ça que nous avons à l'Assemblée nationale, décalé, tout ce qui, toutes les villes qui devait s'arrêter en juillet à fin 2020 pour se laisser le temps de la discussion, le 2ème axe strict stratégique, pardon, c'est la question de la politique de la ville, je voudrais insister évidemment sur la rénovation urbaine et Madame la sénatrice Annie Guillemot, ce que vous avez dit est strictement faux, je suis désolé de le dire en ces termes, je suis quand je suis moi, il y a 2 ans et demi nommée en charge du logement, l'ANRU étaient à l'arrêt dans notre pays, l'ANRU était à l'arrêt dans notre pays, les grues n'était plus là, on a passé un an à essayer de comprendre pourquoi ANRU est à l'arrêt, alors les leçons aujourd'hui venons nous dire vous allez pas suffisamment vite sur la rénovation urbaine, pointant du doigt par exemple qu'on rénove pas d'école depuis mai 2018 depuis mai 2018 et 190 écoles dont nous avons lancé la rénovation 80000 logements dont nous avons, nous avons lancé la rénovation et c'est le doublement des moyens de l'ANRU avec avec Action Logement avec des bailleurs sociaux que nous sommes en train de, de mettre en oeuvre, monsieur le le sénateur Dallier s'agissant des conditions de financement,

sur les sites que plusieurs d'entre vous ont mentionné également, c'est pour moi un projet extrêmement structurant dans cette politique de réussite républicaine pour nos quartiers qui vient en complément de la politique de reconquête républicaine auquel nous sommes tous attachés, le 3ème, axe stratégique, c'est la question du logement social, il y a plusieurs questions dans ce budget, il y a tout d'abord la réforme des APL en temps réel, c'est-à-dire cette contemporanéité ation des appels qu'on appelle à peine en temps réel, c'est à la fois plus claires et plus simple à prononcer les appels en temps réel, je crois qu'ici personne ne peut comprendre que le montant de vos appels jusqu'à présent étaient définies en fonction de qui vous étiez et de quels étaient vos revenus il y a 2 ans, c'est une aberration quand il y a 2 ans, vous étiez par exemple une femme avec un travail à temps plein et que, aujourd'hui, vous êtes mère célibataire avec un re avec une activité à temps partiel, hé ben vous n'avez pas accès aujourd'hui au montant des appels auxquels vous auriez droit ceci : personne ne peut le comprendre, nous ne pouvions pas faire des appels en temps réel, avant que l'impôt à la source ne soit fait, parce que nous profitons de la remontée des informations de l'impôt à la source pour pouvoir créer justement ce système des APL en des APL en temps réel, alors il y a une question qui est posée, et moi je, je, je, elle tout à fait légitime, c'est la question posée par le sénateur Dallier de savoir est-ce que le fait d'avoir cette Athènes en temps réel, c'est-à-dire que tous les 3 mois on va calculer vos appels en fonction des revenus de vous 12 derniers mois, est ce que, oui ou non, cela peut créer des effets de marché d'arrêt pour un certain nombre de nos concitoyens qui serait au bord des limites alors ce qui est sûr c'est qu'avec les appels en temps réel, vous avez cela tous les 3 mois, c'est à dire que si à un moment donné vous perdez le bénéfice et les droits aux appels pendant 3 mois, vous pouvez les récupérer les 3 mois suivants, là où dans le système actuel, lorsque vous perdiez parce que vous étiez aussi autour de ces plafonds voulait perdu pendant un an. Pendant un an, et donc moi je crois profondément que le système telle qu'il est conçu, est à mes yeux plus protecteur parce que s'adaptant précisément à chacune des situations, il y a ensuite la question de la ALS et je vous remercie madame la sénatrice Estrosi Sassone et Monsieur le Sénateur Dallier d'avoir mentionné tous les 2, le fait que dans cette loi de finances, comme je m'y étais engagé, nous avons repris l'entièreté désaccord suite à la clause de revoyure dans lequel vous vous étiez chacun investi et qui a permis de signer cet accord important avec les bailleurs sociaux un accord visant à apporter des accompagnements supplémentaires de la part de l'État, de la Caisse des dépôts et d'Action Logement et des objectifs à la fois de construction 110000 agréments par an et de rénovation de la part des bailleurs sociaux sur Action Logement je vais être très clair avec plusieurs d'entre vous qui ont évoqué le sujet action logement est un partenaire de l'État, j'ai eu l'occasion de dire encore récemment action logement non c'est pas un partenaire malmené, c'est un partenaire de l'État et je crois pouvoir dire que si c'était un partenaire malmené, nous n'aurions pas conclu avec Action Logement : un plan d'investissement volontaire de 9 milliards d'euros, qui est quelque chose de totalement inédit avec les partenaires sociaux et ce qui est faux, madame la sénatrice Guillemot, là aussi, ce qui est strictement faux c'est quand vous vous portez une suspicion auprès du gouvernement qu'il voudrait financiarisé le logement social, je tiens à rappeler que je me suis opposé à tous les amendements à tous mais je suis le ministre du Logement, Madame la sénatrice Guillemot je me suis opposé à tous les amendements qui visaient par exemple à revoir les règles dans le capital des et bailleurs sociaux et je crois que cette constance, elle a été réitérée sur ces, sur ces bancs, et à cette tribune pendant à de nombreuses reprises alors plusieurs d'entre vous ont évoqué un sujet d'importance également qui le revenu universel, l'activité le revenu universel d'activité, je voudrais là aussi être clair sur 2 points : le revenu universel d'activité, il n'y a sa grande concertation qui a été entamé dans cette concertation, j'ai obtenu le fait que les appels seront traités comme en supprimant logement ça veut dire quoi, ont 2 vertus absolument essentiel qu'il nous faut préserver la première c'est de solvabiliser un certain nombre des publics et donc il faut à ce titre que ce soit un supplément logement et le 2ème, c'est que ça nous permet de lutter contre l'habitat insalubre, j'en ai fait un marqueur fort de mon action, du fait du tiers payant qui aujourd'hui est opéré dans les appels et donc il nous faut garder les appels comme un supplément logements dans ce revenu universel d'activité, c'est ça qui est y compris donner à la concertation, en ces termes dans le cadre D D, des groupes de travail qui ont été faits vous appelez de vos voeux le retour de l'encadrement des loyers, il s'avère que cet encadrement des loyers dans la carte de la loi élan et vous avez activement participé, je vous en remercie, non on a permis de réintroduire aux communes qui le demandent et qui ne justifie, c'est cette réintroduction, on a fait pour Paris, et ça arrive maintenant sur l'île avec le l'accord que j'ai donné suite suite aux demandes et toutes les communes éligibles au dispositif évidemment verront mon ministère travailler à leurs côtés. Enfin, sur la lutte contre l'habitat insalubre et la rénovation énergétique l'année qui vient, or, à un moment important, c'est le passage du crédit d'impôt rénovation énergétique ont une prime, une prime qui permet de ne pas attendre 18 mois avant d'avoir le bénéfice de l'accompagnement de l'État, je crois que là aussi, tout le monde le comprend et c'était important de le faire et sur le l'habitat insalubre et le logement. On ne peut pas dire que ce gouvernement est resté les bras croisés à la suite du drame, madame la sénatrice de la rue d'Aubagne, on ne peut pas dire ça, surtout quand on a ici débattu de la proposition de loi de monsieur le sénateur, Gilles, 3 semaines avant le drame de la rue d'Aubagne, j'étais de plusieurs d'entre vous à Marseille pour annoncer ce plan initiative copropriétés dégradées, doté de 3 milliards d'euros dédiés justement à la lutte contre l'habitat insalubre dans le cadre de la loi élan nous avons aujourd'hui permis de faire en sorte que les marchands de sommeil soient considérés comme des trafiquants de drogue et, dans le cadre des discussions que nous avons eu avec Monsieur le Sénateur, Gilles ou avec des députés, comme le député député Volter, nous sommes en train d'accélérer les démarches localement pour pouvoir encore plus rapidement résorbé les cas d'insalubrité alors le dernier acte ce 4ème et dernier axe, c'est la question de l'hébergement d'urgence d'hébergement d'urgence est un sujet incroyablement compliqué, ce sont, au moment où je vous parle des milliers de personnes qui continuent à dormir à la rue, dont des femmes et des enfants, je crois pouvoir dire et je ne m'en félicite aucunement mais je crois pouvoir dire que l'effort sur l'urgence, n'a jamais été aussi fort en 2 ans nous avons pérennisé, près de 15000 places au moment où je vous parle, le dispositif d'émergents d'urgence et 150000 places, c'est plus que la ville du Mans et c'est sans compter le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile, je voudrais vraiment saluer le rapport et l'excellent rapport fait par messieurs les sénateurs, Armelle et Morrissey qui pointe du doigt tous tous la façon que le système a de fonctionner aujourd'hui et ma vision elle est très claire, il faut continuer, continuer à appuyer l'ouverture de places d'hébergement d'urgence, vu la gravité du moment pendant l'hiver, j'ai annoncé que nous pourrons ouvrir jusqu'à 14000 places supplémentaires, nous sommes déjà plus de 6000 places ouvertes pour permettent de gérer cette urgence et en même temps, la politique de l'hébergement d'urgence, elle doit reposer sur un 2ème volet qui est cette politique du logement d'abord de permettre à des personnes de sortir durablement de ces situations de détresse parce qu'on leur donne, non pas un abri n'non pas un moment de de répit mais on lui donne un vrai chez soi une vraie adresse c'est cette politique du logement d'abord qu'il dernière mesdames et messieurs les sénateurs, a permis de sortir 70000 personnes de ces abris de fortune 70000 personnes, c'est dire la gravité, encore une fois, et des drames humains auxquels nous assistons et donc ma position et de travailler avec énormément de détermination énormément d'humilité aussi, à la fois en renforçant l'hébergement d'urgence et en mettant en oeuvre cette politique du logement d'abord et Madame la sénatrice, Estrosi Sassone vous avez 1000 fois raison d'insister sur. le sujet de le sujet de l'accompagnement cet accompagnement et notamment l'accompagnement social, est l'une des clés à la fois dans l'hébergement d'urgence, mais surtout dans la politique du logement d'abord c'est un sujet sur lequel nous avons déjà eu l'occasion de travailler à de multiples reprises, ce qui fait que dans le budget que je vous présente aujourd'hui les crédits dédiés à l'hébergement d'urgence et dédiée au logement d'abord sont en augmentation, respectivement de 55 millions d'euros et de 45 millions d'euros au final mesdames et et messieurs les les députés. J'avais, presque j'avais presque terminé, je vous prie, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mesdames et messieurs les les sénateurs, j'ai été troublé par le les dernières notes que j'avais prise et je ne voudrais pas ne pas répondre à Monsieur le Sénateur Dallier, monsieur le sénateur Maurice sur la question de la sincérisation du budget du programme 177 vous avez raison de mentionner, du fait qu'on a encore ouvert des crédits en fin d'année, ce qui montre que cette sincérisation du budget, on doit la continuer, on a déjà fait beaucoup de progrès et d'ailleurs, le rapport de messieurs Armelle et et Maurice et le montre, on a fait beaucoup de progrès notamment, il y a un an et demi, on a remis beaucoup de sincérité et rebaser beaucoup de choses dans le programme 177 il est il est vrai qu'il faut continuer à aller dans ce sens-là, parce que les Budgets exécutés à la fin de l'année montre très souvent qu'qui dépasse les Budgets initiaux, c'est également la question de la convergence tarifaire sur lequel il y a eu des inquiétudes, nous sommes en train de les résorber et je crois que c'est très important ainsi voilà Mesdames et messieurs les les sénateurs, c'est un budget important, c'est un budget qui aujourd'hui traduit notre volonté de lutter contre ces fractures territoriales et je crois que c'est un un budget qui est d'autant plus essentiel dans le moment que traverse notre pays et je suis sûr que nous aurons mesdames et messieurs les sénateurs, des débats constructifs sur ce budget je vous remercie, merci monsieur mener. Nous allons maintenant procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission mission cohésion des territoires et nous sommes à l'état B. Nous allons commencer la discussion de 24 amendements en discussion commune ces amendements en discussion commune traite de thématiques très variées, outre l'existence d'incompatibilité de fond, la discussion commune est nécessaire pour tous les amendements qui prélèvent des crédits sur l'action du logement sur 35 pour un montant cumulé supérieur aux crédits inscrits en conséquence en cas d'adoption d'amendements, des amendements qui conduirait à dépasser les crédits inscrits tomberait automatiquement cette précision étant apportées, je vais passer à la présentation des amendements. Tout d'abord n'amendements qui porte numéro 723 il est présenté par Madame Lienemann et ses collègues du groupe communiste républicain citoyen madame Cukierman excusez-moi. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec les APL, finalement, votre gouvernement a un un problème puisque ce pognon de dingue comme vous l'aviez qualifié serait effectivement mieux employé à financer les cadeaux aux plus riches, en effet, après la baisse de 5 euros, nous avons encore un bel exemple avec cet exercice budgétaire puisque c'est une économie de que ce gouvernement s'apprête à faire sur le dos des plus fragiles, grâce à la réforme dite de la contemporain n'a été si nous pouvons discuter du principe de mieux coller aux ressources des allocataires, comment ne pas voir que la seule finalité de cette évolution, c'est de faire des économies, selon les différentes projections environ 1,2 1000000 d'allocataires devraient ainsi voir le montant de leur être diminué et 600000 pourraient même voir la prestation supprimer les premières inquiétudes se portent notamment sur la situation des jeunes et en particulier ceux de moins de 25 ans, qui ne sont pas éligibles aux minima sociaux tels que le RMI, le RSA et pour qui les APL constitue un véritable filet de sécurité, ce qui justifie le dépôt de notre amendement permettant l'instauration d'un régime transitoire nécessitant de remèdes 700 millions au compte des aides au logement, en effet, les conséquences de cette réforme sont dramatiques, dans une note transmise à Capital, l'Union nationale pour l'habitat, des jeunes, a ainsi calculé qu'un jeune isolé de moins de 25 ans entrant dans la vie active avec un revenu autour de 750 euros et payant un loyer de 400 euros touche actuellement 366 euros d'APL, avec la réforme, au fil des revalorisations trimestrielle successives de ces aides, il ne percevra plus que 165 euros, au bout d'un an son taux d'effort passera alors de 6 à 31 alors même que ce sont les jeunes qui sont les plus frappés par un taux de pauvreté, comment ne pas avoir qu'une telle réforme incarne encore un mépris de dingue à l'égard de notre jeunesse, nous souhaitons donc, à l'instar de ce que proposent les associations qu'un dispositif soit mis en oeuvre pour que les jeunes conserve la sécurité des APL, alors qu'il se lance dans la vie et ne voit pas fondre comme neige au soleil, leur pouvoir d'achat. Merci l'amendement 593 rectifié oui s'il est présenté par notre collègue, Monsieur Touraine, vous avez la parole.

l'instruction des APL, il n'en reste pas moins alors au-delà du mot, mais nous sommes dans un nouveau monde et par conséquent il y a beaucoup de mots, on a entendu énormément tout à l'heure. J'ose dire que le résultat de tout le discours, c'est quand même qu'il y a moins de construction et qu'il y a beaucoup plus de personnes qui en ont besoin. Pour l'APL, ça a des conséquences qui peuvent, qui peuvent être nocifs, ça a été développée, il y a quelques instants, je n'y reviendrai pas, ne pas oublier. Que. Pour un tiers des jeunes, ils n'auront leur 1er emploi qu'au bout de 6 mois. La moitié, au bout d'un an. Et que non, ils y resteront 6 mois où ils y resteront un an et il leur faudra en moyenne de 3 à 4 mois pour trouver le 1er emploi, c'est dire qu'il leur faut être extrêmement mobile, trouver des des logements là où l'emploi peut leur être procuré et par conséquent, il leur faut aussi des ressources parce que tout ce qui est à noter, c'est que le 1er salaire sera un salaire extrêmement bas, par conséquent, il serait utile de maintenir un régime dérogatoire que le mode de calcul utilisées pour l'ensemble de la population ne soit pas applicable aux étudiants, ils sont déjà 25 pourcent vivent dans la précarité et 25 pourcent des jeunes de 18 à 24 ans, vivent dans la précarité, donc il faut les aider à trouver leur 1er emploi les aider à être mobile et par conséquent la proposition qui est faite, c'est de dire, d'une part qu'on utilise l'ancien système qui leur permet d'avoir un temps un petit délai d'un an, voire un an et demi, peu d'adaptation et d'autre part d'instituer un minimum pour que ça ne descendent jamais en dessous d'une certaine somme qui se qui deviendrait dans ce cas, dérisoire et ne les aiderait pas du tout, voilà, c'est l'esprit de l'amendement qui est déposé, qui correspond à un certain nombre de ceux qui ont été présentés. Merci l'amendement 641 n'est pas défendu. Le 714 rectifié monsieur Bovary. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, cet amendement propose de limiter les pertes d'être personne et le logement pour les jeunes entrant dans la vie active avec de petits salaires, du fait de la mise en oeuvre et de la réforme de la contemporanéité de l'APL, les moins de 25 ans n'ont aucun filet de sécurité apparenté au RSA pour conforter leurs moyens d'existence, les aides personnelles au logement ont une fonction assurantielle forte pour celles et ceux qui se lancent dans un processus de décohabitation en lien avec la formation ou l'entrée dans la vie active, aussi il est important de maintenir un régime dérogatoire au bénéfice des moins de 25 ans, sans pour autant remettre en cause le principe d'une appréciation contemporaine des ressources, l'idée est de définir un dispositif de maîtrise de la baisse du montant de l'aide au logement d'une actualisation à l'autre pour le public cible et que le montant de l'aide au logement ne puisse être inférieur de plus de 20 pourcent au montant de l'aide perçue avant la dernière actualisation cette solution ne va ainsi pas à l'encontre du principe de contemporanéité de l'aide cet amendement tend par conséquent affecté 300 millions d'euros de l'action 12 du programme 177 hébergement parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables à l'action 01 du programme 109 aide à l'accès au logement. Merci l'amendement 594 qui fit et Monsieur Touraine. Oui, Monsieur le président, c'est un amendement qui ne diffère du précédent que sur un seul point : il s'agit d'un amendement de repli qui exige l'inscription d'un crédit supplémentaire de 300 millions au au au lieu de 700 millions compte tenu du fait que, il propose de de ne pas à adapter ou ne pas mettre en place un plancher pour les étudiants c'est sachant que nous raisonnons dans une enveloppe et que toute demande de crédits supplémentaires compte tenu des règles qui s'imposent aux parlementaires doit être, doit trouver un gage et ce gage, il n'est pas forcément populaire et il n'est pas forcément d'ailleurs justifié compte tenu de l'importance des autres politiques mais c'est un appel au gouvernement pour trouver les fonds nécessaires pour régler ce type de situation qui est particulièrement injuste et qui pourrait être douloureux pour des étudiants qui ont déjà suffisamment de difficultés. Merci l'amendement 703 monsieur roule présente. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, l'Agence nationale de la cohésion des territoires verra le jour le 1er janvier 2020 la raison d'être de l'institut ne peut se résumer à la seule aune rationalisation du paysage administratif, à un changement de culture certes cela est bien nécessaire pour assurer de manière Agile, la coordination et l'efficacité des politiques publiques sur nos territoires, ainsi que pour leur apporter une réponse cohérente de l'État dès le départ, le groupe RDSE a voulu inscrire dans son génome que l'agence favorise un accompagnement de proximité et c'est bien ce type qu'elle est très attendue dans les territoires qui, par leur taille et leur enclavement ne peut se doter de moyens d'ingénierie, or le projet de la loi de finances 2020 prévoit un financement de l'État limité à moins de 50 millions d'euros en AE et CP dans 10 millions d'euros dédiée à l'ingénierie territoriale à ce qui était suffisant pour venir à un soutien des collectivités territoriales et leurs groupements en tenant compte de leur particularité, là c'était ne doit pas constituer uniquement un outil de redéploiement des moyens existants, celui qui ne correspondraient pas aux attentes des élus porteurs de nombreux projets qui craignent risque d'asymétrie entre l'action urbaine de l'agence et son action au détriment de cette dernière, les programmes territoire d'dénutris Action coeur de ville petite centralité l'agenda rurales la couverture numérique du territoire ou encore la transition énergétique sont autant de défis à relever sur la sous-utilisation de fonds européens, en France, nous serons se livrant à la recommandation de la mission d'information sénatoriale qui propose de doter l'agence de moyens supplémentaires pour permettre de les mobiliser l'enveloppe de 10 millions d'euros dédiée à l'ingénierie ne peut donc correspondre à ses exigences, le présent amendement vise inconséquent à apporter le financement de l'agence, un peu moins de 150 millions d'euros en abandonnant son budget de 100 millions d'euros pour permettre à la fois de renforcer les moyens en ingénierie et un effectif comme nous sommes au contraire en matière de recevabilité financière et uniquement dans ce seul objectif cet abondement est financée, à due concurrence par des transferts de crédits issus du programme 135. mon numéro 5, monsieur le Président d'alliés au nom de la commission des finances. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, nous voilà sur un autre sujet : les 50 millions dont je parlais en discussion générale visant à rétablir la paix, l'accession.

et auquel notamment, il peut se trouver qu'un bailleur social leur propose d'acquérir leur logement, puisque c'est une politique que vous encourager la vente du logement social les premiers bénéficiaires, ce sont bien évidemment ceux qui habitent ces logements sociaux l'APL accession pour cela en tous les cas, mais pas forcément que pour cela était utile et voilà pourquoi, pour un coût de 50 millions, ce qui est relativement modeste, nous proposons son rétablissement. amendement 422 notre collègue suédois. anciens situées en zone détendue avec une enveloppe de plus de 700 millions l'APL accession permet à plus de 450000 ménages modestes d'acquitter une partie de leurs mensualités afin d'acquérir leur logement or très nombreux sont les projets d'accession qui sont remis en cause en l'absence de cette aide, donc l'amendement vise à augmenter de 50 millions les autorisations pour pouvoir rétablir l'APL accession pour tous, logements, neufs ou anciens, sur l'ensemble du territoire sur l'hypothèse de 30000 nouveaux ménages aidés, le coût annuel pour les finances publiques et de 50 millions merci. L'amendement ça sur 91 Madame Artigalas la parole. Merci monsieur le président, notre amendement est le même que celui que les 2 précédents mais je voudrais quand même insister sur le fait que l'APL occis accession à vocation à soutenir des ménages aux revenus modestes dans les zones détendues, particulièrement dans les centres bourgs et parfois dans des zones où il n'y a pas d'offre locative adaptée pour ces familles, dans beaucoup de cas, le projet d'acquisition n'aurait pas pu être possible sans le soutien de la le soutien de l'APL accession qui intervient comme un réel déclencheur l'APL accession est souvent nécessaire, nous l'avons sous-beaucoup vu pour conforter un prêt aidé pour les ménages, du 1er quartier là le permet de réduire d'un quart les mensualités de remboursement, la suppression, voulue par le gouvernement, une atteinte bien contre-productive car elle a pour effet de bloquer la mobilité des ménages les plus modestes, et elle n'est pas non plus cohérente avec des objectifs du président de la République pour vendre 40000 logements sociaux à leurs locataires, il faudra accompagner les ménages car, pour la plupart, ils n'en ont pas les moyens, l'APL accession hé bien de nature à accroître la mobilité dans le parc social et de faciliter la vente des logements HLM à leurs locataires, c'est pour ça que nous vous demandons de voter cet amendement. L'amendement sur 18 Madame Lienemann. Oui, c'est le même et nous voterons donc celui de monsieur Dallier, qui est le 1er qui mène depuis des années une bataille là-dessus, je voudrais insister sur le fait que globalement l'accession sociale dans ce pays est en chute libre, c'est pour 2 raisons : l'augmentation des prix, mais aussi dans certains secteurs, la réduction qui a eu lieu du prêt à taux 0 et je me réjouis que l'Assemblée nationale, une fois n'est pas coutume et voté le maintien du prêt à taux 0 en zone B2 et C, c'est essentiel pour soutenir l'accession à la propriété sur ces territoires, reste que même avec ce dispositif, l'APL accession permet la solvabilisation de gens qui sont sans se surendetter pourront quand même accéder à la propriété et que c'est essentiel que le parcours résidentiel de nos concitoyens les plus modestes puissent être entretenu pour libérer du logement social et aussi pour répondre à leur aspiration, suis j'ai pas le l'enthousiasme de mes collègues sur l'usage de cette APL pour la vente des logements sociaux, parce que je vous invite, chers collègues, à lire le rapport de la Cour des comptes, qui met en évidence que la vente de ces logements sociaux n'a rien de, d'une bonne solution, s'agissant d'une façon de financer le logement social, néanmoins il y a des personnes qui veulent le faire si ça reste raisonnable, l'APL accession est un outil utile pour eux donc nous voterons cet amendement et nous avions déposé le même. Merci nous allons passer maintenant à l'amendement 704 rectifié. Monsieur Gold. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, donc il s'agit d'un moment d'amendement de repli par rapport aux précédents, un amendement de mon collègue Jean-Yves Roux, qui vise à abonder les crédits destinés à la haine, c'était de 50 millions d'euros supplémentaires, je vous remercie. Merci l'amendement 588 rectifié Monsieur Bigot. Créé à l'initiative du Sénat, l'Agence nationale de cohésion des territoires, annoncé par le président de la République en janvier 2000 en juillet pendant 2017 devrait être opérationnel au 1er janvier 2020, notre ambition initiale était de créer une structure légère dédiée aux territoires les plus fragiles, afin de les accompagner, de les outiller dans la mise en oeuvre et de leur projet : la création de cette agence devaient répondre à un besoin exprimé par les élus locaux de disposer d'un interlocuteur unique, capable d'apporter des solutions opérationnelles pour développer leurs projets de territoire le gouvernement a mis en place une agence d'État assez lourde résultant de la la fusion de 3 opérateurs, à savoir le le paraquat et l'Agence du numérique, il s'agit donc davantage d'un redéploiement de moyens quand l'ensemble des élus locaux attendaient des moyens nouveaux pour les territoires les plus fragiles, cette agence va par ailleurs fédérer de nombreux opérateurs publics via des conventions partenariales, notamment avec l'ADEME, le CEREMA Lana ou encore l'ANRU, elle devra en ou de soutenir des programmes comme Action coeur de ville et Maison France Services, le président de la République ayant annoncé que ces maisons seraient bientôt dans chaque canton de France afin de permettre aux Français d'accéder plus facilement aux services publics, concrètement, il sera demandé à l'agence de coordonner et d'animer des des programmes politiques, allant de la politique de la ville à l'agenda rural de mener à bien une mission de recherche et une prospection mais aussi d'avoir une capacité de projection dans les territoires afin de venir en appui à l'État déconcentrer et décentraliser en matière de mise en oeuvre de projets complexes, cela nécessite des moyens importants qui aujourd'hui ne sont pas mises en oeuvre, le budget de l'ANC était de 50 millions d'euros pour 2020, dont près de la moitié en fonctionnement, nous doutons fortement de la capacité de l'agence à remplir les fonctions qui lui sont assignées, seuls 10 millions sont prévus pour l'ingénierie de projet, ce qui paraît totalement insuffisant au regard des besoins et des attentes des territoires et notamment les territoires les plus fragiles que la c'était doit prioritairement, accompagner la mission agenda rural qui a présenté ses travaux en juillet dernier, préconisait la création d'un fonds d'amorçage de 150 à 200 millions d'euros pour soutenir les premiers projets, projets qui seront portées par la une, on est loin du compte, c'est la raison pour laquelle notre amendement demande la hausse des montants dédiés à la haine, c'était pour développer l'ingénierie des projets, il propose donc de donner à l'agence nationale de cohésion des territoires, les moyens d'impulser, de nouveaux projets et de donner de la crédibilité à ce nouvel outil au service des territoires en conséquence, il est proposé d'abonder les crédits de l'Agence de 10 millions d'euros sans faire supporter cet effort sur les autres programmes de la mission. La parole est maintenant pour l'amendement 705 au président. le coeur du réacteur de la une cité la nécessité, mes chers collègues, a été donc voté au Sénat en première lecture, et c'est le groupe de du RDSE, qui a porté, excusez-moi l'expression, pour des radicaux, mais sur les fonts baptismaux cette agence. Il est

une a ça il été plus forte et qui soit davantage tournée vers les, en particulier pour les petites, les territoires ruraux qui n'ont pas les moyens de se payer donc des bureaux et les cabinets d'études spécialisés. Merci monsieur le président, l'amendement 895 présenté par Monsieur Delcros, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, monsieur le président, Monsieur le mini-chers collègues, plusieurs intervenants avant moi ont évoqué la question de l'ingénierie territoriale, nous savons que c'est un enjeu majeur et que j'ai eu l'occasion de le dire, les écarts en matière de capacité d'ingénierie, de capacité de compétence de ressources humaines finalement cette source de de d'inégalités entre les territoires parce que c'est toujours compliqué de développer des stratégies territoriales d'aller capter des financements d'être réactif pour répondre à des appels à projets et qu'est ce qui se passe, finalement, ce sont les collectivités qui dispose des compétences humaines, des services et d'ingénierie qui vont capter ces ces financements, donc c'est un sujet qui est extrêmement important, c'est l'une des missions aussi principal de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est sur ce sujet-là que les élus locaux attendent des des résultats et une vraie valeur ajoutée à l'agence réjouissons et nous nous réjouissons que dans le cas de l'agence 10 millions d'euros, soit fléchée pour l'ingénierie territoriale il nous sommes cependant que des millions ce n'est pas suffisant, près de 900 EPCI en moins de 30000 habitants près de 3 un peu plus de 300 EPCI en moins de 15000 habitants, c'est vers ces intercommunalités là qu'il faut porter l'effort et donc nous proposons pour une première année de mise en Oeuvres de l'agence de porter le montant des crédits dédiée à l'ingénierie territoriale à 20 millions d'euros, donc 10 millions supplémentaires par rapport à ce qui est proposé dans le texte. Merci l'amendement 595 rectifié monsieur Bourquin présente. gouvernement, chers collègues, le gouvernement a présenté dans le cas de la stratégie nationale de prévention et de lutte conte la pauvreté des mesures pour moderniser la délivrance des prestations sociales et lutter contre le non-recours aux droits. Et dans ce cas la domiciliation administrative est un droit essentiel dont la mise en oeuvre, il conditionne l'exercice effective de l'ensemble de leurs droits, le nombre d'élections domiciliation a connu une hausse significative une hausse régulière qui se concentrent en partie dans les zones urbaines et faute de moyens et de soutien des pouvoirs publics dans l'exercice de leur mission des organismes sont aujourd'hui saturés sont contraints de refuser des domicilié des personnes en situation de précarité d'amendement suggéré par les acteurs de la solidarité comme Emmaüs ou encore le Secours catholique propose d'abonder le budget de la mission cohésion des territoires à hauteur de 10 millions d'euros pour financer les organismes de domiciliation dans l'exercice de leur mission et ainsi garantir l'accès aux droits des personnes en situation d'exclusion, monsieur le Ministre. Je voudrais attirer votre attention sur la gravité de la situation. Du nom de sans abris qui meurent aujourd'hui je met en eu. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur une dernière étude qui disait qu'avec la baisse des APL qui disait aussi qu'avec la situation et bientôt sur la loi qui ne va pas manquer à produire des effets extrêmement négatifs sur la le chômage, hé bien il faut prendre des mesures et ces mesures sont demandé avec force par les associations caritatives et ses 10 millions dans ce budget ne sont pas grand-chose mais on peut éviter des drames sociaux.

l'absence d'adresses constitue à l'évidence une entrave à l'exercice des droits civiques, civils, sociaux pour un trop grand nombre de nos concitoyens, ça ne vaut 1000 si le stable, soit près de 141500 personnes sans domicile et 85000 vivant au sein de l'habitation informel, malgré les efforts consacrés par les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, il est ainsi que les organismes agréés le nombre encore élevé de demandes de domiciliation entraîne des refus lorsqu'il s'agit d'un droit opposable en vertu de la loi Dalo du 5 mars 2007, les personnes concernées sont ainsi éloigné de toute démarche administrative permettant de mener une vie normale, le présent amendement 706 procède donc à une augmentation de 10 millions de crédits consacrés aux associations et notamment au dispositif de veille de veille sociale, voilà l'esprit de cet amendement que je vous propose d'adopter. Merci l'amendement 719 Madame Lienemann le présente, vous avez la parole. C'est le même amendement que mes collègues qui ont très bien plaider cette cause expliquant que quand on ne domicile ils pas les gens, ça ne peut qu'accroître la marginalisation et la difficulté à retrouver sa place dans la société, moi je voudrais mais on ne je crois qu'on en est tous conscients de d'observer une première chose, le président de la République avait dit qu'il aurait pu, de personnes dans la rue, à la fin de son mandat, force est de constater, on pourrait comprendre qu'on règle pas ses problèmes d'un coup de baguette magique et du jour au lendemain, mais là c'est l'inverse qui se passe, ça s'accroît et les raisons de cet accroissement sont nombreux, notamment l'augmentation de la pauvreté, le 2ème accroissement c'est celui des expulsions locatives, le mécanisme pour éviter les expulsions locatives n'est pas opérants et nous le savons aussi l'arrivée de population dans notre territoire, moi j'ai l'intime conviction que si notre pays veut être a minima à la hauteur de cet objectif d'éviter qu'il y a, je ne crois pas 0 SDF mais suffisamment de gens qui ne soit plus du tout dans la rue, il est fondamental de reprendre à 0, un un plan de programmation pour voir comment, territoire par territoire, on est en situation de régler ce problème, vous avez dû lire comme moi dans le monde d'hier qu'il y a maintenant des nouveau-nés. Qui sont dans la rue. à quelques semaines après leur naissance. Croyez-vous que ce soit digne de la France, alors moi je veux bien qu'il ait des tas de problèmes qu'on trouve qu'il y a les problèmes des crimes migration etc, néanmoins ils sont ici, ils sont nés en France, ils méritent d'être traités dignement et donc il faut reprendre à 0 ce dossier, mais pour l'heure, la première des choses à faire, c'est d'éviter les mesures qui appauvrissent les gens et la 2ème raison la 2ème mesure à prendre 7 mètres les crédits pour qu'avec les associations, on puisse réussir leur réinsertion. Merci l'amendement 616 rectifié, madame Guillemot. Si Monsieur le Président, ce présent amendement qui a été donc voté à une très grande majorité, par la commission des affaires économiques visent à rétablir les crédits de paiement dévolu au financement de l'ANRU tels que le gouvernement s'est engagé à les verser au cours du quinquennat en juillet 2018, le président de la République a en effet réaffirmé l'engagement de l'État d'apporter un milliard d'euros dans le cas du doublement du NPNRU, soit 200 millions d'euros durant ce quinquennat or dans le projet de loi de finances, seuls 25 millions d'euros sont inscrits au lieu des 35 millions qui étaient, selon les réponses au questionnaire budgétaire, il s'agirait d'une volonté explicite de l'État de limiter désormais sa contribution à 25 millions d'euros par an sur la période 2020, 2022 ainsi si rien n'était changé la contribution de l'État sur le quinquennat plafonnerait à 115 millions d'euros au lieu des 200 millions d'euros promis remettant à après 2022 le gros de ces versements et la réalisation de ses engagements, l'effort sera donc porté par les bailleurs sociaux et Action Logement, ce sera d'ailleurs le cas dès 2020, où seront appelés 96 millions d'euros sur les 220 millions d'euros de la marge pluriannuel quinquennal mise à disposition par Action logement, rappelons que dans le même temps, les crédits de la politique de la ville sont en recul de 10,5 millions d'euros, ceux du logement, de près de 1,4 milliards d'euros, il est incompréhensible que l'État ne tienne pas ses engagements, alors que même les bailleurs et les partenaires sociaux sont lourdement mis à contribution et verse comme prévu les sommes dues, c'est un signal très négatif au regard de l'urgence des besoins dans les quartiers prioritaires et la nécessité débloquer au plus vite et si possible par avance les moyens financiers pour mettre en oeuvre les projets qui ont été validés par l'ANRU au cours de l'année, rétablir ces crédits dévolus à l'ANRU selon la programmation arrêté donc pour nous une question de principe et d'urgence dans les territoires. Merci, amendement 707 rectifié. Madame Coste présente. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la nouvelle baisse des crédits consacrés à la prime d'aménagement du territoire réduite progressivement fait craindre sa disparition, à terme, la loi de finances pour 2015 consacré 29,6 millions d'euros en autorisant, ancien d'engagement le présent projet de loi de finances n'y consacrent que 6 millions d'euros, soit 5 fois moins en l'espace de 5 ans pourtant, cette aide directe à l'investissement, l'investissement a démontré son intérêt et son efficacité dans l'accompagnement des entreprises et la création et le maintien de la d'emploi dans les zones les plus fragiles de notre territoire, nous, nous nous ne réduisons pas à néant un outil utile au renforcement de l'activité de l'attractivité des territoires, le présente, avant même vise à abonder de 9 millions d'euros supplémentaires, l'enveloppe consacrée à la afin de la porter à 15 millions d'euros en 2020, soit la moitié de ce qui était consacré en 2015, je vous remercie. nous passons à l'amendement 617 rectifié madame Estrosi Sassone. Merci madame la présidente, alors cet amendement a été voté très largement je crois la à l'unanimité par la commission des affaires économiques et il vise à augmenter d'un Euro le forfait journalier des pensions de famille, actuellement fixé à 16 euros par jour et par personne accueillie ce forfait n'a pas été réévalué depuis 2008, s'il avait été indexé sur l'inflation, il serait fixé aujourd'hui à 19 euros un rattrapage est donc nécessaire, cet amendement a pour but de l'amorcer les pensions de famille sont au coeur de la politique de logement adaptés que vous défendez monsieur le ministre, en créant d'ici 2020 22500 pension de famille, il s'agit de structures de petite taille, comportant une vingtaine de logements combinant logements privatifs et espaces collectifs, elles sont destinées à l'accueil, sans limitation de durée des personnes en forte exclusion sociale, forme de logement autonome, elles offrent un cadre de vie, convivial et chaleureux, grâce à la présence au quotidien donne autre elle permet également la réadaptation à la vie sociale et elle vise à faire retrouver durablement tous les aspects de la citoyenneté à des à des personnes en situation de grande exclusion mais aujourd'hui pour atteindre pleinement les objectifs fixés en termes de réinsertion et vous l'avez encore rappelé : Monsieur le Ministre dans votre intervention, il convient de donner plus de moyens à l'accompagnement social et de rehausser progressivement le forfait de prise en charge la politique du logement d'abord et de réinsertion par le logement ne peut réussir que si l'accompagnement social est au rendez-vous et cela à une hauteur suffisante, c'est la raison pour laquelle je crois que nous pouvons tous nous retrouver autour de cet objectif que je vous présente dans cet amendement je souhaiterais profiter encore du temps qui me reste pour vous dire qu'il serait important, Monsieur le Ministre, véritablement, de pouvoir bénéficier de véritables données sur le nombre de personnes sans domicile dans notre pays, en effet, depuis, des enquêtes à la fois de l'INS et de l'INED, qui ont date de 2012, il n'a jamais été réalisé de véritables études pouvant nous dire combien de personnes aujourd'hui sont sans abri les publie pays, or il s'agit là d'une véritable politique publique que nous devons accompagner avec des mesures efficaces mais encore faut-il avoir de véritables données. Merci, nous avons maintenant 3 amendements identiques, nous devons d'abord l'amendement numéro 7 rectifié monsieur Delcros. Oui merci madame la présidente, plusieurs sénateurs ont déjà évoqué la question de la prime à l'aménagement du territoire et ma collègue Josiane Costes a rappelé tout à l'heure, l'importance qu'elle qu'elle qu'elle avait dans les territoires les plus fragiles, on n'est pas sur des sommes. Très importante, on est en train de parler encore une fois, de quelques millions d'euros, mais on sait que l'effet levier dans les territoires pour soutenir les entreprises et donc soutenir l'emploi et du coup la dynamique économique extrêmement importante et donc cette prime à l'aménagement du territoire en 2019, elle était à 10 millions d'euros aujourd'hui, il est proposé 6 millions d'euros, ce qui ne veut plus dire grand chose, vous vous en pensez-vous le Conseil et donc nous proposons au nom de la commission des finances je, je tiens à le dire, nous proposons cette les crédits dédiés à la prime à l'aménager un territoire soit rehaussé au niveau de 2019, c'est à dire 10 millions d'euros, de vraiment prendre en considération ce sujet, on est en train de parler 4 millions d'euros, mais qui sont importants pour les territoires ruraux, donc je demande vraiment de voilà, de faire preuve de bienveillance sur ce sujet-là, comment je vais dire ça de ne pas conforter le sentiment perçu parfois d'abandon des territoires ruraux, je vous remercie. Merci, nous passons à l'amendement 520 monsieur de Nikolaï. Oui merci madame la présidente, monsieur le ministre, au nom de la commission du développement durable, je soutiens à travers cet amendement la position aussi de la commission des finances sur notre volonté de voir rêver l'inscription budgétaire à 10 millions d'euros pour la prime d'aménagement du territoire, je crois que, une fois de plus, si ça n'était pas le cas, les territoires ruraux qui ont souvent des difficultés pour accueillir des investissements d'entreprises importantes, et Dieu sait s'ils en ont besoin, je crois que les territoires ruraux, une fois de plus, on montrerait qu'ils ne sont pas entendus de la part du gouvernement et qui serait laissée à l'heure à simple appréciation, je crois que Monsieur le ministre, nous comptons beaucoup sur vous pour faire en sorte que, il y a un signe fort donné au développement économique de nos territoires. Merci, nous passons à l'amendement 587 Monsieur Joël Bigot. et dont les effets sont évalués de façon très précise, chaque année, c'est un effet de levier qui conduit chaque année à créer ou à maintenir des emplois et donc se présente le présent amendement vise à ce que c'est, pour que cet outil reste efficient qu'on puisse augmenter de 4 millions d'euros, le budget de la prime d'aménagement du territoire pour éteindre les 10 millions au total en 2020, cet outil est vraiment important pour les territoires. Merci, nous passons à l'amendement 726 rectifié madame Jasmin. Merci madame la présidente. La mission cohésion des territoires prévoit les crédits budgétaires du plan encore l'icône 3 dont l'objectif est de réduire l'impact de l'Exposition des populations de Martinique et de la Guadeloupe au chlordécone le budget alloué à ce plan pour 2020, elle est seulement de 3 millions d'euros, soit un 1000000 supplémentaire environ par rapport à 2019 qualifiée de scandale environnemental, la lutte conte la pollution du chlordécone mérite d'engager bien plus largement la responsabilité de l'État dans la réparation du préjudice subi par la population, la commission d'enquête parlementaire présidée par le député Serge Letchimy et initiée par madame Vainqueur Christophe Hélène député suite à son rapport il sur la proposition de loi, le rapport du mardi 26 novembre avec les 49 préconisations propose justement que des tests 3 aux populations la Commission considère l'État comme le 1er, responsable de cette pollution, pour avoir autorisé la vente de ce produit pendant des années en tout six qu'on connaissance de cause, elle préconise également la mise en place de dépistage pour toutes les populations vulnérables et des mesures de traçabilité de tous les produits alimentaires issus des circuits formel et informel dans les 3 années à venir ces recommandations devront souscrire dans le 4ème plan prévu en 2020, mais en attendant nous ne pouvons rester insensibles et attentiste pendant le temps de la concertation prévue pour le plan en 2021 aussi, il est proposé par cet amendement, une prise en charge gratuite du dépistage de la population du taux de chlordécone dans le sang : actuellement, le dépistage coûte entre 80 et 140 euros et ce n'est pas remboursé, il apparaît donc préalables à ce à cette politique publique d'envergure que l'État prenne en charge intégralement et gratuitement ce dépistage de l'ensemble des personnes en lice en lançant une grande campagne de dépistage sur les territoires concernés, je vous remercie. Merci alors. Nous allons maintenant solliciter l'avis de la Commission pour l'ensemble de ces amendements. Monsieur le rapporteur. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons quand même une difficulté parce que nous avons 24 amendements en discussion commune sur des sujets. Complètement différent, certains me concerne en tant que rapporteur d'autres : Bernard Delcros, donc on voit bien que les sujets ne sont absolument pas les mêmes, mais ils sont en discussion générale parce que. On déshabille Pierre pour habiller Paul, et comme beaucoup des habits le même Pierre effectivement si un amendement a été adopté il y a le risque qu'il fasse tomber tous les autres, voilà pourquoi nous sommes en discussion commune, ceci dit, ça pose un un vrai problème parce que je vais être amené à donner, comme Bernard Delcros des avis sur des sujets très différents, mais la discussion, point par point, je ne sais pas trop comment elle peut s'organiser, voilà, c'est une vraie difficulté qu'on ne rencontre pas que sur cette mission, mais là je crois qu'on est dans le dans le le paradoxe le plus absolu. Alors je vais commencer par les amendements 723 593 rectifié bis le 641 n'a pas été soutenu le 714 rectifié et 594 rectifié. Ces amendements concernent la mise en place de la réforme de la prise en compte des ressources des allocataires de l'APL alors rappelons d'abord qu'on ne touche pas aux règles de calcul, on ne fait que changer effectivement les ressources qui sont prises en compte et un point de sémantique quand même si déjà contemporaniste c'est difficile à dire, et ça n'est pas très correct par rapport à ce que nous allons faire temps réel, Monsieur le Ministre, encore pire, parce que pour moi le temps réel, ça serait prendre les revenus du mois précédent pour calculer l'APL du mois suivant sa ça serait du temps réel, au sens où les informaticiens excusez mon métier revient mais ça serait du temps réel, là ce que l'on fait, c'est qu'au lieu de temps les revenus et moins de on prend sur les 12 derniers mois glissants et tous les 3 mois on recalcul, donc c'est mieux que rien de moins de mais ça n'est pas tout à fait contemporain et encore moins temps réel. Alors d'abord un mot sur le le principe de la réforme est ce qu'elle est juste pas juste, chacun peut avoir son point de vue, première chose qu'on peut dire que c'est à coup sûr une une réforme de rendement budgétaire puisqu'elle va rapporter grosso modo 1,2 ou 1,3 1000000. Ce que, dans tous les cas de figure, ce que nous allons faire est effectivement juste dans certains cas, à l'évidence, par exemple, un jeune et tu un étudiant qui bénéficient des APL qui trouve un job bien payé ou très bien payés qu'on calcule, effectivement les APL sur ses revenus les plus contemporains, c'est normal et donc effectivement, enfin c'est normal oui c'est normal et donc dans ce cas-là, il y a strictement rien à dire que vous disiez monsieur le Ministre que parce que c'est toujours pareil, c'est un peu comme sur la réforme des retraites, on a toujours à à la tendance à présenter que les cas favorable, il y a aussi les cas Fabre vous disiez une femme qui est seule avec un enfant qui voit ses revenus chuter elle étaient obligés d'attendre effectivement non, monsieur le Ministre, il y avait 2 cas de figure effectivement où on pouvait faire réactualiser l'APL, il y avait le cas de longue maladie et, le cas du chômage où là il y avait un abattement possible de 30 pourcent sur les revenus et moins de donc, il y avait déjà un mécanisme qui permettait de faire réévaluer ce n'est pas l'équivalent du système actuel, mais il y avait déjà un mécanisme là ce que je crains mais nos collègues évoquent des sujets différents, c'est qu'effectivement, pour les publics les plus précaires, ce qui effectivement vont être à la limite du seuil et qui vont peut-être une fois et trop dessus une fois en dessous avant le tourniquet, c'était une fois par an. mais il y avait une certaine prévisibilité. Là on va avoir un tourniquet tous les 3 mois et je crains effectivement que cette mécanique là sans autre effet de lissage que celui qui existe avec la prise en compte des revenus sur 12 mois glissants, je crains qu'effectivement on est une nouvelle trappes à inactivité parce que quelqu'un qui prendrait des heures supplémentaires pendant 2, 3 mois ou quelqu'un qui prendrait un contrat pendant une période courte notice pose la question de l'impact sur les APL, 3 mois après, et je pense que les gens vont se la poser la question, alors maintenant il y a des amendements qui propose un changement de règles de calcul pour prendre en considération les cas particuliers, notamment les jeunes. Il y a 2 questions à se poser avant de donner un avis, l'impact budgétaire, alors certes, on a des amendements à 700 millions des amendements à 500 millions à 300 millions. ça n'est pas rien, même si la règle des 3 pourcent est un peu moins prégnante en ce moment, mais ça n'est pas rien. Mais il y a un 2ème problème que je vais aussi soulevé. Quelle capacité, avons-nous à modifier les règles du jeu pour le 1er janvier 2019. Quand on sait que l'enjeu principal de cette réforme et on l'a bien constaté l'an dernier, puisqu'elle devait entrer en application à la mi-2019 à 100 septembre 2019, et puis finalement devant le danger que représente, j'allais dire, cette modification importante, on a reculé au 1er janvier 2019 moi je pense qu'on est pas capable en souffrent, qu'est que Monsieur le ministre me disent le contraire, mais je pense qu'on est pas capable de mettre en oeuvre un changement comme celui-là dans les semaines qui viennent, donc moi je ne peux pas donner un avis favorable sur ces amendements pour ces 2 raisons, mais Monsieur le Ministre, je suggère fortement que vous regardiez les effets de bord de votre réforme pour ceux effectivement qui risque de faire le yo-yo une fois au-dessus, une fois en dessous avec l'impact que sa voix à voir. Donc, je suis au regret, mes chers collègues, mais de donner un avis défavorable sur l'et 1, 2, 3, 4, 5 premiers amendements jusqu'aux 594. Ensuite, les 4 suivants, enfin il y en a trois identique au mien, rétablissement de l'APL accession, pas de commentaire supplémentaire. Je vais passer la parole à Bernard Delcros pour les faire dans l'ordre, madame la présidente. Oui, c'est 700. 703 rectifié si voilà, monsieur le rapporteur. Oui merci, donc cet amendement concerne une fois de plus, l'ingénierie qu'apportera l'agence nationale de cohésion des territoires ce et les crédits dédiés à la chanson, je le rappelle, de 49,7 millions d'euros dans 10 millions pour l'ingénierie, nous sommes d'accord pour dire qu'il faut rehausser un peu les crédits à l'ingénierie mais cet amendement propose d'augmenter de 5 millions d'euros. les crédits dédiés à l'agence et notamment l'ingénierie, donc ça ne sent pas être au niveau de la commission des finances, le bon niveau pour une première année de mise en oeuvre et donc la commission proposera un amendement pourrait au CAA de 10 millions donc porter à 20 millions et je vous demanderai de retirer cet amendement au profit de celui de la commission si vous allez d'accord.

alors sur les amendements 595 rectifié Terre 706 rectifié. Et 719 moi j'en ai 3, madame la présidente. Ah non, il y a 616 pardon. Qui va avec. 422 591 et 78. Je ne peux que donner un avis favorable parce que c'est le même que celui de la commission des finances, je suis désolé, j'étais un peu perdu. Il vont donc favorable pour l'ensemble. excusez-moi au 595 rectifié terre. On essaie de les balayer dans l'ordre et j'ai présenté les 5 premiers, puis les quatre suivants : Bernard Delcros, a pris la suite.

reste, c'est très compliqué, vous l'avez bien évoqué tout à l'heure donc, si nous pouvons les prendre dans l'ordre, ça sera beaucoup plus sympa, on va et puis il y a aussi. Donc, le 704 c'est l'amendement de notre collègue monsieur Roux toujours c'est les crédits d'ingénierie et propose de les rehausser de 50 millions d'euros, donc passer de 10 milliards 50 millions je lui propose le retrait de cet amendement au profit de celui de la commission, ensuite, on a l'amendement proposé par Joël Le Bigot et un certain nombres de collègues sénateurs qui propose de rehausser les crédits de 10 millions à 20 millions d'euros, donc c'est un amendement identique à celui de la Commission, donc évidemment un avis favorable ensuite l'amendement de notre collègue, Jean-Claude Requier et de plusieurs sénateurs de son groupe, qui propose également de rehausser les crédits à hauteur de 10 millions d'euros, donc identique à celui de la commission, je n'ai jamais un avis favorable et enfin de l'amendement de la commission que que je propose, qui est de doubler les crédits dédiés à l'ingénierie territoriale, ça me semble être le bon niveau pour une première année de mise en oeuvre et là aussi, Monsieur le Ministre, je vous demanderais beaucoup de bienveillance sur sujet extrêmement important dans les territoires ruraux. Monsieur le rapporteur, donc simplement pour être très clair : l'amendement 588 rectifié, vous avez un avis favorable n'est-ce pas. Les 3 sont identiques : voilà, c'est-à-dire celui de la Commission et les 2 précédents dans évidemment c'est un avis favorable

Présenter trop tôt les amendements sur l'APL accession alors maintenant 3 à 3 amendements identiques ou quasiment 595 rectifié Terre 706 rectifié et 719 qui propose effectivement d'abonder de 10 millions les crédits du programme 177 afin de financer les associations qui porte les dispositifs de veille sociale, alors c'est vrai que le sujet qui est évoqué est un vrai sujet, mais mes chers collègues, je rappellerai quand même que les crédits en question sont passés de 126,5 millions en 2018 à 134,2 millions en 2000 19 et à 148,4 millions pour le projet de loi de finances 2020, ce qui fait une augmentation de 22 millions d'euros sur 3 exercices budgétaires, ça n'est pas rien, donc je pense effectivement que, il y a là un effort significatif et que nous pourrions peut-être nous en tenir là. Donc ça serait un avis défavorable. L'amendement numéro 616 rectifié de madame Guillemot, là on est sur le sujet de l'ANRU. Alors je peux comprendre l'argumentaire politique de notre collègue qui souhaiterait que l'État montre. Ces affaires écho au nom du rapport. Au nom de la commission des affaires, pas de problème. La commission des affaires économiques, souhaiterait, effectivement, j'allais dire, faire plus un geste politique qu'un geste budgétaires et techniques, la question est de savoir si oui ou non l'ANRU aura encaisse sonnante et trébuchante, les moyens dont elle aura besoin pour financer ce qui va se réaliser au cours de l'année prochaine, là-dessus, moi je n'ai pas d'inquiétude, et je l'ai dit en discussion générale, on en reparlera en 2023 2024 parce qu'effectivement, sur le milliard d'euros que l'État doit apporter, on voit bien que l'essentiel viendra après ce quinquennat 2023 2024 et la question se reposera alors on peut souligner, je l'ai fait, mais de là à en conclure qu'il y a un risque que l'an prochain, on manque de crédits de paiement, moi je ne le crois pas, et c'est pourquoi je ne peux proposer qu'un avis défavorable. Maintenant, nous passons à l'amendement 607 rectifié ces pardon 707 rectifié bien sûr. Oui merci, donc cet amendement concerne la la prime à l'aménagement du territoire, dont on a beaucoup parlé, et nos collègues proposent de rehausser d'augmenter les crédits dédiés à la prime à l'aménagement des territoires de 9 millions d'euros, alors comme vous avez pu le constater, la commission des finances propose d'augmenter ses crédits de 4 millions d'euros pour les remettre au niveau de 2019 donc on propose un retrait de cet amendement au profit de celui de la commission. Merci, nous passons à l'amendement 617 rectifié. Alors au nom de la commune, mission des affaires économiques, alors d'abord, je précise que la commission des finances n'a pas pu examiner l'amendement, puisque dans un 1er temps, il avait été déclarée recevable et il a été repêché. Chers collègues, donner, je vais donner un avis à titre personnel, donc il s'agit effectivement de majorer 8 25 millions d'euros, les crédits du programme 77 hébergement parcours vers le logement et insertion des personnes. Vulnérables afin d'augmenter de 1 pourcent un Euro pardon le forfait journalier des pensions de famille, je pense que cet amendement est intéressant. Le financement des patients de ceux des pensions de famille est en effet passé de 8 à 12 euros par jour en 2005 puis à 16 euros de. Depuis le 1er janvier 2007 mais ce montant n'a pas été revalorisée depuis donc ça fait déjà à bientôt 12 ou 13 exercice budgétaire et nous pourrions effectivement décidé d'augmenter ce forfait d'un Euro, donc c'est un avis favorable de la commission est enfin pas de la commission des finances à titre personnel du rapporteur. Merci, nous avons ensuite 3 amendements identiques cette rectifié, je crois que, au vu de la complexité de l'exercice, les nécessaire de les nommer à ce moment 520 et 587. Voilà 3 amendements identiques qui concerne donc la prime à l'aménagement du territoire et qui propose de revenir au niveau de crédits affectés en 2019, c'est-à-dire 10 millions d'euros le l'amendement pardon, présenté par la Commission et les 2 autres pour Monsieur Nikolaï pour la commission de l'aménagement du territoire, le développement durable et ensuite notre collègue Joël Bigot, donc évidemment c'est un avis favorable sur ces trois amendements. Qui et nous passons dernier amendement l'amendement 726 rectifié. Le 726 rectifié concerne un autre sujet, il concerne en fait le programme 162 et l'action 8 je crois, du programme d'intervention territoriale de l'État sur le plan chlordécone cet amendement propose d'augmenter un peu les crédits dédiés au plan chlordécone 3 millions d'euros et sont prévues dans le texte qui nous est proposé et cet amendement propose de rajouter 2 millions d'euros pour porter les crédits à 5 millions d'euros, nous avons accès évidemment cet amendement en commission des finances on, ça a été rappelé tout à l'heure, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale ah est arrivé un certain nombre de conclusions, notamment la conclusion qu'il fallait en particulier améliorer les financements dédiés à la recherche sur le chlordécone, on est sûr vraiment sur un enjeu de santé publique aujourd'hui, la recherche est accompagné à moins de 100000 euros, c'est la raison pour laquelle, compte tenu de l'enjeu de santé publique sur ces territoires et la nécessité d'accroître les crédits, notamment en direction de la recherche, la commission des finances, et a, lui, favorable à cet amendement. Merci, alors Monsieur le Ministre vous saurais gré de de pouvoir nommer les les amendements afin de ne pas faire d'erreur sur la vie que vous allez émettre sur chacun d'entre eux. Merci, je vais tenter, merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, alors il y a plusieurs sujets qui sont abordés, je vais essayer d'avancer les idées simples vis-à-vis de ces amendements réparties de manière compliquée, le 1er sujet concerne la question des appels en temps réel, modulo le sujet de sémantique, soulignée par le rapporteur d'alliés, la question du principe de la réforme, je crois qu'il est extrêmement simple, c'est de se dire effectivement on va actualiser le calcul des appels en fonction de la situation et du montant que gagnent nos concitoyens au moment où on donne ces aides personnalisées au logement, concrètement, comment ça va se passer tous les 3 mois, on va regarder quels sont les revenus des 12 derniers mois et on va faire ça, ainsi de suite. C'est totalement nouveau puisque, auparavant, on prenait une photographie de quelle était votre situation il y a 2 ans, ça c'est le principe, ce qui veut dire, et j'insiste dessus, c'est que ça n'est en rien, en rien des modifications et monsieur le rapporteur Daniel à la, à juste titre juste type pardon dit en rien des modifications de calcul si votre situation était la même : il y a 2 ans par rapport à aujourd'hui votre niveau d'appel ne change absolument pas votre niveau d'appel ne change absolument pas si vous êtes étudiant, par exemple, quand vous êtes étudiant, ce sont des forfaits qui ne change absolument pas en revanche le 2ème élément, qui est le 3ème élément qu'il faut avoir en tête, c'est que dans ce système d'aujourd'hui, qu'est ce qui se passait bien, on allait prendre le revenu d'il y a 2 ans, et donc on mettait en place un nombre incalculable d'effets correcteurs et le rapporteur d'allier on a mentionné un quand par exemple il y a 2 ans, vous aviez un travail aujourd'hui, vous êtes au chômage, on prenait un élément correcteurs quitter ont considéré que votre chômage était égal considérer ça à 70 pourcent de votre revenu de salarié, mais ce qui veut dire que quand vous faites votre chômage était inférieur à ses 70 pourcent vous n'aviez pas le montant d'APL auquel vous devriez avoir le droit, et là je parle par exemple des chômeurs mais prenez un retraité de moins de 2 ans, on faisait le même système quand vous étiez jeune retraité. à ce moment-là, ont considéré que votre niveau de retraite était égale à 70 pourcent de votre dernier salaire. Et donc on calculez votre appel on considérant, vous aviez 70 pourcent de votre dernier salaire comme revenu alors que vous étiez jeune retraité mais plein de cassez pas la réalité et donc aujourd'hui ce qu'on fait c'est qu'on prend le niveau de pension et donc toutes les personnes par exemple et jeune retraité dont le niveau de pension est inférieure à 70 pourcent du dernier salaire, ce sont des gagnants dans la réforme, alors aujourd'hui j'entends, parce que beaucoup disent, mais c'est une réforme d'économie non, et j'insiste dessus cette réforme-là, elle fait des économies, dès lors que le chômage diminue, le jour où le chômage augmente, c'est une réforme qui est coûteuse parce que votre filet de sécurité votre filet et aider et des situations auxquelles vous êtes confrontés, je vais même à des plus loin parce que c'est des populations auxquelles il faut apporter un accompagnement très spécifique. J'ai parlé des étudiants, ça ne change rien, j'ai parlé des retraités, soit ça ne change rien, soit c'est bénéfique, j'ai parlé des personnes qui étaient en situation de salariat ou de chômage, ben c'est en fonction de l'évolution est-ce que oui ou non, vous avez trouvé un emploi,

quand vous étiez un indépendant, vous n'aviez pas accès au aux appels vous deviez attendre 2 ans avant d'avoir accès aux appels parce qu'on prenait en compte dans les mêmes forfaits, le fait ben probablement pendant les 2 premières années, vous gagnez tant il y avait un forfait qui vous excluez par là même des appels, c'était absolument scandaleux pour des personnes qui, aujourd'hui, d'ailleurs, souvent très jeunes, maintenant se lance vers l'entreprenariat auto-entrepreneur ou indépendants et l'autre exemple concerne les jeunes actifs, alors vous avez le cas des jeunes actifs évoqués par le rapporteur d'alliés qui est un cas réel ou dans ce cas-là, vous pouvez avoir moins d'appels que vous ne l'aviez avant mais songez aujourd'hui que dans le système si vous étiez un jeune actif qui avait les appels quand vous étiez étudiant c'est le cas évoqués par le rapporteur d'alliés, vous continuez à avoir les appels jusqu'au moment ou soit vous déclariez que vous aviez un emploi soit la CAF vous vous notifier que par vous êtes dans une situation d'emploi et donc on va adapter, mais si vous étiez un jeune actif qui n'avait pas d'appel quand il était étudiant. Parce que, et c'est souvent d'ailleurs des publics plutôt Pauvre que des publics parce que vous n'aviez pas les moyens de vous payer un logement parce que vous dormiez chez un proche, ah ben dans ce cas là, pendant 2 ans, même système des forfaits évaluatif vous n'aviez pas accès aux APL un jeune actif qui n'avait pas d'appel quand il était étudiant à quitté donc, primo demandeurs devaient attendre 2 ans avant d'avoir une APL mais ces systèmes ne pouvait pas être conforme la réalité et l'accompagnement auquel on doit donner alors le rapporteur Dali a tout à fait raison quand vous faites ce type de réforme, il faut veiller au maximum à limiter les effets de seuil et si vous avez des effets de bord, notamment la question de la mobilité, qui a été évoqué tout à l'heure, bah cette mobilité, il faut l'accompagner, c'est, c'est, par exemple, pour ça, que dans le plan d'investissement volontaire, on a mis en place ces prix mobilité qui concernent notamment. Les jeunes actifs, c'est très important j'aurais un avis défavorable sur les amendements, madame la présidente, 723 593 rectifié ensuite le 2ème, sujet qui a été très largement évoquée concerne l'agence nationale de cohésion des territoires sur les crédits accentué sur l'ingénieur il on a aussi ma position avec un avis défavorable ne va pas vous étonner, moi, ce que ce que j'ai j'ai. Piqué tout à l'heure à la tribune, c'est que aujourd'hui on a un montant un budget de l'Ordre de 50 millions d'euros et qu'en fait l'objectif de ce budget, c'est surtout pas de s'arrêter là, c'est d'aller prendre les forces vives qui de l'ANRU qui de l'Anaes qui ne l'Epareca qui de la mission France très haut débit qui la mission France Mobile de la mission Coeur de ville pour aller accompagner donner cet ingénieur il je crois véritablement que le fondement et d'ailleurs, la valeur ajoutée et d'ailleurs ça marchera ou ça marchera pas uniquement sur le volume d'ingénierie la une, c'était c'est un accompagnement d'ingénierie au bénéfice des élus locaux dans le montage de projets, je ne peux pas être plus clair, mais je pense qu'il faut voir si cette année ça marche ou pas avec eux, le budget de l'accompagnement que j'évoque, et puis on évaluera en fin d'année pour pourvoir. Effectivement, si on est au rendez-vous, ou pas, et, et, en ce sens, je réponds à la fois au au président Ruquier ou au rapporteur Delcros, et donc j'aurais un un avis négatif sur le 703 rectifié le 704 le 588 rectifié le 705 et le 895 895 3ème sujet : l'appel accession, on l'appelle n'a déjà eu longuement l'occasion de d'en débattre ici, je voudrais juste souligner un point et je sais que la ministre Lienemann il était extrêmement attaché, c'est le fait que pendant la loi de finances pendant cette loi de finances, comme je m'y étais engagé, on va étendre le PS la aux logements anciens. Et on va également permettre aux titulaires d'un bail réel solidaire de souscrire prêts à l'accession sociale madame la Ministre Lienemann, c'était un engagement que j'avais pris je ne sais pas si Madame, la ministre entend mais en tout cas, Madame la Ministre, sachez honorer mon engagement, voilà, je disais qu'il avait honoré mon engagement sur le le Pass BRS ensuite se pose la question de la domiciliation et donc, pardon, ça veut dire que j'aurais un avis négatif sur madame la présidente, l'amendement 5 422 591 et 718 ensuite, il y a la question de la domiciliation avec plusieurs amendements qui ont été posées dessus, et sur la question de de de cette domiciliation alors le le sénateur Martial Bourquin a totalement totalement raison et et d'ailleurs toutes celles et ceux qui ont déposé cette. Amendement moi je partage totalement le fait que la domiciliation, c'est un élément essentiel, ça fait partie de cet accompagnement que j'évoquais, en réponse à Madame la rapporteure Estrosi Sassone mais la domiciliation aujourd'hui tout ce qu'on fait dans les politiques d'accompagnement repose avec une Pierre fondamentale qui est la la domiciliation, dire que lorsque, par exemple dans les crédits en augmentation, comme le souligne le rapporteur d'alliés, on va cet hiver, ouvrir plus d'accueil de jour dans les accueils de jour, on fait en sorte qu'il y a le service de domiciliation quand on augmente les crédits sur le logement d'abord le logement d'abord, c'est d'abord une politique d'accompagnement par exemple sur les sorties d'hôtel et comment on fait, bah c'est d'abord la question de la domiciliation en gros quand on gère un centre d'hébergement d'urgence, il y a 2 priorités qu'on fait, collégialement, élus locaux, associations, État, c'est de faire en sorte que les enfants soient scolarisés et de faire en sorte que les parents puissent être domiciliés parce que si vous avez des enfants qui ne sont pas scolarisés, vous n'êtes pas en phase avec la promesse républicaine et si vous ne domicilié pas les personnes dans les Centres d'hébergement d'urgence, hé ben vous n'avez absolument pas la même chance de pouvoir ensuite être dans un parcours d'intégration et donc c'est un principe alors faut-il dédié au sein de l'enveloppe des crédits dédiés à la domiciliation, moi ce que je vous dis, c'est que dans toute l'enveloppe générale et et je crois que messieurs les sénateurs, Morrissey Armel Le le pourrait le dire aussi dans toute l'enveloppe générale de mon programme sur le logement d'abord et l'hébergement d'urgence, on met une priorité sur la domiciliation donc. Je j'émets un avis négatif sur le 595 rectifié de terre le 706 rectifié le 719 tout en vous disant que c'est une priorité de mon action au sein des enveloppes que et et je salue les propos du rapporteur d'alliés qui souligne que ces enveloppes sont en augmentation depuis maintenant 2 ans, il y a ensuite la question 5ème sujet de l'ANRU avec l'amendement 616 rectifié, je ne saurais dire mieux que les propos de l'argumentaire du du rapporteur en haut niveau en ouvrir plus que prévu, mais comme on n'en a pas besoin de plus que ce qu'on ouvre et ceci étant établi avec ceux qui gèrent l'ANRU au quotidien, hé ben je vous propose donc un avis, enfin j'ai

plusieurs années de ma vie à accompagner les entreprises en difficulté dans les territoires les plus ruraux et c'est vrai qu'on utilisait beaucoup la pâte mais on utilisait aussi d'autres instruments, comme Larry. Le prêt ou la subvention Harry ou comme d'autres politiques de revitalisation industrielle alors après c'est un choix qui est fait de se dire que la pâte est en réduction depuis des années, elle État 40 millions, monsieur le rapporteur Delcros, vous l'avez dit 40 millions d'euros il y a quelques années, elle est à à 6 millions d'euros aujourd'hui, c'est parce que aujourd'hui on on fixe la rénovation et l'accompagnement de ces entreprises par d'autres outils que celui de de la pâte, il ne faut pas et j'entends vos votre désaccord, il ne faut surtout pas que ce soit interprété comme soit un abandon de nos. Territoires euros soit un abandon de notre accompagnement vis-à-vis des des petites et moyennes entreprises sur ces territoires, l'avant-dernier sujet concerne amendement donc j'aurais un avis négatif sur le 707 et le 7

chaque. Le projet de loi de finances on on discute de ce sujet, il y a une différence massive, c'est que pour la première fois cette deuxième fois consécutive, on augmente les crédits des pensions de famille et pour autant on n'augmente pas le le forfait parce que je crois que je n'ai plus à démontrer mon attachement à renforcer les pensions de famille mais c'est vrai que, aujourd'hui, donc, dans le budget que je vous présente, on a 45 millions d'euros sur le logement d'abord, dont une partie dédiée aux pensions de famille pour faire 10000 pensions de famille supplémentaires sur le quinquennat qu'on qu'on qu'on a pris ce que j'ai prise, c'est de se dire cet argent supplémentaire sur les pensions de famille donc je vous rejoins totalement sur l'insisté le plus ces accompagner on aimait surtout pour ouvrir plus de pensions de famille c'est là où il y a et et j'entends le le débat, moi j'ai fait ce choix-là parce que pour en ouvrir plus de places mais mais évidemment je je comprends le sens de votre amendement sur la question des études vous dire également que c'est un élément essentiel, en fait, la dernière étude, elle date de 2012 elle était fait dans le cadre de l'INSEE, aujourd'hui on a mis en place des travaux avec notamment les associations sur cette question de l'étude et on a de nouveau de nouvelles manières si je puis dire de pouvoir mieux connaître les publics on accompagne grâce aux nuits de la solidarité, porté par beaucoup de collectivités locales et que moi je soutiens que ce soit Paris à Grenoble et dans d'autres villes, à Toulouse ou dans d'autres villes c'est nuit de la solidarité je salue l'engagement et des collectivités et des citoyens qui participent, on travaille également avec eux pour ça, pour accompagner les informations recueillies pendant ces l'une, de la solidarité, mais on a aussi d'autres remontée grâce aux centres sociaux ou autres, et donc on travaille avec les associations pour qu'aujourd'hui on puisse faire en sorte de mieux connaître ses publics sans forcément utiliser la même méthodologie qui était celle de 2012, qui donnait des résultats qui n'étaient pas forcément suffisamment utilisée par rapport aux politiques publiques que nous menons donc je partage votre constat et voilà comment on est en train d'y répondre, enfin, dernier point d'et donc j'aurais un avis négatif sur le 600 au regard de ce que j'ai dit : vous comprenez, quelle est ma position de soutien au. France : une famille enfin sur le la, le sujet de la chlordécone madame la sénatrice en fait aujourd'hui on met strictement en application ce que le président de la République a annoncé avec les montants qui l'a annoncé et qui sont en cours de déploiement et donc les crédits qui sont adoptés, la pré-pardon qui vous sont présentées là sont conformes à l'engagement du président de la République telle qu'il l'avait annoncé, j'entends le fait que vous souhaiteriez que ce soit encore plus, je souligne le point sur le fait qu'on ait un président de la République qui est reconnu la situation, la gravité de la situation, suite à la chlordécone et ce n'était pas forcément ce que tout le monde avait fait auparavant et puis deuxièmement. Qui a tenu des engagements sur les crédits auxquels il s'était engagé, et qui sont répercutés dans le budget aujourd'hui ce qui m'amène à avoir un avis demande de retrait si je puis dire, sur le 726 telle que vous l'avez présenté voilà madame la présidente, j'espère que j'ai été clair et exhaustif. Merci, Monsieur le Ministre, vous l'avez été l'exercice assez difficile, mais je crois que nous en sommes bien donc, le pire est à venir : mais non monsieur Dallier c'est positif. Bien nous passons donc au vote de l'amendement 723 avec 2 oui. Madame si bien sûr, si bien sûr. Mais encore faut-il lever la main pour prendre la parole, ou vous souhaitez.

oui madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur, et, et, évidemment, peut-être, comme l'a rappelé le rapporteur et et Monsieur le Ministre, un exercice compliqué, vu l'étendue des sujets évoqués évoqués peut-être avant de rentrer dans le détail de chaque vote dire que il y a une question qui me turlupine beaucoup, Monsieur le Ministre, sur laquelle j'ai pas la réponse et je pense que c'est clair, nombre de nos collègues l'APL. Dans son nouveau mode de calcul envisage-t-il tous les 3 mois, de mettre en place un mois de Caron, c'est dire qu'on revoit le on repart sur une base annuelle tous les trimestres, on réajuste les choses mais compte chaque trimestre on réévalue l'attribution ou non de l'APL est ce qu'on a un mois sans perception sans financement de l'APL ou pas, voilà la question que je voulais vous poser dans le cadre du temps qui m'est imparti pour les explications de vote, sinon dire qu'évidemment en tant que membre de la commission des affaires je soutiendrai les amendement des rapporteurs madame Estrosi et madame Guillemot, d'une part, surtout sur le NPNRU Monsieur le Ministre, vous dire que les crédits d'Action Logement qui sont significatifs sur la mission budgétaire et qui justifie effectivement la présence d'un budget, c'est bien, mais les crédits d'Action Logement sont pour le logement, les crédits de l'État permettent de compléter les financements sur les investissements nécessaires en matière d'équipements publics d'infrastructures qui ne sont pas prises en compte normalement par les crédits d'Action Logement qui devraient être dédiées au logement. Merci madame la présidente, effectivement, de points sur l'APL je reprends pas le mot de carence que vient de dire Valérie Létard. Mais je voudrais aussi insister parce que si c'est tous les 3 mois, je voudrais savoir comment les CAF vont faire, elles sont pas aujourd'hui en état de verser la prestation petite enfance depuis près de 8 mois pour un certain nombre de familles, donc je voudrais bien savoir comment ça va se faire au mois de janvier, parce que moi je ne comprends pas, et je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir leur APL, 6 mois, 8 mois après, parce que vu ce qui se passe pour la prestation, petite enfance, et ce qui s'est passé encore pour la prime d'activité, je pense que là, vous pouvez peut-être nous donner des précisions, surtout que cette réforme à l'a quand même été décalée d'un an, la 2ème chose, moi je veux bien qu'on donne des leçons à tout le monde, je voudrais dire quand même à Philippe Dallier, que c'est un peu contradictoire de mettre un amendement pour enlever 500 millions à Action logement et de refuser de soutenir l'amendement qui a été votée, y compris par son propre, les membres de son groupe sur l'engagement de l'État, je reprends ce que dit Valérie Létard, effectivement, c'est pas la même chose, l'État peut faire ces crédits de paiement sur d'autres choses que le logement, alors que le logement, c'est vraiment action logement mais ceci étant, s'il y a une trésorerie de combien 700 millions sur la rue, vous vous êtes content qu'il y a une telle trésorerie mais pourquoi on n'enlève pas 10 millions à Action logement ou à l'USH pour c'est l'État qui se permet de faire ça, pourquoi pas les autres. L'État, mais même le rapporteur devrait dire hé bah, écoutez, puisque c'est 10 millions de crédits de paiement, on n'en a pas besoin, c'est le ministre qui le dit lui-même, enlevons long à nos partout, puisqu'il y a aussi un amendement qu'on va soutenir où on nous dit que la ponction de 500 millions d'euros sur Action Logement, il faut l'enlever, mais pourquoi l'État ne donne plus à parité, ne respecte pas la loi pour le FNAP moi je trouve que c'est vraiment tout à fait contradictoire et il y a des leçons qui sont bonnes à recevoir pour tout le monde. Merci madame Jasmin, vous avez la parole. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, le président de la République a effectivement lors de son déplacement à la Martinique, annoncé le dit bien annoncé que l'État prendrait toutes ses responsabilités. Aujourd'hui, vous êtes discordants parce que, entre temps il y a eu cette commission d'enquête, présidée par Monsieur Letchimy et le 26 novembre dernier il y a eu un certain nombre de recommandations qui ont été faites et parmi les préconisations qui ont été faites il y a évidemment cette proposition de permettre justement de faire le diagnostic biologique, donc les haines, les analyses pour les personnes, pour la population, je crois, je ne comprends pas que vous puissiez tenir un discours discordants par rapport à ce que le président de la République avait demandé je remercie la commission qui a émis un avis favorable parce que les personnes qui sont la commission sont à l'écoute des populations, vous ne pouvez pas dire que on va s'arrêter à ce que propose le président de la République, alors qu'il a bien dit et c'est vérifiable qu'il prendrait toutes ses responsabilités, donc quand vous me dites que par le passé, les autres n'ont pas fait, on n'est pas là, on est dans le présent maintenant et il faut se mettre en perspective pour la santé des gens et c'est pas parce qu'il y a eu probablement des carences à un moment donné que vous qui dites que vous allez tout changer quand vous allez tout revoir quand vous puissiez tenir discours donc je souhaite maintenir je ne retirerai pas et je souhaite que mon amendement soit votée et que vous puissiez prendre vos responsabilités, maintenant que vous êtes au pouvoir, merci. Merci Monsieur Touraine, vous avez la parole. Oui merci madame la présidente, juste de 2 observations, l'explication de Monsieur le ministre sont remarquables d'une grande habileté indéniablement avec. Une procédure qui est un peu compliqué qui permet, qui oblige en tout cas aller très vite dans les explications à passer sur un certain nombre de choses voir affirmer de façon un peu rapide des choses qui sont, qui sont au moins sujette à caution.

D'ailleurs, si ça ne changeait pas, vous n'auriez vous feriez pas des économies d'un milliard 300 millions, c'est bien qu'il y a un certain nombre de choses qui change en bien, parfois en moins bien d'autrefois pour les étudiants, ce qui rentre dans la vie active et qui ont des besoins d'argent, ne serait-ce que pour s'installer, ne serait-ce que pour assumer leur mobilité. On calculait sur Rennes, moins de maintenant, on va actualiser, trimestre par trimestre et par conséquent, ils vont voir baisser, trimestre par trimestre, l'APL qui l'aurait affecté ou alors j'ai rien compris, alors que c'est une période de leur vie où justement on devrait les aider, par conséquent je crois utile de regarder ça de près et alors j'ai je je comprends bien que l'amendement que j'ai déposé ne sera pas voté parce qu'il y a d'autres priorités et que les contraintes qui pèsent sur l'enveloppe budgétaire font qu'il y aura d'autres, d'autres dispositions qui seront prises, mais je souhaiterais quand même que que vous le regardiez de la même façon, je ne comprends pas, mais peut-être que c'est moi qui me trompe cette fois je ne comprends pas le fait que quelqu'un qui n'avait pas d'APL soit obligé d'attendre 2 ans pour en bénéficier, c'est pas possible puisque n'importe quelle famille rentrant dans un logement qui ne bénéficiaient pas antérieurement d'une APL peut en bénéficier, simplement ces ressources seront évalués et ne seront pas calculé sur une moins de mais je ne connais pas de ménage qui soit obligé d'attendre 2 ans avant de bénéficier de l'APL ou alors c'est d'une gravité énorme auxquelles il qui il convient de remédier. Monsieur Roux, vous avez la parole. Merci madame présidente, monsieur le Ministre, c'était juste pour dire, par rapport aux demain demain 703 7 5 4 c'est ça c'est ce que nous avons déposés nous nous alignons sur la proposition de la commission finances.

alors je l'ai pris pour moi et comme lui aussi l'a pris pour moi, il me suggérait de répondre ah vous voyez comme quoi, parfois, parfois, mais parce que enfin, ceci étant dit. Sur le financement de l'ANRU il y a un accord signé par tous, on sait combien doit amener chacun : voilà l'État à 100 milliards les autres acteurs, après il y a la programmation alors effectivement la programmation, on peut en discuter, et moi je suggère qu'on appelle les fonds. la même les crédits de paiement au moment où on en a besoin, ça me paraît logique, sur les 500 millions pris à Action logement, là ça résulte de du fait du prince, alors même qu'il y a eu un engagement fort d'Action Logement en 2018 et puis il y a la clause de revoyure est tombé à l'été, ce prélèvement de 500 millions donc autant d'un côté, je peux dire donner un avis défavorable avait autre amendement considérant qu'on n'a pas besoin des crédits de paiement autant sur la ponction de 500 millions, c'est surtout la manière dont elle est amenée et et qui qui est choquante, à mon avis. merci madame la présidente, monsieur le ministre, concernant la prime à l'aménagement du territoire, je voudrais apporter un élément nouveau, puisque le le Commissariat général à l'égalité des territoires, donc, a publié un petit focus sur la pâte en en 2018 et il stipule que 68 de ces projets sont localisés dans les territoires à très fort enjeu alors c'est pas exclusivement les territoires ruraux, mais c'est aussi les quartiers de la politique de la ville, et ça c'est extrêmement important, ou encore les villes moyennes que 2 tiers de ces projets correspondent à des créations d'établissements et qu'enfin, un tiers des projets sont portés par les entreprises étrangères ce qui ce qui fait que que fin de compte, la patte à bien un triple effet la contribution certes au rééquilibrage des territoires, mais le soutien aussi au développement endogène et puis le renforcement d'attractivité des territoires pour des implantations d'origine extérieure et à ce titre, je voudrais souligner, donc les excellents résultats de de Business France et son efficacité, à la fois au service des entreprises qui souhaitent s'implanter à l'étranger faire des joint-ventures, mais aussi dans dans l'accueil des projets d'investissements étrangers en France, puisque je crois que, en 2018 on a battu un record.

oui, allez-y monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci madame la présidente, bon courage, mais n'dames et messieurs laissez sénateur je voudrais juste apporter quelques éléments de réponse très claire d'abord un madame la sénatrice l'non, il n'y a pas de mois de carence aucun moins de carence, donc ça je l'ai

madame la sénatrice Guillemot. Comment la CAF est capable de faire ben la CAF et je salue leurs agents, il s'avère que, ils sont aujourd'hui peuplée de personnes qui font un boulot formidable, alors certains des critiques, moi je les soutiens pleinement, je peux vous dire que je travaille au quotidien avec eux, ils dépensent énormément d'énergie pour être à l'heure au rendez-vous, son songez que la réforme telle que je l'indique aujourd'hui au moment où je vous parle, c'est plus de 30000 hommes jour de travail pour vous dire la l'ampleur du chantier qui explique d'ailleurs que cela n'avait pas été fait jusqu'à présent, c'est sa nécessité d'abord d'avoir l'impôt à la source et donc il fallait faire, d'abord, cette réforme de l'impôt à la source et ensuite de Metz, c'est 30000 hommes jours de travail et pourquoi on ne l'a pas fait avant parce que, évidemment, on appuie sur le bouton du lancement de cette réforme comme nous sommes sûrs qu'il n'y a aucun impact technique sur les allocataires aux appels, ce sera ma responsabilité avant de de donner le Go final de m'assurer qu'il n'y a pas d'impact sur les allocataires, c'est pour ça que je n'ai pas donné logo cet été, attendant les travaux qui sont temps court, enfin, Monsieur le Sénateur Touraine alors je vous confirme un étudiant, un étudiant n'est pas du tout impacté par la réforme, une personne statut d'étudiant, pas du tout impacté par la réforme, tout comme les apprentis, pas du tout impacté ce n'est pas le même statut, mais pas du tout impacté ce sont des, des, des personnes, des statuts, si je puis dire, qui sont aujourd'hui dans le calcul des appels fondée sur des forfaits et donc ils ne sont pas du tout impacté la question que vous posez concerne les jeunes actifs sur les jeunes gens actifs, c'est-à-dire les personnes sortant du statut d'étudiant et pendant les 2 premières années, alors là il y a différents cas de figure, il y a le cas évoqués par monsieur le rapporteur, d'allier tout à l'heure qu'il est un jeune actif qui devient en situation de travail jusqu'à présent, ils continuent à percevoir une tant qu'il déclare à la cave, qu'il était en statue de travail ou que la casse qui détend statut de travail aujourd'hui, on le sera automatiquement, c'est-à-dire que pendant les 3 premiers mois, ou un salariat, il n'y aura aucun impact parce que on calculera les 12 derniers mois, où il était étudiant pendant les 3 mois suivants ben pendant les 12 derniers mois, il aura été 3 mois, salariés et 9 mois étudiant donc il continuera à avoir un niveau significatif d'appel et ça diminuera comme cela au lieu de rester stables, comme ça l'était avant, mais, mais ces mêmes jeunes actifs, ce que personne ne dit, et je dois l'avouer, moi je l'ai découvert en ouvrant le capot et en mettant les mains dans le moteur, il s'avère, et je le redis, je le redis, quand vous êtes un jeune actif primo demandeurs d'APL, c'est à dire que vous n'aviez pas les appels quand vous étiez étudiant et que vous rentriez dans le statut de l'emploi ben figurez-vous que vous n'aviez pas les appels vous deviez attendre 2 ans,

qui devenait indépendant il y en a, et d'ailleurs il y en a de plus en plus dans notre pays, de la même manière, il avait un forfait évaluatif qui faisait qu'qui devait attendre 2 ans avant d'avoir des APL et donc c'est contre toutes ces situations que personne ne peut accepter auquel on met fin dans le cadre de cette réforme des APL en temps réel si monsieur le rapporteur accepte cette merci beaucoup. Merci, il n'y a plus de demandes de parole. Non, je ne vois pas bien, donc nous allons passer au vote des amendements. L'amendement 723 2 avec 2 avis défavorables qui est pour.

qui compte n'est pas adopté 794 rectifié même vote. Nous avons 4 amendements identiques avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement qui est pour. avons le j'ai demandé confirmation à Monsieur route, donc nous avons le 703 et le 704 ont été retirés, voilà donc c'est pour ça que nous sommes maintenant à l'amendement 5 422 591 et 718 amendements identiques : avis favorable de la commission avis défavorable du gouvernement qui est pour, qui est contre, il est, ils sont adopté 3 amendements identiques 788 705 et 895 avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour, qui est contre, ils sont adopté 3 amendements identiques 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement maintenant 795 706 et 719 qui est pour. Qui est contre. Ne sont pas adoptés amendement 616 rectifié avec 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre, il n'est pas adopté. Amendement 700 cette demande de retrait de la commission avis défavorable du Gouvernement. Monsieur, vous le maintenez. Oui, on le maintient en s'aligne sur la proposition de la Commission. rectifie rectifier vivant qui possède. Donc il est rendu identique à l'amendement numéro 7 donc je vais mettre aux voix l'amendement 617 rectifié avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour, qui est contre, il est adopté, donc nous avons maintenant quatre amendements identiques, amendement 7 rectifié 520 587 et 707 rectifié bis avec un avis favorable de la commission avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre, ils sont adoptés, amendement 726 rectifié : avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre, il est adopté. Eh bien, nous passons à 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune : l'amendement 589 rectifié, madame Guillemot, vous avez la parole. nous revenons, madame la présidente, un autre sujet, il est prévu avec les 450 millions d'euros du Fonds national d'aide à la Pierre de financer 40000 logements très sociaux et 80000 logements au total pour les étudiants le désengagement total de l'État du financement des aides à la Pierre est assumé le fond donc le FNAP et financée par la cotisation des bailleurs sociaux pour 75 millions 375 millions d'euros en 2019 le reste, soit 350 millions d'euros par action logement alors qu'en 2019 il versait 50 millions cette répartition résulte du pacte d'investissement 2020, 2022 ce désengagement complet de l'état des aides à la Pierre, rompt l'équilibre qui a prévalu à la création du FNAP en 2016, c'est-à-dire une parité de financement entre l'État et les bailleurs et une gouvernance équilibrée autour de l'État, les collectivités territoriales et les bailleurs, la question qu'il faut quand même se poser, c'est comment l'État peut-il continuer de fixer les orientations d'un. Font qu'il ne finance plus du tout. Le FNAP est un outil de solidarité nationale au sein duquel l'État doit pourtant garder toute sa place au regard des engagements pris par le président de la République dans le cadre du plan logement d'abord qui doit accélérer la production de logements sociaux et très sociaux notre amendement propose d'inscrire la contribution de l'État au FNAP à hauteur de 200 millions d'euros sans faire supporter cet effort encore sur les autres. Merci, nous passons à l'amendement 722 rectifié Madame Lienemann. Oui, c'est un amendement identique je crois très grave que l'État se désengage complètement de l'aide à la Pierre pour plusieurs raisons : d'abord parce que globalement l'action l'argent d'Action Logement, aller au logement, donc c'est de toute façon, moins d'argent pour le logement et notamment l'âge, le logement des salariés, la 2ème raison c'est que je sais bien, Monsieur le Ministre, que c'est pas votre intention, mais permettez-moi de douter, de celle de Bercy, je vois très bien ce qui se profile à l'horizon, on nous explique que l'État n'a plus les moyens d'accompagner l'aide à la Pierre et donc il faut faire rentrer dans les organismes HLM des financements privés, je n'ai pas inventé il y a une mission qui a été réalisé par le CGEDD et le ministère des Finances, or chacun sait bien qu'à partir du moment où vous avez des actionnaires privés, il y a un besoin de rendement ne fût-il modeste mais néanmoins, il faut que ce soit rentable pour ses actionnaires privés et quelle va être la conséquence, hé bien évidemment un renchérissement du loyer et par ailleurs un renchérissement des logements, la 2ème menace ce que je vois poindre à l'horizon, même si je sais que vous-même sur la question du rapport du CGEDD, vous vous êtes exprimé mais comme j'ai hélas l'expérience de la ténacité s'est aux fonctionnaires qui pense que, contre vents et marées, ils finiront par imposer leur point de vue, j'ai des inquiétudes pour l'avenir, la 2ème inquiétude, c'est le financement par le Livret A parce qu'un député, monsieur Jolivet de la République en marche, a expliqué que le système du livret actuel n'était plus tenable, ce n'est pas la première fois qu'on voit dans les rangs libéraux, la mise en cause du Livret A pour financer le logement et du livret A plus généralement quand j'entends tous ces petits bruits de fond qui finissent par se concrétiser que je vois qu'il y a plus d'aides directes de l'État, je me dis il y a péril l'oeil du cyclone est en train de se profiler sur le logement social, c'est pourquoi, de toute façon, il est fondamental, et juste de Rome et des crédits d'État du FNAP parce que la solidarité nationale est essentiel, ça peut pas être les locataires du logement social qui finance le futur logement social tout seul, ça peut pas être les seuls salariés qui finance toute la solidarité nationale, c'est bien le rôle de l'État, d'y prendre sa part. Merci. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Bon, on pourrait ré ouvrir les débats que nous avons eu, il y a 2 ans, bah oui, parce qu'en fait, c'est un peu ce que vous venez de refaire, chers collègues, on sait déjà dit beaucoup de choses sur le sujet.

on prend date, et puis on verra bon, on a eu 2 années de débats intenses autour de tous ces sujets, moi, je retiens la clause de revoyure et l'accord, on pourrait dire toujours forcé et contraint des différents partenaires, mais en tous les cas, il y a un accord pour trouver une solution qui permette de continuer à financer le logement social dans les meilleures conditions possibles, on va dire cela comme ça, étant donné la situation donc, moi, je vous suggère le retrait de cet amendement ou alors, à défaut, ça sera un avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre, quel est l'avis du gouvernement. Merci madame la présidente. Aujourd'hui, je pense que il y a au moins un point sur lequel on peut s'accorder, c'est que les engagements que j'ai pris, je les ai tenus. Je m'étais engagé à faire une clause de revoyure. On a mené 10 mois de discussions et beaucoup de travail associés. On s'est mis d'accord sur 2 éléments importants qui étaient d'un côté, cet engagement avec les bailleurs sociaux, signé en avril et de l'autre côté, se prend d'investissement volontaire avec Action Logement qui constitue un tout et dans ce tout, il y a notamment le fait qu'Action Logement participent aux Fnac en substitution des bailleurs sociaux et je crois que de la même manière ou ou depuis 2 ans, j'ai une constance sur un certain nombre de positions comme sur la question de la financiarisation, vous m'avez toujours entendu dire la même chose, je crois que vous pouvez au moins me donner crédit du fait que des engagements que j'ai pris devant vous, je me suis toujours à la fois engagé mais faire en sorte que la France se soit tenue et qu'on aille jusqu'au bout et la clause de revoyure la montrer ensuite la question qui est posée par Madame, la sénatrice Guillemot et Madame la Ministre, Lienemann c'est la question de l'engagement de l'État au titre du FNAP le point le plus important, je suis sûr qu'on sera tous les 3 d'accord là-dessus, c'est est-ce que oui ou non le FNAP finance suffisamment de logements adaptés notamment de paix Bailly l'année 2018 a été une année record en terme de logements PLI l'année 2019, c'est très difficile de savoir, et je suis très prudent dessus parce que, comme vous le savez, toutes les 2 par coeur, on connaît véritablement les sacrements en fin d'année, mais au moment où ce qu'on se parle par rapport à l'année dernière au même moment, modulo ce que je viens de dire, sur la fin de l'année, on est à un niveau encore supérieur à l'année dernière, donc moi ce qui m'importe à la fin, c'est que le FNAP idée les moyens de la production du pédalier adapté et en fait la question vous renvoyer, c'est : est ce que l'abandon du un pour un, qui qui date des gens cet abandon du un pour un et ce qu'il avait déjà commencé, merci, Madame la Ministre, est ce que il remet en cause la gouvernance que l'État peut avoir avec les gestionnaires du FNAP dans le cas de la production de logements adaptés, moi en tant que ministre, je dis que non aujourd'hui et et et je me repose notamment sur ces chiffres du du du pareil, je dis qu'on arrive très bien à gérer cette gouvernance sans le un pour un et avec des financeurs qui sont ceux que vous mentionnez tout à l'heure, le 2ème, élément que vous soulevez, c'est la question de des acteurs privés de ce fameux rapport, mais là aussi je je ne sais pas comment être plus clair pendant la loi élan il y a eu des amendements dans les 2 chambres visant à déplafonner la rémunération du capital des bailleurs sociaux, je me suis toujours opposé toujours, ensuite il y a eu la question de la vente avec ce rapport qui dit est-ce que que plutôt commander des investisseurs privés cette fois-ci, peuvent participer à l'achat dans le cadre de ce qui a été définie par la loi et non et je vais même aller plus loin, le rapport lui-même ce fameux rapport sur lequel j'ai tout de suite réagi en disant ma position de manière publique, très claire et jusqu'à preuve du contraire, le ministre du Logement, ce n'est pas un rapport, c'est la personne qui est en face de vous, jusqu'à preuve du contraire, et donc je, je, là aussi, j'ai exprimé ma position mais, mais, quand bien même vous ne me croyez toujours pas regardez ce rapport, qu'est ce qu'il dit ce rapport, le rapport lui-même met en avant les dangers d'une financiarisation, il le met en avant, et donc on pourrait même plutôt sont satisfaire en disant : enfin, on a un écrit de celles et ceux que vous craignez disant eux-mêmes que la financiarisation du modèle HLM il faut y faire très attention et prendre garde, donc je veux vraiment avoir un discours rassurant là-dessus avec la constance de mes propos depuis maintenant 2 ans et demi madame la Ministre. Qu'il soit clair, je ne mets pas en cause la parole de Julien Denormandie du ministre du Logement de ce gouvernement, je la mets pas en cause, on peut avoir des désaccords, je ne la met pas en cause mais force de constater que, quand on ne met pas les verrous. à un moment donné les engagements d'un gouvernement sont aisément remis en cause, pas forcément, même avec des gouvernements qui ne veulent pas avoir la même attention d'origine mais parce que la haute fonction publique et Bercy vous trouve 25000 argumentaire pour, finalement, de proche en proche, vous amener sur la stratégie que vous ne vouliez pas, je pourrais vous donner 25000 exemplaires et donc au nom du fait qu'il y aura pas d'argent que ceci, que cela, que c'est pas grave que quand même on va limiter la rentabilité du privé, vous allez vous risquez d'avoir ce ce dérapage, donc il faut maître des clichés et pour maître de cliquet : la nécessité de l'aide à la Pierre, financé par l'État, me paraît un déclic est important : la 2ème, chose que je voudrais dire à notre rapporteur, je comprends sa logique, je veux quand même dire que la politique de la France, de logements, en tout cas le budget voté par le Parlement et il n'est pas voté par un accord, Dieu sait que je suis attaché au mouvement HLM entre le mouvement HLM, le gouvernement et le 1 parce que chacun sait bien que les compromis ben ça suppose des rapports de force, on le vrai rapport de force démocratique, il est au Parlement, je n'ai pas contesté cet accord, je pense que vous avez inscrit dans le budget, l'accord, je dis que cet accord, on doit l'améliorer et d'ailleurs chers collègues d'Dallier, vous l'avez amélioré en puisqu'on a vu, on nous avez voto ensembles, la restauration de la TVA sur le plus, je pense qu'on peut faire un effort supplémentaire pour l'améliorer en restaurant un niveau d'aide à la Pierre, financé par le budget de l'État. Si Madame la présidente, oui je vais réagira aux propos de monsieur le ministre, un petit peu comme Marie-Noëlle Lienemann sur plusieurs plusieurs points sur les engagements de l'État, moi je veux bien qu'on dise, l'État. Ne respecte pas ses engagements, ni sur le FNAP la loi, c'est pourtant la parité, ni sur l'ANRU etc mais on continue de faire les poches des autres, et comme le dit Marie-Noëlle Lienemann c'est nous qui votons le budget et donc même si la clause de revoyure a été c'est vrai et vous l'avez dit. Il y a un moment où on peut quand même se poser la question, c'est comme pour l'APL, ce que dit Marie-Noëlle Lienemann c'est vrai. Vous êtes ministre du Logement. Mais Bercy fait ce qu'il veut, quand il. Et tout Ministre du logement que vous êtes malheureusement vous n'arrivez pas à maître cliquet effectivement et c'est comme ça qu'on traîne le boulet, comme le dit le président de la République de l'APL et puis je parlerai de de beaucoup de choses sur ce que vous nous dites sur le rapport, mais le rapport, il a été fait par l'IGF à la demande du. Donc après que vous nous disiez que vous partagez pas, moi, je peux l'entente lui j'ai la même position que Marie-Noëlle Lienemann mais ça n'empêche pas qu'il a été demandé à la demande du gouvernement

Si vous demandez ce rapport c'est qu'on se pose la question, on s'est posé la question sur la réforme, la tout ça et vous continuez, vous continuez, vous continuez, troisièmement, moi je n'ai pas vécu comme vous, la réunion, la convention nationale d'Action Logement. Pourquoi les représentants de l'État ne viennent plus au conseil d'administration, Monsieur le Ministre, pourquoi les représentants de l'État ne viennent plus au conseil au conseil d'administration d'Action Logement. Moi j'ai pas vécu la convention nationale comme vous quand Action logement, on parle d'un certain nombre de choses. Qui ne peuvent pas par exemple faire leur plan de 9 milliards parce qu'il y a eu un véto. Non mais attendez, c'est pourtant ce qui nous a été dit, donc vous, vous avez cette perception, nous on a une autre perception et on sait qu'il y a eu véto des représentants du gouvernement et qui ne viennent pas siéger le dernier CA donc expliquer peut-être que vous avez des explications là- dessus mais enfin quand même quand département parle du mépris du gouvernement je pense quand même qu'il faut s'interroger. Si monsieur Dallier, vous avez demandé la parole. Merci madame la Ministre, Monsieur le Ministre, oui pour revenir sur la clause de revoyure et la souveraineté du Parlement. La preuve que je ne me sens pas absolument liée par la clause de revoyure section en première partie, la TVA à 5 5, nous l'avons voté tous ensemble ici, à l'unanimité, mais moi ce que j'ai envie de vous dire, imaginons dans nos rêves plus fous que au moment de la CMP, on puisse discuter avec nos collègues de l'Assemblée nationale. Bon, il faut peut-être choisir un peu nos combats, je préférais effectivement qu'on soit sur la TVA à 5 5 plutôt que sur le retour des aides à la Pierre, alors certes, philosophiquement, on peut en discuter mais moi je préfère la TVA à 5 5, donc il faut peut-être pas tout demander si jamais on veut discuter un peu sérieusement et en leur suggérant même si la CMP n'était pas conclusive de conserver certaines mesures de la même manière sur le PTZ dans les zones détendues, voilà c'est tout ce que je dis. Merci madame la présidente, je voudrais répondre à Madame la sénatrice, la première chose sur le rapport, moi j'adore, je veux bien entendu toutes ces critiques en disant : ce rapport, c'est pas bien, etc, vous nous dites vous-même que vous n'avez pas lu. d'accord, mais donc je vous dis moi que ce rapport, en plus, il permet, il permet aux même que vous critiquez au même que vous critiquez qui écrivent qu'il faut faire attention à la financiarisation et vous dites l'inverse et après, vous nous dites que vous n'avez pas lu, donc, croyez-moi, si si, moi je vous dis que je me si moi je vous dis que le ministre que je suis s'oppose à tout ça et qu'en plus on a un rapport qui va dans mon sens, ben, au contraire, ça fera date, ça fera date 2ème élément sur actions sur Action logement je veux vraiment qu'il y ait aucun malentendu Action logement, on est des partenaires, je peux vous dire que si il y avait une difficulté de communication avec la qui font de logement, on n'aurait pas conclu ce plan d'investissement volontaire de 9 milliards on aurait pas depuis lors lancé la structure qui permet de transformer les bureaux au logement mais ce n'est pas, mais ce n'est pas à l'arrêt, madame la sénatrice, mais ça n'est pas à l'arrêt, aujourd'hui la la la la la la courroie de transmission permettant de faire les 3 mesures ménage le transformation je vous en ai déjà parlé 1000 fois 200000 baignoires en 200000 douche, vous savez, cette mesure auquel je tiens tant le 0 970 830131 c'est en cours de déploiement, la transformation de la rénovation énergétique des bâtiments, c'est en cours de déploiement, la prime de mobilité, c'est 300 par jour qui sont, la Madame, la sénatrice de la même manière, l'État, il est faux, il est faux, il est faux de dire que l'État ne siège pas Action logement c'est pas vrai, c'est pas vrai que les décrets ne sont pas pris, ils sont pris, hier encore, on a signé avec Action Logement Le plan logement outre-mer un milliard 5 qui est en cours de développement, il y a quelques jours, on en sait, le le le véhicule nationales sur l'acquisition des logements sociaux, donc Action logement, on est dans une relation de partenaires après un partenariat, c'est comme un ménage, c'est comme un couple parfois vous dites les choses et parfois vous dites les choses un peu brutalement, bah ça fait avancer la la la vie, il n'est pas un un fleuve tranquille et c'est pas parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille que le partenariat n'est pas. Seul le ministre Bien, je vais mettre aux voix l'amendement 589 rectifié avec 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Ce n'est pas adopté l'amendement 722 rectifié avec 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. N'est pas adopté, nous passons à l'amendement 590 Madame Artigalas. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, toujours sur les aides au logement, le gouvernement poursuit la sous-indexation des APL, en fixant leur révolution Il vous plaît, on on écoute l'oratrice et après le gel de 2018 et la baisse de 5 euros en 2017, il s'agit là d'une nouvelle atteinte au pouvoir d'achat des ménages les plus modestes car cette évolution ne correspond ni à l'inflation, environ, ni à la hausse de l'indice de référence des loyers 1,5 pourcent lors d'un échange avec des étudiants de l'énergie, de l'université d'Amiens, le président de la République, je le redis à regretter la baisse des 5 euros des APL en cohérence, il apparaît nécessaire d'arrêter de faire chaque année des économies sur les ces aides au logement notre amendement propose donc d'indexer les aides au logement a minima sur le taux d'inflation et de majorer en conséquence, les crédits du programme 109 sans faire supporter cet effort aux autres programmes de la mission, je vous remercie, merci monsieur le rapporteur. la revalorisation de 0,3 pourcent avait été voté pour 2019, et pour 2020, mais que le Conseil constitutionnel avait censuré, considérant que, au titre de l'annuité budgétaire l'annualité budgétaire, on devait y revenir, donc nous y revenons. La l'amendement, vous le chiffrez à 83 millions d'euros, je voudrais d'abord vous dire que je pense que c'est un peu plus que ça, puisque l'enveloppe, c'est 15 milliards donc 0 7 pourcent sur 15 milliards, ça me semble difficilement faire 83 millions d'euros, plutôt un peu plus d'une centaine. Alors après, sur le fond. La commission des finances ami a émis un avis défavorable, maintenant moi je suggérerais au gouvernement d'y réfléchir à nouveau parce que c'est vrai que ça a été rappelé, et le président de la République l'a reconnu, depuis 2017 et l'Automne 2017, ça fait beaucoup. Et je rappelle quand même que l'APL et la presse, enfin la prestation l'allocation la plus redistributive de nos aides sociales, donc il y a un vrai sujet voilà alors l'avis de la commission des finances est défavorable, je le redis, mais pour autant il y a un sujet. Merci madame la présidente, sur ce volet de la revalorisation mais c'est un sujet dont on a déjà parlé notamment de l'année dernière, donc j'aurais la même position, on a fait des choix, des choix de de revalorisation d'un certain nombre de prestations à hauteur de l'inflation, d'autres à une hauteur inférieure, vous me direz, gouverner, c'est faire des choix, ce sont les choix que nous avons fait et j'entends le monsieur le le rapporteur d'alliés qui ne partagent pas forcément de ces mêmes choix c'est c'est le principe même de la démocratie. Vous émettez un avis défavorable, donc mettre aux voix l'amendement 590 avec 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre, n'est pas adopté, nous avons 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune : l'amendement 720 rectifié Madame Lienemann. Pour être franche, c'est plutôt un amendement d'appel puisqu'il s'agit de renforcer les crédits de l'Anah et il est certain que la somme que nous avons mis ne réglera pas l'ensemble des problèmes de l'Lana et que par ailleurs avec le jeu des inscriptions des recettes et des dépenses prendre sur les autres secteurs du logement était évidemment un problème néanmoins je pense que, chers collègues, il faut donner ce signe politique l'Lana est un outil incomparable pour la rénovation de l'ancien, ça va des centre-ville ça va de l'habitat insalubre, ça va en particulier sur la question de la transition énergétique avez vous rappeler on a débat au moment de la loi de programmation énergétique sur les fameuses passoires thermiques, on a eu le débat sur la manière de justement veiller à ce qu'enfin on fasse ses travaux de d'économie d'énergie dans le bâtiment, on avait souhaité qu'il y ait des sanctions pour l'échéance de 2028. Et le gouvernement nous a dit non, on ne va pas maître de sanctions, mais on va d'abord mettent massivement des aides. Eh ben massivement des aides, les aides, elles ne sont pas là, c'est la raison pour lequel nous souhaitons un accroissement des crédits de l'Anah et particulièrement sur l'insalubrité et sur les économies d'énergie. Merci, monsieur, nous passons à l'amendement 592 rectifié monsieur Gillet. Merci madame la présidente, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, alors effectivement en prolongement par rapport à l'Anaes, donc l'année un objectif 60000 logements donc à rénover an son budget, donc financée par une contribution budgétaire piloté par le ministère de la transition écologique pour prendre en charge la transformation du CICE en prime destinée à financer les travaux de rénovation et bénéficie également d'une part de la taxe sur les logements vacants pour 40 millions d'euros et d'une part des recettes issues des ventes aux enchères de quotas carbone pour 110 euros 110 millions d'euros, ces montants sont plafonnées dans le cas de la première partie du PLF et donc, compte tenu des règles de recevabilité appliquée au Sénat, il n'a pas été possible pour les parlementaires d'intervenir sur ce levier, compte tenu des missions essentielles d'accompagnement des ménages les plus fragiles dans la transition écologique il paraît légitime de donner à la n'a les moyens de réaliser correctement toutes ses missions, à ce titre-là, nous avons tous été dans nos permanences, interpellé par des personnes souvent en difficulté pour lesquelles nous avons été obligés de mettre en place des médiations pour instruire des dossiers parce que les dossiers sont souvent instruit à distance et ne permettent pas des personnes particulièrement en difficulté de pouvoir déposer les dossiers dans de bonnes conditions

mais compte tenu de ses ressources contrainte n'a dû récemment par exemple revoir à la baisse le plafond des aides aux travaux de programme Habiter mieux agilité au regard des engagements que l'État s'est assigné en matière de transition écologique notre amendement propose donc de renforcer de 30 millions d'euros pour 2020 les moyens dévolus à l'sans faire supporter cet effort aux autres programmes de la mission, il s'agit donc principalement d'améliorer la qualité de l'accompagnement et de l'instruction des dossiers auprès des plus précarisée se sont, sinon ce sont toujours les plus opportunistes qui en profite. Merci, quelle est la ville de la commission, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors oui ou non l'Anaes aura-t-elle besoin de moyens supplémentaires en 2020 effectivement, voilà la question qui est posée, moi je suis plus inquiet pour l'année suivante que pour l'année 2020, mais difficile effectivement d'y voir clair

et vous savez comment les choses se passent, ce sont ceux qui vendent ou installer chaudière qui font la publicité en disant votre chaudière pour un Euro, c'est vrai que ça semble sympathique, sauf que quand on y regarde dans alors évidemment on a multiplié le nombre de dossiers, sauf que quand on me regarde dans le détail, c'est ce que nous ont dit ce que nous avons auditionnés le prix des chaudières à augmenté de 20 à 30 C'est quand même un vrai problème, alors on peut effectivement être content qu'un certain nombre de propriétaires puissent remplacer leur chaudière avec effectivement une meilleure efficacité énergétique, mais quand même, toutes les aides que nous pouvons attribuer, il y a une partie qui part en fumée au travers du tuyau de la chaudière en question, c'est quand même, c'est quand même un vrai problème, alors ceci étant dit, alors je sais pas comment on peut effectivement parce qu'après on peut discuter avec les, les, les syndicats professionnels, etc, j'imagine que vous le faites, monsieur le mini-je ne sais pas très bien quelle efficacité ça peut avoir parce qu'après, sur le terrain, une fumée blanche à la sortie, la négociation, mais pour autant les résultats ne semble pas être tout à fait là voilà donc moi je propose au nom de la commission, le retrait de ces 2 amendements, je pense que le vrai sujet, ce sera effectivement 2021 plutôt que 2001. Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente, je crois que beaucoup a été dit par monsieur le rapporteur, le 1er point qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement aujourd'hui l'est victime de son succès et alors, objectivement, je préfère me présenter devant vous en vous disant : on a un problème de financement parce qu'on est victime de notre succès, plutôt que de me présenter devant vous en vous disant modifions les Budgets parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on avait dit qu'on ferait songer le plan, je veux dire, comme l'a dit monsieur le rapporteur effectivement a incroyablement bien marché continue à très très bien marché, mais de la même manière que moi j'ai été nommée en charge de donc, du logement et donc la tutelle de l'Anah j'avais fixé pour l'année 2018 Alan, un objectif de transformation de 75000 logements c'était 25 pourcent d'augmentation par rapport à ce qu'il faisait avant, Obtenu entre 60 et 65000 rénovations, donc on l'année dernière on était, on était pas au 75000 logements de rénover que j'appelais de mes voeux en termes d'objectifs fixés cette année on va terminer l'année entre 100 à 120000. Pour vous dire le déploiement à quel point il a augmenté en l'espace de simplement 2 ans grâce notamment au boulot fabuleux des équipes de l'Anah, que ce soit sur la rénovation énergétique des bâtiments, avec en plus, ma prime 9 que nous lançons dans quelques jours, que ce soit dans la lutte contre l'insalubrité des bâtiments, le plan co-prod dégradé, que ce soit dans l'adaptation des des logements, notamment pour les personnes en mobilité réduite et aujourd'hui tous les programmes de l'Anah, madame la sénatrice Valérie Létard le le connaît mieux que quiconque, sont en cours de déploiement d'une manière très très forte et très accéléré et c'est très bien ainsi, mais c'est vrai que ça nous pose ensuite des difficultés qui sont des difficultés de financement qu'il va nous falloir traiter et je je plussoie aux propos de de monsieur le rapporteur, l'année clé, c'est l'année 2021 et non pas l'année 2020 donc 2020 on sait gérer, même si c'est pas forcément évident mais on va voir un vrai sujet sur l'année 2021, on est en train d'y d'y travailler pour être sûr que on n'ait pas de, de, s'agissant du dernier point sur les prix qui augmentent ou les fraudes, on annonce avec ma collègue Agnès Pannier Runacher un grand plan dessus à la fois d'améliorer des contrôles à la fois de la dette des entreprises mais aussi de lutte contre vous savez ces appels un temps pestiféré ce harcèlement téléphonique par certaines personnes qui par exemple se font passer pour l'État, alors que l'État ne démarche jamais par téléphone jamais et qui font qu'un certain nombre de personnes, notamment de nos aïeux doivent parfois se des prêt déplacer 5, 6, 7, 8 fois par jour pour aller répondre à un démarchage téléphonique ben là on a lancé ce ce grand plan de de lutte contre ça qu'on est en train de de déployer donc avis défavorable. Merci. Donc maître oui pardon Madame Létard, vous avez demandé la parole. Oui merci madame la présidente, monsieur le ministre évidemment. Comme tout le monde, j'ai entendu les arguments et les éléments et je partage le fait que l'Anaes a eu des moments où il s'est. L'organisme a eu du mal à mener toutes ces politiques a bien mais pourquoi elle avait du mal à les mener à bien, hé bien, pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui elle est victime de son succès, à savoir où on met les curseurs. à quel niveau on positionne des critères d'éligibilité quel public peuvent bénéficier à quel niveau des aides, il y a eu des années effectivement pas très lointaine, où on avait limité par exemple aux ménages très modestes, l'éligibilité au plan Habiter mieux et c'est vrai que quand vous me mettez en place des politiques de rénovation thermique des logements ou d'autres politiques publiques ou limiter fortement et les contributions financières et les publics éligibles forcément hé ben vous n'atteignait pas tout de suite les objectifs cette année, on l'a vu, on a le gouvernement a fait un effort pour aller beaucoup plus loin, effectivement dans l'accompagnement des ménages et d'un certain nombre de politiques, peut-être trop sur le plan, je veux dire, il faut l'recalibrer mais attention yo-yo Monsieur le Ministre, je comprends bien, 2020, ça va passer parce qu'on va resserrer les critères, mais attention de ne pas rendre les choses incompréhensibles aux populations mais aussi aux collectivités qui vont plus savoir sur quel pied danser parce que la solution de l'avenir de ça donc vraiment, monsieur le ministre et monsieur le rapporteur oui 2020 peut-être, on peut en sortir, on peut en sortir en resserrant les boulons mais reconnaissez que 840 millions de recettes de quotas carbone 420 affecté à l'c'est absolument pas satisfaisant, surtout quand le CICE est en train de s'éteindre petit à petit, c'est pas possible qu'on mette le paquet sur les plus modestes, mais qu'on le mette vraiment et que l'argent qui est estimé aux enjeux climatiques à la réduction des émissions de CO2 et aux ménages qui sont les plus en difficulté, vraiment, là, c'est vraiment le message à passer aujourd'hui au gouvernement. Merci. Bien, je vais mettre aux voix, donc l'amendement 720 rectifié avec une demande de retrait, un avis de la part de la Commission et un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre, il n'est pas adopté même vote pour le 792 rectifié. Même vote. L'amendement 695 rectifié, monsieur merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, pour constituer un progrès, la dématérialisation des démarches administratives, doit être Monsieur le Ministre, inclusive afin d'assurer l'accès de tous aux services publics, l'État doit remporter l'adhésion de l'ensemble de nos concitoyens qui, pour 13 millions d'entre eux rencontrent des difficultés avec les nouvelles technologies ce qu'il exerce, exclus de fait de ces avances, l'absence d'accompagnement de la dématérialisation pourrait être contre- productive et renforcer davantage la fracture numérique, un effort conséquent doit être consacré à l'inclusion numérique alors que les crédits précédemment inscrit au programme 134 de la mission, Économie et qui permettait de financer cette politique ambitieuse ont été réduits à néant, dans le cadre à la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires par cet amendement, Monsieur le Ministre, nous vous proposons de rétablir ces crédits destinés au financement de l'inclusion numérique et d'accompagner la montée en charge du plan national pour un numérique inclusif dès 2020, ils ont proposé d'abonder à hauteur de 22,3 millions d'euros en autorisations d'engagement il y a un crédit de paiement, le programme 212 afin de financer 5 politique : la première, le budget d'intervention du programme inclusion numérique de la haine, c'était à hauteur de 4 8 millions d'euros, deuxièmement, le lancement des compteurs numériques, la belle qualité des lieux d'accompagnement numérique de proximité à hauteur de 500000 euros, troisièmement, la formation des aidants numériques et des ressources pédagogiques à hauteur d'un 1000000 d'euros, quatrièmement, le plan de montée en charge des dames comme service public numérique qui permet de sécuriser l'accompagnement des usagers par le service de proximité, à hauteur d'un 1000000 d'euros également, en fait, le lancement d'une seconde vague pardon vague de déploiement du Pass numérique et ce à hauteur de 15 millions d'euros, mes chers collègues, comme vous pouvez le constater ce sont autant d'initiatives qui sont bienvenus dans nos territoires, indispensable pour ne pas exclure une partie importante de nos concitoyens, les règles de ce recevabilité financière nous imposant de prélever des crédits au sein du programme

Madame la présidente, monsieur, monsieur le ministre, chers collègues, le le sujet qui est posé par Yvan Colonna et ses collègues est extrêmement important, c'est celui de l'inclusion numérique parce qu'on sait que l'arrivée du numérique a été à la fois une formidable ouverture, il a ouvert de nouvelles opportunités nouvelles perspectives, et en même temps, s'est accompagnée de nouvelles fractures territoriales d'ailleurs, vous l'avez rappelé monsieur le Ministre, mais aussi d'une nouvelle fracture sociale parce que tout le monde n'a pas la même agilité avec l'usage du numérique et du coup, ça crée des exclusions et donc la question qui est posée est très importante et et du coup, notre collègue dit les crédits qui était avant fléchée sur le programme 100 34 ans disparue, donc moi je me retourne vers vous monsieur le Ministre, pouvez-vous nous éclairer sur les crédits qui sont consacrés aujourd'hui à l'inclusion numérique ou retrouveront on retrouve tant les crédits qui était avant fléchée sur le programme 100 34 ans, s'il y a des réponses concrètes sur sujet si on est assuré que ces crédits sont bien présents dans le PLF qui nous est présenté, on demandera le retrait de cet amendement. Monsieur le Ministre, quel est l'avis du gouvernement. gros au sein du gouvernement, moi j'ai la charge, du déploiement des infrastructures, ce que j'indiquais tout à l'heure avec aujourd'hui un rythme qui s'est profondément accéléré et aujourd'hui notre principal défi c'est l'usage, et d'ailleurs j'en veux pour preuve, c'est que la perception qui compte à la fin que aujourd'hui on nous parle beaucoup plus d'usage que d'infrastructure, cela ne peut pas du tout dire que les infrastructures sont terminées, mais enfin, ça veut dire que ça veut dire que l'accélération sur l'un des infrastructures qu'elle commence à se faire ressentir alors sur l'usage maintenant je, je prends votre point que vous avez profondément raison je sais que que le secrétaire d'État, Cédric O travaille avec beaucoup de, de, de talent, mais surtout de détermination pour trouver les voies ses moyens de financer les différents outils, il y a notamment la question du Pass numérique qui fait l'objet de toutes ces contractualisation en particulier avec souvent l'échelon départemental, il y a la question d'un certain nombre d'accompagnement que nous traitons, y compris au type d'ailleurs du FSM et puis il y avait la question de ces Budgets dédiés sur certaines opérations qui évolue au fur et à mesure, moi j'ai un problème fondamental, c'est que ça ne peut pas être les opérations de la politique de la ville qui finance ces opérations là. Donc je vous proposerais volontiers un retrait pour que ces discussions puissent notamment les avoir avec le secrétaire d'État, je vous donne juste un exemple, par exemple dans le crédit politique de la ville, cette année, on les a renforcés, y compris pour faire ses fabrique du numérique dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est-à-dire des endroits qui sont des fabriques où on vous donne des cours sur le numérique, on vous accompagne pour déterminer vos projets numériques et donc ça, ce sont des crédits qui sont dédiés mais je je ne peut avoir qu'un avis défavorable, surtout si cela conduit à limiter l'action qu'on fait et qu'on porte dans les quartiers prioritaires de la ville qui parfois sont liées au numérique, donc je vous proposerai une position de retrait. Monsieur le rapporteur, vous devez vous avez demandé l'avis du gouvernement, vous le suivez. Oui, j'ai demain surtout des, des, des informations, enfin : un éclairage au gouvernement et donc je je m'associe au retrait de cet amendement. Monsieur Collin le retirer très bien, passons à l'amendement 596 rectifié, madame Guillemot. Madame la présidente, je serai très bref, il s'agit d'un rappel c'est la loi élan qui a fait passer de 100 pourcent à 20 pourcent la part des logements devant être construit dans le respect des normes handicapés au sein des immeubles d'habitat collectif en prévoyant que les autres logements seront évolutifs, à l'issue de travaux simples gouvernement fait peser sur les personnes en situation de handicap, la contrainte de faire des travaux d'adaptabilité, nous avions déjà attiré l'attention que cette mesure compliquer fortement l'accès des personnes handicapées, au logement et, généralement, un dossier, c'est plus de 6 à 8 mois l'est chargé de les accompagner, elle doit ainsi verser des subventions pour travaux bailleurs on sera content, on sera heureux d'avoir un bilan pour co-financer donc les travaux au bénéfice des personnes en situation de handicap et c'est pourquoi nous proposons de renforcer 10 millions d'euros les moyens dévolus à l'pour remplir cette mission. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'était un moment que la commission n'a pas pu examiner puisqu'il a été repêché au type de la recevabilité alors il concerne effectivement les moyens de l'mais spécifiquement orientée sur la mise aux normes pour les personnes handicapées, donc je vous propose de nous en remettre à l'avis du gouvernement. Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente j'aurais un avis, une demande de retrait sinon défavorable en fait c'est exactement la même question qu'on évoquait tout à l'heure, la question de l'accompagnement de l'adaptabilité ou l'adaptation du terme, l'adaptation des logements aux personnes à mobilité réduite, vous avez 1000 fois raison, Madame la sénatrice cet essentiel jusqu'à présent de la Nahe faisait entre 10 et 15000 projets d'adaptation par an, cette année, j'attends les résultats consolidés, on va dépasser les 20000 on sera autour des 20000 donc on a là aussi profondément accéléré qu'on fait et ce que je disais tout à l'heure donc, pour moi, il ne le la question, c'est pas de faire une enveloppe dédiée au sein de l'ANA c'est la question du budget de l'ANA de manière générale on augmente dans la lutte contre l'habitat insalubre dans l'accompagnement rénovation énergétique dans l'adaptation des logements, on simplifie d'ailleurs par la loi, l'adaptation des logements, j'en veux pour preuve l'ordonnance que j'ai présenté en conseil des ministres sur les copropriétés qui favorise la aussi, la mise au fin des travaux, la mise en oeuvre et des travaux pour rendre accessibles les logements, y compris dans les parties communes, qui était attendue depuis longtemps par les associations de personnes en situation de handicap, donc je vous proposerais volontiers une position de de retrait sinon défavorable en renvoyant cela dans les discussions budgétaires de la 2021 qui est vraiment le le sujet qui va nous occuper cette année. Eh bien, madame Guillemot. Oui, nous allons pas le retirer, nous nous maintiendrons cet amendement en disant : vraiment, monsieur le ministre, contre le temps du dépôt et le temps où l'argent arrive demander aux familles, moi j'ai dit familles que j'accompagne et je peux vous dire que c'est pas très drôle. Merci donc je mets aux voix l'amendement cette 596 rectifié avec 2 demandes de retrait habite donc défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour.

Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, après le drame d'Aubagne, celui de Saint-Denis 7 Montreuil, il y a 2 jours qu'un immeuble où s'est effondré, témoignant de la difficulté des pouvoirs publics à appréhender ses enjeux et ses urgences. Monsieur le ministre, je sais que vous êtes sensible sur cette question, mais nous voulons maintenant des actes tangibles. Que constate-t-on dans ce budget. Dans les crédits de la mission cohésion des territoires et dans le programme Urbanisme territoires et amélioration de l'habitat pour l'action de 3, ces crédits sont en baisse, ce n'est pas au niveau de la crise et des défis que nous avons devant nous, c'est donc 32 pourcent en moins en autorisations d'engagement et 20 pourcent en moins en crédits de paiement alors même, alors que les mêmes. Les événements et les drames nous oblige à intensifier la lutte contre l'habitat indigne, en mobilisant mieux encore, notamment les préfets on constate notamment et selon les bleus budgétaires que plus un seul Euro n'est prévu pour l'hébergement ou le relogement des occupants en cas de défaillance des propriétaires, comment l'expliquez-vous est-ce à dire que vous vous reposez encore une fois, uniquement sur les collectivités territoriales, comment expliquer encore que l'aide aux travaux pour les propriétaires modestes et des milliers de moitié, passant de 17 à 10 millions que vous nous vendez la transformation du site et eux comme un progrès recentrés sur les personnes les plus fragiles, nous voulons mais attendons des réponses car si la lutte contre l'habitat indigne mérite de renforcer l'arsenal juridique, le Sénat a déjà travaillé sur cette question, cela ne suffira pas, la police de l'habitat a besoin des moyens financiers et humains pour se réaliser, l'État, l'État doit prendre financièrement de ses responsabilités au travers des préfets dans la lutte contre leur l'habitat insalubre, notamment dans la lutte contre le saturnisme, comment accepter aujourd'hui que l'habitat tu que des millions de personnes souffrent du mal-logement que 2 8 millions de personnes vivent encore dans des conditions de logement très difficiles, c'est-à-dire en manque de confort flagrant ce qui peut englober l'habitat dégradé indignes et insalubres par cet amendement, nous demandons un minimum le maintien des crédits à un niveau équivalent à 2019, et nous espérons que le gouvernement lèvera le gage je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors cet amendement n'a pas été examiné par la commission des finances, donc je vais donner un avis à titre personnel, vous avez raison de pointer une diminution des crédits entre 2000 19 et 2020, mais il faut remonter à l'année précédente, les crédits en 2018 n'étaient que de 7,2 millions donc ils sont passés à 15 millions l'année dernière à 20,5 millions et dernière ils redescendent à 5 1 mais cela s'explique et je m'en remettrai donc à l'avis du gouvernement à une expérimentation par une expérimentation d'une aide aux travaux les propriétaires modestes en vue de la résorption de l'habitat insalubre en Outre-mer, instauré en 2019, donc il y avait une expérimentation, ce qui expliquait l'augmentation des crédits, donc les crédits redescendent cette année, bon je souhaite entendent l'avis du gouvernement sur le sujet. Eh bien, nous allons passer à l'avis du gouvernement avec Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, madame la présidente, monsieur le le sénateur gay d'abord je voudrais vous remercier parce que vous avez mentionné le toute implication qui est la mienne dans la lutte contre s'habitat cet habitat indigne, il s'avère que la rue d'Aubagne, j'y étais au moment où le 3ème immeuble s'est effondré et donc on a énormément travaillé, on a fait d'abord des modifications législatives contre les marchands de sommeil dans la loi élan et ensuite ici dans le cas de la PPL du sénateur Gilles on a ensuite lancé cette ce plan de lutte contre les copropriétés dégradées ce plan co-prod dégradé que j'ai annoncé justement à Marseille, quelques semaines avant le drame votre question, elle porte sur un point très précis que sont les crédits alloués à la lutte contre l'habitat insalubre, ce qui est clair c'est que lutter contre l'habitat insalubre, ça nécessite des moyens financiers, alors dans ce budget-là et je et je vous remercie de de votre amendement ça permet vraiment d'exposer pourquoi aujourd'hui à cette ligne qui qui qui baisse, pourquoi il y a cette ligne qui baisse parce que, comme l'a très justement rappelé monsieur le rapporteur, cette ligne qui. Est un niveau très faible avant on a augmenté de 17 millions d'euros, pourquoi, pour faire face aux conséquences de la suppression de l'APL accession dans les Outre-mer parce que la paix, l'accession dans les Outre-mer était l'outil utilisé et et mesdames les sénatrices, je me souviens qu'on avait eu ce débat l'année dernière était l'outil utilisé pour lutter contre l'habitat insalubre et l'habitat indigne, il s'avère que, dans ce budget, on réintroduit l'appel accession Outre-Mer, on le réintroduit donc de facto l'expérimentation en question et les moyens et donc on fait des transferts parce que précisément on réintroduit l'APL accession donc si cette ligne est en baisse, ça n'est en rien un symbole d'une d'une moindre implication du gouvernement, bien au contraire, l'appel accession Outre-mer, on l'a réintroduit précisément pour aller lutter contre l'habitat insalubre ensuite ou est-ce qu'on finance la lutte contre l'habitat indigne, principalement à travers l'. Qui l'organisme d'action du ministère que je pilote dont j'ai la la tutelle pleine et entière, si je puis dire l'aujourd'hui c'est près de 300 millions d'euros qu'on met dans la lutte contre l'habitat indigne, ce plan copropriétés dégradées que j'évoquais, 3 milliards d'euros sur 10 ans le plan coprs dégradée avec des éléments essentiels comme le prêt finance. Des travaux d'office, c'est-à-dire des travaux d'urgence lorsqu'un immeuble est en train de s'effondrer, y est quelque chose de totalement nouveau que j'ai proposée par exemple par la collectivité marseillaise pour aller plus vite dans la réparation des des immeubles concernés enfin 3ème élément et j'en terminerai là il y avait quelque chose d'aberrant dans la lutte contre l'habitat insalubre, c'était le le les astreintes qui était fait les astreintes, dans le cas de la loi élan on a considérablement élargi la possibilité donnée aux élus locaux, de mettre des astreintes vis-à-vis de ces criminels, que sont les marchands de sommeil avant c'était la galère, si vous ne perd pas l'expression pour pouvoir mettre ses astreintes aujourd'hui c'est beaucoup plus facile, mais le truc qui ne pouvait pas marcher, c'est que les astreintes, une fois que la collectivité locale l'avait prononcé parce que c'était, c'était souvent elle qui allait qui ouvrait la porte du marchand de sommeil, le montant des astreintes, il dans mon budget. J'ai changé la chose, c'est une enquête de la loi élan et depuis le 1er janvier maintenant les astreintes ne sont plus reversé au budget de l'État, mais ils sont reversés au budget de la collectivité locale, et c'est bien mieux, bien mieux ainsi parce que ça incite à, collectivités locales, il s'accompagne la collectivité locale qui fait l'effort d'aller porter justement ces astreintes et par là même, avec le financement récupérer étayer ses services etc, voilà tout ce qu'on fait, monsieur le sénateur, donc j'avais une position de de retrait sinon défavorable. Madame Lienemann. Oui, Monsieur le Ministre, loin de nous, de dire que rien n'a été fait pour essayer de combattre l'habitat indigne, le problème c'est que plus le temps passe, plus l'habitat indigne, se développe, ne serait-ce que pour une raison purement technique, c'est-à-dire que toute une série de nos bâti son ancien, et s'il y a pas des investissements, le nom de, de logements qui se détériore est important donc, vous l'avez dit nous on avait soutenu dans la loi élan c'est bien dit rare sujet ou sur la loi et là, on était d'accord, la la stratégie qui avait été améliorée sur l'habitat indigne, on a aussi apprécié la vous ne l'avez pas cité, donc vous voyez le l'amortissement fiscal que vous avez mis en oeuvre pour essayer dans le secteur privé, j'espère que ça va marcher en dans dans l'océan, j'espère que ça va marcher, c'est un outil, après il y a évidemment les crédits de d'autre n'a vu que quand même les marges de manoeuvre et de n'était pas à la hauteur de tous les besoins à couvrir alors franchement cependant l'un des l'année dernière, vous avez fait un effort particulier pour les Outre-Mer compensée par l'APL accession restaurer, 10 c'était cet argent était nécessaire parce qu'il y a encore beaucoup d'énormes problèmes et si on ne si un des rouages n'est pas au rendez-vous quand il faut combattre l'habitat indigne, hé ben on sait que ça prend du temps, du temps et du temps et on n'y arrive pas, donc je veux bien comprendre que vous ayez des exigences budgétaires qui vous soit donné mais je pense quand même que politiquement comme techniquement. au moins maintenir les crédits de l'habitat indigne serait indispensable car sinon ça veut quand même dire que pour les fictions dans l'Hexagone, on l'a même pas actualisé au report au regard de de l'inflation.

Qui est contre. Il n'est pas adopté, nous allons procéder au vote des crédits de la mission cohésion des territoires figurant à l'état B je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite je mais aux voit les crédits de la mission qui est pour. Qui est contre, ils sont adoptés, j'appelle en discussion : les articles 73 à 75 et les amendements qui sont rattachés pour leur examen aux crédits de la mission cohésion des territoires article 73 Madame Lienemann, vous avez la parole. Nous avons déjà eu l'occasion de parler du FNAP je ne vais pas répéter ce qu'on a dit et notamment sur la ponction qui est faite sur Action logement mais c'est aussi l'occasion, Monsieur le Ministre, de vous interroger sur les intentions du gouvernement concernant Action logement car tous les x mois quand on a besoin de faire quelque chose, on dit, mais on va prendre un de l'argent chez Action logement. D'abord, ça a des limites de l'exercice parce que ce qu'on prend d'un côté on l'enlève de l'autre,

Il y a une 3ème tentation qui serait de baisser encore la ressource parce que je vous rappelle que déjà on finance plus au même taux, ce qu'on appelle le 1 pourcent on en est loin encore baisser et notamment pour un certain nombre d'entreprises, or je rappelle que les PME, beaucoup de besoins en matière de logement bon bref, à la fois l'extinction du prélèvement ou en tout cas sa réduction et la budgétisation du 1 pourcent. Or, plus l'État est en train de faire de la pression à longueur de journée sur Action Logement, pour prendre cet argent, plus on tue ce qui était l'histoire, c'est-à-dire l'histoire du paritarisme entre le patronat et les syndicats pour la gestion de de ce prélèvement pour le logement des salariés ça jamais été un vrai paritarisme, enfin, il y avait l'état d'esprit du paritarisme, alors quand on voit que le paritarisme disparaît de plus en plus, on en a discuté sur la sécurité sociale, on le voit sur l'Unédic. C'est un projet de société qui finit par être menacée donc nous on veut tirer la sonnette d'alarme le 1 pourcent doit rester gérées paritairement prioritairement à en direction des salariés avec une part pour la solidarité nationale, mais pas à coup du sport relèvement permanent, permanent, permanent pour assécher la capacité d'intervention et, par ailleurs, peut-être pour budgétiser si je dis peut-être, c'est que cette tentation est ancienne, tous, le ministre du Logement et je pense que Valérie a dû vivre ça en d'autres temps puisque je crois que c'était à peu près la seule ancienne ministre qui, touché au logement merci il faut ce que je vais vous dire, c'est que tous les ministres ont vu Bercy les menacer de fiscaliser le 1 pourcent donc je sais que vous résistez mais je veux vous dire que le Parlement, en tout cas notre groupe vous accompagne dans cette résistante et vous demande des engagements.

qui est contre, il est adopté l'article 75 Monsieur Gay, vous avez la parole. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, cette prise de parole vaudra explication du vote sur l'amendement de du rapporteur monsieur Dallier. Cet article dans la lignée de l'article 73 via encore puiser dans les réserves de du 1 pourcent logement 500 millions d'euros, c'est pas une petite bagatelle, nous sommes très inquiets de ce mouvement de désengagement de l'État au moment même où celui-ci serait à réaliser des économies sur ces aides personnelles au logement de l'or de 1 milliard 4, nous l'avons dit lors du présent article il est dangereux d'aller piocher au gré des désengagements dans les ressources du 1 pourcent et c'est trop facile et trop injuste, nous rappelons d'ailleurs que le 1 pourcent de finances selon le plan d'investissement volontaire d'ores et déjà pour près de 800 millions d'euros, ce fonds, les ressources du 1 pourcent ne sont pas extensibles, ce gouvernement s'il continue dans cette direction sera confronté à un choix prendre plus pour les aides au logement, donc retirer au fond des aides à la Pierre ou ralentir le rythme de réalisation des plans de rénovation urbaine de l'ANRU, c'est donc une équation impossible que vous nous proposez pour nous, nous refusons de choisir, nous considérons que les ressources du Fonds national des aides au logement doivent évoluer, mais nous pensons à d'autres évolutions possibles que d'aller piocher dans le homme pourcent nous pensons bien sûr à une dotation de l'État renforcé mais également une participation des employeurs, non pas à partir de 20 salariés mais en salariés comme cela prévalait avant des dépenses fiscales inutiles, pourraient également être réorientée nous pensons notamment à toutes les niches fiscales dans l'investissement qui ne profite qu'aux premiers de cordée favorise la rente immobilière, alors que tant de nos concitoyens et concitoyennes ont un besoin vital des appels pour se loger, depuis le début de ce gouvernement, vous rabotez les APL et c'est une obsession, ce qui a conduit à une baisse cumulée de 7 milliards d'euros dans les poches de ceux qui en ont encore moins nous demandons pour notre part une revalorisation nette des APL pour revenir sur toutes ces mesures injustes, nous demandons, parallèlement à l'État de s'engager dans un grand plan de construction pour faire baisser les prix, bref, nous soutiendrons donc l'amendement de notre collègue et rapporteur monsieur Dallier de suppression de cet article en considérant que cet article fragilise l'homme pour logement et crée un risque sur l'avenir des aides au logement, je vous remercie. Merci monsieur Dallier, vous avez la parole pour présenter l'amendement numéro 6. Merci madame la président monsieur le Ministre, mes chers collègues, bon, j'ai déjà évoqué le sujet, à plusieurs reprises, donc je vais être relativement bref, effectivement, monsieur le ministre, cette ponction de 500 millions elle apparaît vraiment comme une mauvaise manière en ce sens que il y a eu beaucoup d'occasions pour le gouvernement, en discuter avec l'ensemble des acteurs du logement social, voilà un accord avait été trouvé et puis à l'été, badaboum, cette ponction de 500 millions tombe alors déjà rien que pour le principe, je pense qu'il faut que le Sénat marque le coup en la supprimant mais il y a une 2ème question Monsieur le Ministre, c'est : quid de l'année prochaine. Parce qu'effectivement, peut se poser la question : 500 millions cette année, ça s'arrête là où 500 millions l'année prochaine et les années suivantes, auquel cas il est absolument certain que les engagements qu'Action Logement a pu prendre, et ils sont nombreux à hauteur de 9 milliards, ils ne pourront pas détenir. Donc je ne peux même pas imaginer que l'idée soit venu à quelqu'un, alors à Bercy ou ailleurs effectivement que ce prélèvement de 500 millions pourraient être pérenne, mais si vous pouvez nous rassurer, Monsieur le Ministre, nous serions très heureux de vous entendre quoi qu'il en soit, je pense que il serait bon que le Sénat vote cet amendement de suppression. Merci, monsieur le Ministre. Merci beaucoup alors plusieurs points, il faudrait vraiment être très clair dans la relation qu'on a avec Action Logement chez déjà préciser les choses, tout à l'heure, suite à une réponse à Madame la sénatrice Guillemot Action logement c'est vraiment et Madame la Ministre, Lienemann, vous connaissez ça très bien, c'est vraiment un partenaire du ministre du Logement, traditionnellement avec Action Logement chaque quinquennat et signé une convention quinquennale qui se représenter en 2017 15 milliards d'euros d'accompagnement des politiques publiques par Action logement en Suisse, de ce que fait Action logement de manière générale, au titre du 1 pourcent logement traditionnel. Et qu'est ce qui s'est passé l'année dernière au regard des disponibilités financières d'Action Logement au regarde, deuxièmement, d'une volonté commune, partagée entre le paritarisme Action logement et l'État, le gouvernement et notamment ma personne, on s'est dit que nous allions mettre en place ce plan d'investissement vous mon, de 9 milliards d'euros, qui va venir s'ajouter au plan quinquennal traditionnel, c'est-à-dire une mesure totalement exceptionnelle qui pour le coup, n'avait jamais eu lieu au au au dans le cadre d'un quinquennat de se dire on peut aller encore plus loin que la convention quinquennale 3ème élément, Madame la Ministre, moi je le dis très clairement, je crois au paritarisme et je peux vous dire même une chose : le paritarisme a montré que ça fonctionnait, y compris dans un dialogue très fort entre les partenaires sociaux et le gouvernement, dans le cas de ce plan d'investissement volontaire parce que le plan d'investissement volontaire, il est pas né comme ça en une soirée, par la volonté de simplement quelques personnes non ce plan d'investissement volontaire c'est des mois de travail entre les partenaires sociaux, le gouvernement pour obtenir et arriver sur ce que nous avons signé en avril dernier, donc moi je crois dans un partenariat très fort entre le gouvernement et Action logement je crois dans une gouvernance paritaire Action Logement je crois donc dans le volet du 1 pourcent logement et je dirais même plus aujourd'hui, on a un objectif qui nous oblige, action logement le gouvernement mais Action logement en 1er lieu c'est que nous avons une convention quinquennale de 15 milliards un plan d'investissement volontaire de 9 milliards, ça fait 24 milliards d'euros de mesures très concrètes d'accompagnement des ménages vis-à-vis du logement ou de la construction qu'il nous faut mettre en oeuvre, donc la priorité aujourd'hui, elle est pas du tout de se poser des questions sur c'est quoi le meilleur des systèmes non, la priorité, elle est de faire en sorte qu'on mette en oeuvre les 24 milliards d'investissements prévus par Action logement, dans le cas des conventions passées avec l'État, alors après il y a la question de cette ponction soulevée par monsieur rapporteur d'alliés. Autant le pif, c'est quelque chose de très nouveau, autant une telle fonction c'est quelque chose que vous avez déjà vu et je m'en félicite pas, non, mais ce que je veux dire c'est un étonne un étonnement généraliser en disant tiens, qu'est ce qui se passe est ce que ça veut dire qu'on va faire la mainmise sur Action Logement non c'est c'est quelque chose qu'on est, et je dirais même plus si tenté si jamais on avait voulu mettre la main mise sur Action Logement, je peux vous dire que jamais on aurait créé un plan d'investissement volontaire de 9 milliards d'euros avec de nouvelles modalités de financement, y compris de la levée de dettes par Action logement dans les prochains mois, évidemment, donc je le confirme, en aucun cas c'est une mainmise de près ou de loin son action logement avec son logement est un partenaire, un partenaire avec qui on a cette politique du logement et un partenaire à qui on a demandé d'accompagner l'effort de réduction de la dépense publique, aussi simplement que cela, comme d'autres et notamment certains de mes prédécesseurs avaient déjà fait tout simplement, mais il faut dire les choses très clairement, voilà comment. On a fait, ne veut absolument pas dire effectivement que c'est un un prélèvement pérenne qui serait instaurée et je crois d'ailleurs que par le passé, on a vu que une ponction ici ne voulait pas dire prélèvements pérenne. Merci Madame Létard. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre évidemment. Je pense que mon groupe va soutenir le l'amendement de Philippe Dallier alors Monsieur le Ministre, complètement convaincu que vous souhaitez un véritable partenariat et vous avez essayé de le construire, dans le cadre du pif du plan d'investissement volontaire avec Action Logement. C'est vrai, les 500 millions. Ils sont quand même très important, il est important de savoir s'ils vont être une fois ponctionner ou régulièrement ponctionné, si ce n'est pas pérenne, c'est une première réponse mais très honnêtement, c'est une inquiétude de la part de tous ceux que de voir ces 500 millions aujourd'hui prélevé ce qu'il faut savoir Monsieur le le le ministre, c'est que, pour y voir un peu plus clair aussi sur le fonctionnement d'Action Logement et être un peu plus en phase et en connexion avec ce qui s'y passe, qu'il serait bon que le décret qui permet de créer le comité des partenaires qui associerait à la réflexion sur l'avenir d'Action Logement sorte rappelez-moi de quand date l'habilitation à légiférer par ordonnances, ça se chiffre en années et donc là, on est loin des 6 mois nécessaires pour sortir des décrets d'application et je pense qu'il aurait beaucoup moins d'incompréhension entre le Parlement, les élus le terrain et vous, monsieur le ministre, si les décrets manquent en on y verrait plus clair et je pense qu'Action Logement a aussi besoin qu'un certain nombre de dispositions sortent rapidement que les emprunts, les prêts qu'il est nécessaire de contracter pour pouvoir pousser encore plus fort, y compris en Outre-mer, qui a besoin d'investissements d'Action Logement, que ce soit la Foncière Logement qui est en lien avec Action Logement pour traiter les questions d'Aubagne, autant de sujets monsieur on vous êtes convaincu mais où on voit aujourd'hui qu'il y a un blocage des commissaires du gouvernement, il faut lever tout ça, il faut surtout qu'il y ait mieux plus de discussion plus d'échanges entre nous et donc, sortez les décrets qui permettront un comité des partenaires de faire le clair avant de rencontrer des problèmes, c'est pourquoi nous voterons l'amendement de monsieur Dallier en attendant et en espérant que vous dites la vérité, mais nous en sommes convaincus mais que vous serez suivi par le reste du gouvernement, merci. Merci, je vais donc mettre pourvoi à l'amendement numéro 6 avec un avis défavorable. Gouvernement qui est alors c'est un amendement au nom de la commission des finances, Qui est contraint, il est adopté, donc, l'article est supprimée et après l'article 75, nous passons à l'amendement 910 présenté par le gouvernement, Monsieur le Ministre. Eh bien écoutez, là aussi, je m'étais engagé à à mettre en oeuvre ses titres participatifs et donc j'ai l'honneur de vous présenter l'amendement du gouvernement qui avait été déposée par certains d'entre vous, mais jugé irrecevable et donc l'amendement a été repris par le gouvernement, qui vise à ouvrir les titres participatifs aux collectivités locales, c'est à dire que les collectivités locales puissent demain souscrire à ces titres participatifs à la fois pour les OPH et à la fois pour les ESH, dont la majorité du capital est détenu par une collectivité locale, je crois que c'était un élément très important, poussé notamment par la Fédération des des OPH en profite pour saluer son président, heureusement qu'il y a beaucoup bataillé là-dessus, mais aussi par la Fédération de de l'USH et le président du monde, je crois que c'est un élément très important de la aussi je m'étais engagé à le faire, ben c'est chose faite. Merci, quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente, monsieur le ministre de la commission n'a pas d'avis, puisqu'elle n'a pas pu discuter l'amendement qui est tombé après sa réunion pour autant à titre personnel, hé bien, je ne peux. Que constate M. chemise que nous allons finir sur une note positive puisque je vais suggérer à mes collègues effectivement d'adopter cet amendement des engagements avaient été pris dans la loi élan certains craignent la finance la financiarisation du secteur du logement social, là on est dans une autre logique, mais qui permet d'apporter des ressources supplémentaires donc autoriser les collectivités territoriales à souscrire, me semble une excellente idée. Merci Madame Lienemann, vous avez la parole. oui, nous sommes favorables à l'esprit de l'amendement, mais je voudrais vous interroger Monsieur le Ministre, parce que j'ai une crainte technique votre amendement, il est, il est valable pour les offices pour les sociétés anonymes d'HLM et les coopératives, or la formulation dans votre amendement les entités, actionnaire de référence, il n'y a pas d'entité actionnaire dans les coopératives, le droit des coopératives ne prévoient pas cela, je vous suggère donc, si vous en étiez d'accord que l'on puisse mettent les collectivités associées par les collectivités locales, mais les collectivités associées dans lequel, soit vous avez les associe coopératif, soit les entités d'actionnaires dans les jets j'insiste un peu sur le le côté technique de l'affaire pour que, en tout cas à la fin de toutes les lectures on soit sûr que la formule la n'exclut pas les coopératives. Oui, monsieur le ministre. Oui, madame la présidente, madame la ministre, effectivement, il faut qu'on rajoute juste un point, on va le travailler dans la navette, il faut qu'on puisse inclure les, en revanche, on ne peut pas changer collectivités majoritaire par. Collectivités associées parce qu'il ne faudrait pas que dans des structures qui ont un capital non mais même, parce qu'il ne faudrait comme justement je suis opposé à la financiarisation, je ne voudrais pas que les rôles soient inversés là, mais comme je suis précisément à la financiarisation, il ne s'agit pas d'ouvrir ces souscriptions de titres dans des structures où vous avez une collectivité qui est simplement actionnaire de l'actionnaire, mais qui n'est pas l'actionnaire majoritaire et donc travaillons le dans la navette pour trouver le bonne rédaction mais effectivement les comme tels que ces rédigé ne sont pas de nom, il faut qu'on trouve la solution. Merci madame Estrosi Sassone. Merci madame la présidente, non, je voudrais également très sincèrement remercier monsieur le ministre, qu'on puisse enfin voter aujourd'hui, donc, que la souscription de ses titres participatifs auprès des collectivités locales, c'est vrai que c'est une demande qui a été formulée, qui est partie de la loi élan puisque je vous le rappelle, que c'était la rédaction du Sénat qui a été adopté lors de la commission mixte paritaire et qui prévoit que les titres participatifs sont émis dans dans des conditions qui sont fixées par le code de commerce qui n'avait jamais été le cas, c'est également une demande très forte qui était portée, plus particulièrement par la Fédération des offices publics de l'habitat, vous avez fait référence au président de la fédération, j'en suis moi-même la la secrétaire générale, c'est la raison pour laquelle, comme d'autres membres ici on avait déposé ces amendements qui ont été déclarés recevables et heureusement que le gouvernement a pu s'en saisir, donc merci, merci d'avoir tenu parole merci puisque vous l'aviez également annoncé au congrès HLM d'ouvrir les titres participatifs à la souscription pour les collectivités locales, c'est effectivement un nouvel outil qui va permettre au logement social dans nos territoires, de pouvoir nous l'espérons, en tout cas se développer assurer plus facilement les investissements, l'équilibre des opérations qui, aujourd'hui, vous le savez, sont de plus en plus compliqué à obtenir du fait de la RLS et puis aussi d'assurer une part de financement du parc ne serait-ce qu'au niveau de l'entretien courant et d'aider également à la restructuration du secteur HLM qui continue, mais ça sera aussi de nature à aller dans ce sens-là et dans le sens de ce que nous avions voté dans le cas de la loi est lente, donc je tiens à vous en remercier.

5 amendements, dont celui du rapporteur de la commission qui était irrecevable, donc je pense que vraiment, là, vous tenez votre promesse que vous avez fait au congrès HLM, donc nous ne pouvons et j'espère que tout le monde votera c'est un amendement et effectivement sur les offices simplement Monsieur le Ministre, je reviens aussi sur ce qu'a dit tout à l'heure sur Action Logement Madame Létard qui rejoint les mêmes questions que je vous ai posée mais qu'il n'y a pas suscité la même indignation que ce que vous avez fait, donc j'espère qu'on aura vite aussi des réponses sur Action Logement. Merci Madame Létard, de la parole. Oui, en 2 mots : donner la position favorable, Monsieur le Ministre de du groupe Union centriste évidemment cette cet amendement va dans le bon sens et permettre aux collectivités d'entrer dans ces souscriptions me paraît être extrêmement nécessaire et utile, dans un contexte où de toute façon, il va falloir trouver des solutions pour accompagner demain politique du logement et nos bailleurs, mettre les collectivités dans cette boucle était une nécessité, en tout cas, permet de rééquilibrer les choses et va dans un bon sens. Merci. Si je vais donc mettre aux voix l'amendement 910 présenté par le gouvernement avec un avis favorable de la commission qui est pour. Qui est contraint, il est adopté, nous terminons en effet sur un point très positif, je vous remercie, je vais suspendre la séance quelques instants pour permettre un changement d'équipe, elle sera ensuite reprise pour l'examen de la mission Agriculture : la séance est suspendue.

la séance est reprise nous poursuivons l'examen des différentes missions : le Sénat va examiner les crédits de la mission Agriculture alimentation forêt et affaires rurales et du compte spécial Développement agricole et rural, la parole est à Alain Houpert, rapporteur spécial de la commission des finances pour 7 minutes

On a trouvé en bonne politique le secret de faire mourir de faim, ce qui en cultivant la terre font vivre les autres cette phrase Monsieur le Ministre, de Voltaire. Mais elle est toujours tristement d'actualité. Le nerf de la guerre, on le sait, l'argent est bien le nerf de la Terre, Monsieur le Ministre, l'est aussi. Et force est de constater que ce budget manque singulièrement de nerf. Si 2019 nous avait déjà confirmé que ce quinquennat ne serait pas celui d'un nouvel élan de la politique agricole française. 2020, trace le sillon d'une réduction programmée des soutiens dans notre agriculture a terriblement besoin. saison Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Par rapport à la loi de programmation pluriannuelle, il manque 58 4 millions d'euros d'autorisations d'engagement et plus de 125 millions d'euros de crédits de paiement, les crédits constate consacré aux aides aux exploitations augmente de 0 4 pourcent c'est-à-dire qu'il baisse en valeur réelle, c'est en pleine contradiction avec les positions que vous dites défendre dans le cadre de la nouvelle PAC des autorisations d'engagement sont il est vrai plus dynamique, je devrais m'en réjouir, il n'en est rien, j'y vois plutôt l'effet des difficultés chroniques de gestion de nos enveloppes agricole certaines lignes sont sous programmé, d'autres sont sûres exécutées, le tout sur fond de correction financière ces dernières années, alors qu'elles étaient frappées de plein fouet par des crises sans précédent nos agriculteurs ont encore dû faire face aux ruptures de paiement des subventions. Vous nous indiquer que pour les dernières campagnes agricoles, le calendrier est revenu à la normale, qu'en est-il, Monsieur le ministre pour les aides des campagnes du début de la programmation. Des retards sur les grandes priorités de la transition agroécologique semble demeurer. Les aides correspondantes nous vaudront-t-elle à nouveau des centaines de millions d'euros de correction financière. Le gouvernement se vantent de nous présenter des projets plus sincère, ce qui, monsieur le Ministre, mes chers collègues, hé bien le moins qu'on l'on puisse demander, mais à la lecture de ce budget, je demande si le mot sincérité hé bien celui qui convient car que propose ce budget. Il propose de laisser enfler la dette de l'État envers la Mutualité sociale agricole, il propose de compter sur la trésorerie du Front national de garantie des risques en agriculture pour financer des indemnisations régler avec retard, quand elles ne sont pas rejetés dans 20 pourcent Il propose de ponctionner la dotation pour dépenses imprévues, afin de financer des dépenses parfaitement prévisible, il propose de retarder la compensation pour les exploitants, exclu du nouveau zonage de l'ICHN, il propose de provisionner les effets du Brexit, il oublie de provisionner les effets du Brexit pour nos pêcheurs enfin il ne prévoit qu'une partie des compensations du TO-DE et je n'oublie pas, monsieur le Ministre, de risque de voir ce budget encore toiser pour récupérer les 45 millions d'euros, dont vous vouliez amputer les moyens d'action des chambres d'agriculture nous avons compris, Monsieur le Ministre, que vous subissez le pilotage de la rue de Bercy, et en tant que sénateur de la Côte-d Or et des grands crus de Bourgogne je ne peut manquer de rappeler que le quartier de Bercy était autrefois celui des marchands de vin et voir le vin se changer en fonctionnaires chargés de finances n'non c'est rien de bon pour notre agriculture et le passé récent est venu confirmer cette craintes. Toutes les initiatives du Sénat. Pour aider nos agriculteurs à relever les défis permanents auxquels il se trouve confrontés ont été systématiquement censuré par des avis défavorables prononcée en première partie de ce projet de loi de finances par les gens de Bercy, instance une insouciance coupable et j'ose le dire le mépris dans lequel est tenu une activité économique, sociétal, environnemental de première importance pour notre pays, ces territoires prospérité et la capacité de la France à diffuser les fruits de son excellence agricole au service de ceux qui ont faim dans le monde, les orientations données à la politique commerciale extérieure traduisent le même mépris et demain Mercosur combien seront les éleveurs sacrifiés sur l'autel d'intérêt plus puissants nous perdons de la production agricole, notre balance commerciale agro-alimentaire se détériore avec une rapidité et une ampleur alarmante et nous regardons ailleurs. Le budget alloué à notre agriculture est non seulement un médecin, un mépris du présent, mais aussi une insulte à l'avenir il ne permettra pas aux agriculteurs de muscler les infrastructures nécessaires à l'adaptation au changement climatique nos campagnes se vident de leurs agriculteurs, on déplore un taux de suicide alarmant dans cette profession : l'emploi agricole : l'emploi agricole baisse les exploitations disparaissent, le pouvoir d'achat de ceux qui se tuent littéralement au travail et critique. Et rien de significatif n'est fait pour soutenir l'installation, les crédits de la dotation aux jeunes agriculteurs augmentent, mais moins que ne recule le soutien fiscal, la presse s'est largement fait écho de l'émotion ressentie par notre président de la République devant le film Les Misérables, qui évoque les quartiers difficiles, j'aurais aimé savoir ce qu'il a pensé du film, au nom de la terre qui retrace l'histoire tragique d'un agriculteur, mais je crains que ce budget ne permettent d'en avoir déjà une vision assez claire j'en finirai avec quelques mots sur le casse d'art pour vous rappeler ce que nous avons déjà indiqué, nous souhaitons ici que la recherche soit pleinement intégrée à notre politique agricole, nous sommes inquiets de voir le compte d'affectation spéciale accumuler des moyens qui n'est pas en mesure de dépenser, selon les critères admis d'évaluation scientifique, nous nous pressentons que bientôt le produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations qui doit alimenter l'innovation agricole sera détourné de son objet ou des usages sans aucun lien avec l'agriculture pour cet ensemble de raisons, la commission des finances, vous propose de ne pas adopter les crédits de la mission mais donne malgré ses inquiétudes, un avis favorable à l'adoption des crédits du CASDAR merci. Merci Monsieur Yannick. Que Botrel, rapporteur spécial de la commission du. Finances, vous avez la parole pour 7 minutes. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues. Chacun le constate le monde agricole exprime en cette période comme peut-être jamais un profond mal- être et pour le moins un profond malaise. Il a été et est encore déstabilisée par des crises à répétition sanitaire climatique industrielle économique. Dans le même temps, il éprouve le sentiment d'une incompréhension de la société à son égard d'une remise en cause par celle-ci du modèle agricole dans son ensemble, quand lui-même considère avoir considérablement évoluer dans ses pratiques et s'être efforcé de les améliorer, dans le sens des attentes sociétales. Il en résulte chez les agriculteurs, un sentiment d'injustice et même d'atteinte à leur dignité. La difficulté qui n'est pas simple à résoudre, j'en conviens, consiste à trouver les moyens de rétablir le dialogue entre la société et ses agriculteurs. Dans le même temps, ce monde agricole est anxieux devant les perspectives d'une PAC qui seraient moins commune et qui redonnent redeviendrait plus national et qui délaisse réelle ambition agricole de l'Europe. Il a d'ailleurs mal vécu les retards de paiement des subventions et des difficultés rencontrées pour exécuter les enveloppes européenne, il ne se sent pas assez soutenu dans cette transformation pour produire mieux il était en droit d'attendre, surtout après les états généraux de l'alimentation, la politique du nouveau monde qu'on lui laissait alors entrevoir. Alors votre projet de budget pour 2020, ne peut que décevoir les attentes car il accompagne mal le présent des agriculteurs et ne prépare pas l'avenir. Notre base de production agricole se défaite inexorablement diminution constante du nombre d'agriculteurs, difficulté d'assurer la transmission des exploitations. Baisse des volumes de production dégradation de notre solde extérieur. Les interventions baisse en valeur réelle, les soutiens à la modernisation des exploitations ne bénéficie qu'à une partie des exploitants, parti minoritaire des exploitants, les moyens de compensation des handicaps naturels ne sont pas revaloriser les aides aux producteurs bio ne le sont pas davantage. Et comptant sur les consommateurs, pour financer une agriculture biologique que le président de la République souhaite voir occuper 15 pourcent de notre surface agricole vous avez renoncé à accorder de nouvelles aides au maintien. De la sorte, le ministère de l'environnement et des agences de l'eau, vont dans ce contexte, devenir les premiers co-financeurs nationaux de l'agriculture biologique. Je relève encore que la situation des aides correspondant en priorité du programme national de développement rural devient particulièrement critique puisque selon leur localisation, des agriculteurs, confrontés aux mêmes charges vont se trouver plus ou moins accompagné. On peut avoir des débats sur la contribution de la montée en gamme de l'agriculture française comme une issue possible à la crise des productions. Mais lorsqu'on engage agriculture en cette voie, il faut lui en assurer les moyens à cet égard la volte-face sur les financements de l'INAO a été désolante et l'empressement du ministère des Finances à réduire la subvention versée pour compenser le maintien des droits INAO serait dérisoire pour le moins si l'on ne savait combien cet établissement devrait faire davantage encore pour assurer l'intégrité des signes de qualité. D'ailleurs, promu comme les instruments préférentiel de la reconquête de nos parts de marché. Permettez-moi, à ce sujet, de m'interroger, devançant un peu la publication d'une analyse que nous devons produire sur la politique de développement du bio ici même au Sénat sur les capacités de l'INAO à suivre les conditions dans lesquelles les exploitants se trouve certifiés par des entreprises privées auxquelles sont déléguées cette mission. Parmi les volte-face que nous a réservé l'examen du budget, l'affaire du prélèvement sur les chambres d'agriculture n'a pas été La Moindre cette question paraît désormais derrière nous. à moins que Bercy n'y revienne, cependant, le Centre national de la propriété forestière qui s'est trouvé concerné lui aussi par la suppression envisagée de l'affectation d'une part de la taxe additionnelle au foncier non bâti. bâti. D'un autre côté, touchés par la réduction d'un 1000000 d'euros de sa subvention pour charges de service public. Cette disposition, monsieur le ministre, inenvisageable au moment même où cet organisme représentant 75 pourcent de la surface forestière française doit d'une part, se restructurer afin de s'adapter à une situation évolutive et d'autre part de plus en plus apporter des réponses techniques aux propriétaires forestiers, ceci à un moment où la situation sanitaire de nos forêts tend à se dégrader particulièrement. je pense en particulier à l'arrestation des scolytes or, la marge de manoeuvre et du CNPF est inexistante en fait toute notre filière forestière subit une crise, une modernisation de Laval s'impose également, si l'on veut. Qu'soit à même de mieux valoriser la ressource de financement ont été annoncées mais sans aucune visibilité dans le cadre du grand plan d'investissement, où en sommes-nous. Par ailleurs, vous avez été destinataire d'un rapport tendance à vouloir fidéliser la partie commerciale de l'activité de l'eau 9 à titre personnel, je vous l'indique, j'exprime de sérieuses réserves sur cette éventualité, quelles sont vos intentions à ce stade, dans un autre domaine, votre gestion des emplois paraît déconcertante : d'un côté vous nous dites recruter plus de 300 ETPT pour accompagner les contrôles aux frontières post-Brexit, mais il semble en l'état que les effectifs actuellement mobilisés par le service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières afin d'assurer les contrôles sanitaires à l'importation sont de 97 postes dans l'hypothèse de l'augmentation projetée, cela représenterait une croissance considérable, je ne sais qu'pensez mais je relève qu'une partie des nouveaux emplois seraient destinés en fait à établir des certificats d'exportation, il n'y aurait donc pas 300 emplois de plus pour les flux d'importation. à ce sujet d'ailleurs, d'aucuns disent qu'il en faudrait bien davantage afin de garantir la conformité des importations aux normes appliquées à nos propres productions. Sur ce sujet aussi, nous souhaiterions entendre votre réponse, ce qui est acquis, c'est que malgré la montée des périls sanitaires déjà considérable malgré des trous dans la raquette constatée par un autre rapport du Sénat, la politique de sécurité sanitaire ne se verra doté d'aucun poste supplémentaire de même vous allez rendre 130 emplois au titre du programme de 115 alors que les engagements de crédits nécessaires pour achever la programmation actuelle de la PAC sont encore fortes élevé et que des paiements sont loin d'être achevée. Ceci ne sera pas, il faut le crâne de nature à fluidifier le traitement des dossiers par l'administration, ce budget que l'on peut qualifier sans conteste de reconduction ou de prolongement du précédent ne traduit pas de projet politique digne des enjeux dans ces conditions, vous n'avez pas été surpris, monsieur le ministre, d'apprendre le vote négatif émis très majoritairement leurs examens de la mission Agriculture par la commission des finances du Sénat vote qui, en l'absence de modifications substantielles devrait, en toute hypothèse être réitéré aujourd'hui.

madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais commencer en vous faisant part d'une satisfaction, il est vrai que dans le budget de l'agriculture cherchait des satisfactions, c'est quelque chose de difficile, d'autant plus qu'aujourd'hui dans l'agriculture, on arrive à se satisfaire quand ne rien ne bouge, parce qu'à un moment quand eux cela bouge c'est plutôt négatif, je me réjouis du revirement du gouvernement sur la question de la baisse du financement des chambres d'agriculture et de leur régionalisation cette décision avait un bilan très négatif, pas d'économies pour l'État : pas de baisse de charges significatives pour les agriculteurs et une dizaine et une déstabilisation majeure des chambres départementales d'agriculture au moment même où l'État leur confient de plus en plus de missions, c'était une erreur stratégique et il faut se réjouir du maintien de cette taxe une fausse information ensuite le budget de la mission ne se donne pas les moyens d'aider notre agriculteur notre agriculture agrandir en affichage, le budget de la mission qui nous est présentée, après un passage à l'Assemblée nationale nal augmente, mais il leur. mais à y regarder de plus près, l'essentiel des mouvements provient de du réengagement habituel des contrats pluriannuels portant sur les mesures agro-environnementales et climatiques, le MAEC, le reste des décisions sont subi Brexit évolution de la réglementation européenne sur la politique sanitaire correction budgétaire, compte tenu de la budgétisation peu sincère de la loi de finances de 2019 finalement les seules mesures décidées par le ministère pour l'agriculture cette année sont des crédits supplémentaires pour financer des dépenses informatiques et et préparer le recensement agricole à hauteur de plus de 25 millions d'euros, on est loin des Budgets annonçant un grand plan au bénéfice des agriculteurs, pire encore, 7 E hausse de crédit est compensée par une baisse de la réserve pour aller à des agriculteurs de 25 millions d'euros, monsieur le Ministre, ce n'est pas de ce budget de gestion boutiquière dans l'agriculture a besoin, les agriculteurs sont dans la rue car ils veulent avoir un cap clair : ils veulent éviter la politique du en même temps, en d'autres termes, ils veulent un budget visionnaire, or rien n'est prévu pour l'innovation en agriculture pour le développement du numérique pour adapter les agriculteurs au changement climatique et aux risques climatiques auxquels ils sont exposés. Des équipements déjà commercialisé aujourd'hui permettent de réduire à très court terme, l'usage des produits phytosanitaires de 30 à 90 pourcent ces solutions sont pour l'instant très onéreuse : pourquoi l'État ne pourrait-il pas aidé à l'acquisition, individuelle ou collective de ces derniers au regard de leurs effets tant sur l'environnement que sur la compétitivité de notre agriculture, notre sentiment est que l'État en demande toujours plus aux agriculteurs sans jamais lui-même se demander ce qu'il peut faire pour les accompagner, le rapport sur la sortie du glyphosate de nos collègues députés et des répliques des députés en marche le démontre très bien, c'est pourquoi la commission des affaires économiques, a émis un avis défavorable sur les crédits de la mission et vous appelle toutefois en cohérence et pour soutenir l'innovation en agriculture a adopté les crédits du CASDAR merci. La parole est maintenant à Madame Françoise Férat, rapport. Alors pour avis de la commission des affaires économiques pour 3 minutes chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons déploré l'année dernière, un budget qui ne prenait pas la mesure de la détresse agricole en reculant considérablement les crédits de la mission en un an, l'accuse ressenti par le monde agricole s'est faite plus violente : à quand un grand plan agricole, or le budget que vous présentez n'a pas évolué, il ne constitue pas une réponse claire et satisfaisante aux demandes de nos paysans qui sont plongés dans une grande détresse où on est on sur les revenus, la PAC, la réduction des normes, l'export, l'aide au changement ou même pas que l'année dernière, la fréquence des manifestations dénoncent cette inertie, si aucun incident n'est à déplorer, pour l'instant, cela pourrait ne pas durer, et c'est pourquoi il faut agir en fixant un cap rappelons encore et toujours que nos agriculteurs évoluent dans un marché mondial, n'oublions pas l'impératif de compétitivité et je m'étonne Monsieur le ministre, à cet égard le refus du gouvernement de pérenniser le TO-DE dès cette année, allez-vous enfin nous entendre. La France a un système de sécurité sanitaire d'excellence sans doute le meilleur du monde et les paysans en sont les principaux acteurs de cette politique exemplaire, or ce système est confrontée à de pression particulière qui me préoccupe la première pression concerne les risques pesant sur les produits alimentaires que nous importons ne le répéterons jamais assez, les Français consomment de plus en plus de produits alimentaires importés qui n'ont sans doute pas les mêmes garanties en matière de sécurité sanitaire que nos produits, il importe de renforcer les contrôles inopinés pour accroître notre sécurité alimentaire et garantir une concurrence loyale avec nos agriculteurs, je rappelle que les Français dépensent 0 virgule 3 euros par habitant et par an pour les inspections sanitaires sur les produits destinés à la consommation pendant ce temps 7 1,5 euros aux Pays-Bas 1 virgule 7 heures Belgique et 2 4 au Danemark, ces chiffres sont éloquents et se passe de commentaires, la seconde pression s'exerce sur ce les vétérinaires de nos territoires ruraux dès l'année dernière nous alertons sur le risque de voir apparaître des déserts, vétérinaire à l'image, ils étaient déserts médicaux, la tendance se poursuit cette année, faute d'une action résolue du ministère, le nombre annuel de recrutement stagne depuis 2016 avec des spécialisations de plus en plus tournée vers les animaux de compagnie, on constate également un recours accru à des vétérinaires formés à l'étranger, cela représente 43 pourcent des primo-inscrits à l'Ordre national, chaque année, on ne peut pas s'engager à aider nos éleveurs tout en les privant de la relation privilégiée qu'ils ont avec leur vétérinaire, des solutions existent comme le stage tutoré 95 pourcent des étudiants en ayant bénéficié se sont installés dans les zones rurales au bénéfice des animaux d'élevage

Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, le résultat de nos travaux, votre budget ne permettra pas de répondre aux nombreuses attentes des agriculteurs, il témoigne d'ailleurs d'une vision à court terme, à laquelle nous ne pouvons pas souscrire ce que démontre 3 décisions contenues dans ce budget, la première concerne la gestion des risques climatiques, la réserve pour risques pour aléas climatiques et cette année, une nouvelle fois, réduite de 25 millions d'euros, même avec le renforcement de la solution assurantielle, c'est une erreur, car comme l'a démontré le rapport de Nicole Bonnefoy, adopté à l'unanimité de la mission d'information sur les risques climatiques, les agriculteurs vont être exposées à des sécheresses plus nombreux et plus violente, tout comme dit tempête de grêle et de pluie plus violentes et fréquentes et ses effets sont déjà perceptibles, les sécheresses des 2 dernières années, le démontre et les pluies de ce week-end dans le sud de la France le confirme au fond cette réserve depuis sa création n'est qu'une assurance de l'État contre son propre dysfonctionnements depuis sa création, la réserve servi à 70 pourcent à financer les apurements communautaires à l'Union européenne, on est très loin, nous le voyons bien d'une vision stratégique destiné à permettre une meilleure prévention et une meilleure indemnisation des agriculteurs face aux risques climatiques auxquels ils sont exposés la seconde concerne la politique forestière Yannick Botrel a démontré tout à l'heure, très clairement, les crédits de la forêt reste à un niveau bas et en plus ils baissent de 2 et demi pourcent la forêt est surtout confronté à une crise sanitaire majeure or pendant que l'Allemagne consacre 800 millions d'euros supplémentaires pour aider sa forêt, face à la crise, vous avez annoncé un plan scolytes seulement de 16 millions d'euros et ses 16 millions d'euros, il y en a 8 ou 6 6 millions d'euros qui vont aller au transport pour sortir les bois et le budget réduit les dotations au Centre national des propriétés foncières, là encore, la cohérence de la politique est loin d'être rétabli la 3ème concerne les frais le le fonds d'indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques, le Sénat a adopté une proposition de loi visant à créer un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques en 2018 dans une version remaniée ciblée sur les maladies professionnelles lors de la loi Egalim la création du fonds a été voté à l'unanimité. Le gouvernement après l'avoir longtemps repoussé acté à l'article 46 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, la création du fonds, mais elle a la lecture ces propositions gouvernementales la solution proposée n'est pas satisfaisante surtout pourquoi l'État devrait devrait-il être le seul à ne pas participer au financement du fonds d'indemnisation, c'est sous sa responsabilité que sont délivrer les autorisations de mise sur le marché des produits, il est donc normal qu'il assume cette responsabilité, en participant à l'indemnisation des victimes agricole de ces produits sur ces 3 points, je constate trop désaccord profond avec les propositions défendues régulièrement au Sénat, c'est pourquoi la commission des affaires économiques, vous invite à rejeter les crédits de cette mission. Merci, merci. Dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribués à chaque groupe pour chaque discussion qu'on prend le temps d'intervention en général et celui de l'explication de vote le gouvernement dispose au total de 20 minutes pour intervenir et je vous indique également que nous suspendrons la séance à 20 heures la parole est maintenant à monsieur Henri Cabanel pour le groupe RDSE pour 6 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues. La semaine dernière, les agriculteurs ont une nouvelle fois manifesté leur colère. Malgré un niveau de récolte globale même bord Rennes 2019, une majorité d'exploitants demeure dans une situation préoccupante conduisent comme beaucoup d'entre eux a renoncé ou bien pire puisque les derniers chiffres de la Mutualité sociale agricole communiqué septembre dernier indique qu'en 2015, il y a eu 605 suicides, ce chiffre est resté supportable aujourd'hui un suicide par jour, on le sait, l'agriculture fait face à de grands défis, la compétitivité et ça essayer pour maintenir le revenu agricole et la transition écologique encore plus incontournable pour répondre aux attentes et les consommateurs et aux impératifs environnementaux. Les orateurs précédents le souligner, le projet de loi de filage pour 2020 reste stable et manque d'ambition, malgré tout, il ne reflète pas la totalité des soutiens à l'agriculture puisque la PAC apportera de son côté 9,7 milliards d'euros, comme chaque année, à cet égard, mon groupe compte beaucoup sur vous, monsieur le ministre, pour que soit préservé ses moyennes dans le cas de la négociation d'un cours du cadre financier pluriannuel. Le défi de la compétitivité que je souhaitais évoquer et sans cesse à relever les derniers comptes de résultats de l'agriculture font apparaître une embellie en 2018, il faut toutefois reconnaître qu'elle est plutôt conjoncturel que structurel, car la loi Egalim qui devait aboutir au partage de valeur n'est toujours pas au rendez-vous avec le groupe de suivi de la commission des affaires économiques, nous avons auditionné beaucoup d'entreprises qui souffrent notamment du seuil de revente à perte car il défavorise et met en péril la pérennité de certaines, par exemple celles qui ont des produits saisonniers une nous fait le foie, les impacts donc pas assez était mesurer la valeur ajoutée nette de la branche a enregistré une hausse de 22,7 milliards d'euros, mais là le même temps, la chute du taux d'investissement des exploitations agricoles se poursuit une évolution qui risque d'impacter la productivité alors que c'est une condition de la compétitivité du secteur agricole, aussi il est important de conforter tous les outils qui, au sein de ce budget se destine à la à la à l'adaptation des exploitations, je pense par exemple au plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles, dont les crédits augmentent de 5,7 millions d'euros, ce plan mérite cependant d'être reconfigurée pour davantage cibler les entreprises agricoles, notamment dans l'aide à l'innovation pour les appareils de traitement confiné par exemple, qui permettent de réduire de 40 pourcent des intrants mais qui reste très coûteux à l'achat au delà de l'adaptation des structures, le secteur agricole d'anciens doit faire aussi face à des contraintes particulières dont il faut réduire les impacts négatifs, par exemple, mon groupe est attentif aux dotations prévues pour financer l'indemnité compensatoire d'handicap qui stagne alors qu'il faudrait accompagner des exploitants sortie du nouveau zonage dont le nombre est estimé à 3800. Je rappellerai aussi au titre des crédits de paiement prévus pour couvrir la compensation des zones l'exonération de cotisations sociales, notre vigilance sur le dispositif TODE on se souvient, il a été entame menacés de suppression pour le secteur agricole, puis finalement redéfinies dans le cadre du projet de loi de finale, chemin de la Sécurité sociale pour 2019, monsieur le ministre, beaucoup d'entreprises ont été écartés du système, car vous avez souhaité passer de 1,5 à SMIC à 1 virgule 2 mais qu'avez-vous prévu pour 2021. Avez-vous étudié l'impact sur les entreprises, si cette mesure est abandonnée, ce nouveau mandat bornage pourrait aboutir à une perte de 26 millions d'euros qui fragiliserait encore plus l'emploi saisonnier. Par ailleurs, je souhaite aussi évoquer la pêche maritime les crédits consacrés à ce secteur Sonntag, hausse de 2,4 pourcent par rapport au budget 2000 19 mai 52 millions d'euros sont prévus pour le désarmement des bateaux dans la fin d'une activité économique en marge de cette évolution budgétaire, je tiens à relayer l'inquiétude à l'approche du Brexit des pêcheurs français qui évolue dans les eaux anglaises en se souviennent de la guerre franco-anglaise autour de la coquille Saint-Jacques, les eaux anglaises reprennent de 50 pourcent de l'activité des fileyeurs jusqu'à 5 pourcent pour certains chalutiers, avez-vous Monsieur le Ministre, des éléments sur ce dossier, de nature à rassurer les professions la profession même si je comprends bien que cela n'a, nature de la sortie du Royaume-Uni, les règles seront différentes, je rappelle en tout cas, qu'il s'agit de l'avenir de milliers d'emplois amer et de nombreuses autres qui en découlent à terre. Comme je l'ai dit au début de mon intervention, il est également question de poursuivent l'encouragement à l'agroécologie à travers ce budget dans cette perspective, nous observons avec satisfaction l'enveloppe de 128 de 30 millions d'euros en crédits de paiement en faveur des mesures agro-environnementales et climatiques, soit une hausse de 23,7 pourcent des crédits pour 2020, ces mesures sont indispensables pour la déclinaison des directives Natura 2000 et car les accompagnent les exploitations agricoles vers des pratiques plus respectueuses, je le répète aussi : il n'y aura pas de transition écologique ça nos agriculteurs. Je dirais justement sur les moyens consacrés à la forêt, la France y dispose n'est-ce pas ce forestier considérable, un atout à la fois économique et et environnemental qu'il faut davantage valoriser, je veux relayer l'inquiétude des salariés de l'ONF il faudra co-construire avec les éventuelles mutations avec toutes les parties prenantes. Enfin, vous le savez, Monsieur le Ministre, le Sénat s'intéresse de près au pastoralisme il y a traversé un groupe de suivi présidé par notre collègue Patricia Richaud le RDSE particulièrement attentifs à la politique de lutte contre la prédation qui est abondé ici de 6 millions d'euros, il est bénéfique, d'augmenter les débats et ce public pour indemniser les éleveurs qui se une véritable situation de détresse. Mais c'est surtout sur la baisse de cette prédation qu'il faut agir car les bergers veulent le voir cesser les attaques qu'elles viennent du loup de l'ours ou du lynx enfin une actualité qui vient de tomber : le président Trump annonce vouloir surtaxer des produits français comme le fromage, le sac à main, le parfum ou le champagne, que faire face à cette surenchère politique. Parce qu'il portait globalement une stabilisation des moyens mais qui dresse à dessous d'une ambition que la France devrait témoigner à son agriculture, la majorité du groupe RDSE s'abstiendra sur ce budget. Merci. Nous passons maintenant.

Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le gouvernement nous demande d'approuver la mission Agriculture alimentation forêt a fait rural du projet de loi de finances 2020 et ainsi et l'ouverture de 3,0 1 milliard d'euros en autorisations d'engagement et de 2 96 milliards d'euros en crédits de paiement, soit respectivement 6,3 pourcent et 1,2 pourcent de plus que pour l'exercice actuel, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui face à un budget sincère dont le périmètre n'a pas changé par rapport à l'année dernière et qui approfondit des priorités du gouvernement et de notre majorité en préservant les moyens actuels et en préparant l'avenir et la transition agro-écologique l'agriculture subit de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique, 2 années de sécheresse ont déjà beaucoup pénalisés une partie de la profession, l'augmentation des phénomènes climatologiques extrêmes couplé à l'apparition d'organismes nuisibles et de maladies qu'il faudra gérer avec de moins en moins de produits phytosanitaires va ça va frapper durement les rendements agricole. Nous devons prendre en compte les 6 nouveaux enjeux et menaces ce que prévoit le projet de loi 2020, qui consacre une large partie de la mission à des mesures agro-environnementales et climatiques

aussi le volet agricole du grand plan d'investissement bénéficie d'une contribution de 244 millions l'enveloppe des mesures agro-envie normes environnementales et climatiques et des aides bio s'élèvera à 128 millions d'euros, ce qui représente une augmentation de près de 25 pourcent par rapport à 2019 rappelons également que le montant du fonds de Russes de structuration à venir bio a doublé, passant de 4 à 8 millions, il convient de saluer la prudence et la sincérité du projet de loi de finances dans la provision pour aléas créée en 2018 sera reconduite à hauteur de 174,8 millions d'euros, elle va permettre notamment de faire face aux refus d'apurement de la Commission européenne comme a rappelé : Monsieur le ministre en audition, bien que la Réserve diminue, le sujet n'est pas là l'année dernière 200 millions d'euros avaient été alloués, or le ministère a dépassé en réalité près de 300 millions d'euros, à mon sens, ce n'est pas au contribuable français de payer les aides versées aux agriculteurs en compensation des aléas, comme le demandent les principaux syndicats agricoles, nous devons créer une assurance facultative généralisée et mutualiser qui soit accessible aux agriculteurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui le programme 206 Sécurité, sécurité sanitaire de l'alimentation sanitaire de l'alimentation est également en très légère hausse, ce qui permettra de maintenir un haut niveau de vigilance, il est essentiel pour les débouchés de notre agriculture, de préserver la qualification sanitaire de l'élevage français, j'aimerais attirer l'attention, chers collègues, Monsieur le Ministre, sur la question du bien-être animal qui fait l'objet aujourd'hui d'une réelle préoccupation du public, nous sommes dans une situation aujourd'hui où les objectifs sont insuffisants pour assurer la bonne application des règles dans les abattoirs, un effort, même minime, ramené à l'ensemble du programme 206 contribuerait nettement amélioré la situation, aussi je voulais saluer l'engagement de Monsieur le Ministre d'allouer plus de ressources au médiateur commerciale prévue par la loi Egalim afin de renforcer le contrôle des relations commerciales que nous surveillerons de près cette année. Mes chers collègues, nous sommes face aujourd'hui à une profession à bout de souffle pour permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur activité, nous devons tous ensemble prendre la mesure des nouvelles menaces et étudier de nouvelles pistes, la possibilité d'accroître nos exportations, notamment concernant la filière bovine vers la Chine est aujourd'hui une ferme une formidable opportunité pour un secteur d'activité, durement touchée par la sécheresse, je ne peux que déplorer le faible tonnage exporté en Chine qui reste ridicule face à la demande chinoise, nous avons aujourd'hui en France l'offre adaptée qui répond aux besoins des Chinois, sur le sur votre attention sur l'opportunité pour les exploitants agricoles de bénéficier de complément de revenus, notamment par le développement de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles aujourd'hui les freins réglementaires et le manque d'incitations fiscales tend à décourager des petites structures, dont les agriculteurs et les éleveurs, mes chers collègues, notre profession doit faire face à des bouleversements structurels qui devront répondre aux nouvelles attentes de la société à la menace du dérèglement climatique et à la concurrence internationale, nous devons innover et réinventer nos organisations et nos modes de production, dans un contexte d'agribashing nous avons eu l'année dernière 12000 nouvelles installations de jeunes agriculteurs et un quasi-renouvellement de nos filières, ce qui démontre bien que notre profession millénaire reste attractive, mes chers collègues, nous devons continuer et permettent aux agriculteurs de vivre dignement de leur activité, je vous invite à voter les crédits de la mission, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant à Madame Cécile Cukierman. Pour le groupe C, C, E et vous avez 6 minutes. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, produire mieux, ne plus utiliser de pesticides préserver la santé du consommateur, protéger la biodiversité ne pas nuire aux voisins avec des animaux bruyants ou un épandage trop odorant, telles sont les nouvelles injonctions que l'on ordonne aux agriculteurs autrefois professionnelles les plus appréciées de nos concitoyens, les agriculteurs font face aujourd'hui à un désamour qui conduit parfois jusqu'à ce que l'on appelle aujourd'hui l'agribashing évoluant dans un milieu toujours plus concurrentiel ou leur travail ne leur permet plus de vivre car les prix ne sont plus garantis, il nous faut agir envers ces hommes envers ces femmes qui assurent depuis des décennies l'autosuffisance alimentaire de notre pays, et ont participé à élever à élever l'espérance de vie de l'ensemble de la population, il ne s'agit pas de nier l'impact de l'Agriculture, sur l'environnement, la nécessité d'une transition vers un modèle plus vertueux, mais le procès permanent, permanent à l'égard d'une profession en difficulté et qui évolue, n'est pas acceptable le monde agricole est en évolution perpétuelle des modes de production ne cesse d'évoluer depuis les années 60, oui, le métier d'agriculteur n'est plus celui d'il y a 50 ans, l'agriculteur est aujourd'hui plus formés, il doit de plus en plus devenir gestionnaire comptable administrateur et bientôt ingénieur numérique ou robotique dans l'agriculture devient le débouché d'un marché technologique en pleine expansion, faut-il rappeler ici que pour répondre aux exigences de production mais aussi aux exigences sanitaires et environnementales, les agriculteurs ont dû s'endetter à des taux parfois prohibitifs, or ils sont aujourd'hui en première ligne du changement climatique, victime des sécheresses à répétition des inondés, des inondations et de toute autre épisode climatique fragilisant fortement leurs revenus d'une année sur l'autre et navré de vous le dire, ce n'est pas une légère hausse de la mission Agriculture après des années de pénuries qui aidera les agriculteurs à survivre à cette crise désormais structurelle, il est donc temps de reconnaître, comme cela a été fait au siècle dernier mais aussi lors des négociations des accords du GATT, que les spécificités économiques, sociologiques, de l'agriculture, justifie une intervention volontariste des pouvoirs publics, nous devons protéger notre modèle agricole contre les effets de la libéralisation des marchés du rapport de force indécent et déséquilibrée entre la grande distribution et l'agro-industrie, comment ne pas entendre qu'il est impératif de garantir à l'agriculteur les juste prix nécessaires à sa survie, monsieur le ministre, il est temps de l'Euro, connaître les objectifs des états généraux ne sont pas atteints ainsi les prix payés aux producteurs ont continué de baisser, et dans le même temps, les prix aux consommateurs eux ont augmenté, la grande distribution a gagné plus de 800 millions d'euros sur le dos des producteurs et des consommateurs depuis que cette loi a été promulguée, la régulation des marchés agricoles et les politiques agricoles ne doivent plus être perçus comme des entorses au principe de la concurrence libre et non faussée, cela n'est plus soutenable économiquement, ni écologiquement, nous devons donc revenir sur les accords de libre-échange que nous avons ratifié et renoncer à ceux qui sont encore en cours, tels que le Ceta qui, mais nous l'avons déjà dit ici et à plusieurs voix ne va pas dans le sens de l'histoire qui est contradictoire avec ce que ce que vous semblez pourtant, Monsieur le Ministre dire vouloir défendre ratifier ce genre d'accord entraîne et entraînera, nous le savons, une concurrence déloyale avec d'énormes, donc des prix différents, une traçabilité proche du néant, avec la possibilité de devoir faire face à de nouveaux scandales sanitaires, je ne reviens pas ici sur le scandale des faux steaks et le rapport de mon collègue Fabien qui attend d'ailleurs toujours Monsieur le Ministre, de pouvoir être reçus pour échanger réellement sur ces problématiques : sanitaires et de distribution alimentaire dans notre pays,

quelle agriculture voulons nous voulons-nous d'un modèle fortement, constate concentré réduit à 100000 exploitations tourné vers l'agro-industrie et du bio pour les plus aisés ou voulons-nous préserver et encourager ces exploitations familiales qui produisent elles aussi pour le marché, mais qui crée aussi des richesses immatérielles peu marchande une richesse collective au groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, nous faisons le choix d'un modèle d'exploitation familiale qui doit être préservé et d'une agro-écologie comme nouveau modèle, en somme, le choix d'une agriculture saine pour tous une agriculture saine sans fracture sociale sans fracture territoriale une agriculture qui permette à tous ceux qui travaillent, de pouvoir en vivre et à tous la possibilité de se nourrir sainement à un coût abordable sa décision : nous devons bien évidemment l'accompagner, et c'est le sens des pouvoirs publics afin d'exiger les mêmes règles phytosanitaires que celles imposées dans notre pays en matière d'importation, c'est de cela dont ont besoin nos agriculteurs dès à présent, et pour les années à venir ainsi que l'ensemble de nos consommateurs de notre pays, finalement, c'est un défi national auquel il nous appartient collectivement de répondre à la mission en l'état, ne le permettra pas, nous ne voterons pas cette mission.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'agriculture rencontrent de grandes difficultés, cette crise est à la fois économique pour certaines filières de compétitivité mais surtout et aussi morale, en effet, les agriculteurs sont aujourd'hui dans le doute, ils ne savent pas plus que la société et les pouvoirs publics attendent de cette colère ce mal-être, c'est une, c'est une nouvelle fois exprimé la semaine dernière dans les rues de la capitale, les agriculteurs sont pourtant les garants de notre souveraineté alimentaire, il joue un rôle essentiel pour la préservation et la gestion de la ressource en eau, il concourt au maintien de la biodiversité, il contribue aussi à la transition énergétique au travers les biocarburants, enfin, il participe au stockage du carbone levier important quand on connaît les enjeux du réchauffement climatique, la liste bien sûr pourrait être encore être plus longue, pourtant, ils sont 5 jours la cible d'attaques directes ou indirectes, communément appelée agribashing les états généraux de l'alimentation se sont tenus il y a environ 1 2 en un peu plus 2 ans ils ont suscité beaucoup d'espoir et dans cette concertation a vu le jour, la loi Egalim qui aujourd'hui tarde à porter ses fruits et c'est dans ce contexte difficile que s'inscrit votre action et votre budget néanmoins le budget de la mission Agriculture alimentation forêt et affaires rurales que nous examinons aujourd'hui est en légère hausse et par rapport à celui de l'année 2019, et je ne peux que m'en réjouir, si toutefois nous constatons qu'il ne retrouve pas son niveau de 2018 le budget 2020 maintient les équilibres et s'inscrit dans la lignée des années précédentes, malheureusement il nous semble pas à la hauteur des enjeux et des attentes qu'invite à telle contexte dans un 1er temps, je souhaite m'attarder sur le budget de la forêt, monsieur le Ministre, j'ai eu l'occasion de vous interpeller sur la crise sanitaire de la forêt française la semaine dernière et je regrette que cette cette politique soit encore le parent pauvre

268 millions d'euros se mue budget nous paraît manquer d'ambition, et pourtant la forêt doit faire face à un niveau de risque jamais atteint, réchauffement climatique sécheresses successives et multiplication des attaques pathogènes

le CNPF et ses antennes régionales dont sont les que sont les CRPF jouent un rôle essentiel et primordial pour l'accompagnement au quotidien des forestiers, une baisse de leurs moyens seraient donc en totale contradiction avec les les objectifs que vous visez, d'une politique en faveur de la forêt, concernant plus spécifiquement l'agriculture l'agriculture pour la 3ème année consécutive, la dotation aux aléas, a poursuivi une baisse, mais si elle est toutefois beaucoup moins importante que les années antérieures, elle a été réduit de de 25 millions d'euros. Et ce alors même que les agriculteurs n'ont jamais autant subi de été exposés aux aléas et aux risques climatiques dont nous appelons donc de nos voeux à une réforme, mais je sais que vous y travailler profondeur et un renforcement des outils assurantiels du régime des calamités agricoles, je veux aussi revenir sur le budget des chambres d'agriculture, initialement, donc le projet de budget 2020 ambitionné de revoir profondément leur fonctionnement, il prévoyait d'une part, une baisse de 45 millions d'euros de la TFPNB, B et d'autre part, un versement de cette taxe aux Chambres régionales cette régionalisation à marche forcée a été mal accueillie et revenons à anéantir donc le financement des des chambres départementales, je me réjouis que vous que que le gouvernement et votre action, vous soyez donc revenu sur ce dispositif, les chambres d'agriculture sont un partenaire essentiel pour l'accompagnement des agriculteurs et de l'agriculture, il faut donc les mobiliser plutôt que les affaiblir, enfin, je me réjouis que vous ayez aussi maintenu les crédits du castor autre levier important pour le développement et l'innovation, pour terminer, je veux m'attarder quelques instants sur le défi du renouvellement des générations, aujourd'hui, un agriculteur sur 2 à plus de 50 ans 8000 800000 hectares de Terres agricoles ont disparu en 10 ans, soit 4 exploitations par jour, il est absolument indispensable d'assurer la protection des Terres agricoles car plus généralement car plus généralement derrière ceci il y a une véritable question d'avenir de notre territoire aujourd'hui les outils de régulation sont affaiblis par le développement de nouveaux modes de portage foncier une nouvelle valeur foncière doit donc au plus vite voir le jour afin d'enrayer ce phénomène et de faciliter l'accès du foncier aux jeunes générations, dans un contexte de construction du budget de l'État extrêmement contraint, le budget de l'agriculture et d'une relative stabilité, ce qui pourrait à la fois à première vue donc nous satisfaire, d'un au regard des enjeux agricoles en matière d'innovation, de recherche et des nécessités d'investissement pour la forêt, ce budget ne nous semble pas à la hauteur des besoins il est certes stable mais une ne peur mais pas suffisamment de répondre au malaise des secteurs en crise ni de rassurer nos agriculteurs, il n'investit pas sur suffisamment dans l'avenir, mais je sais combien la l'exercice est néanmoins difficile notre groupe donc votera les budget du quasar et s'abstiendra sur les crédits de la mission Agriculture. Merci, je vais suite. La séance, elle sera reprise à 21 heures 30 pour la suite de l'examen de ces. Mission : la séance est suspendue.